La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, nous n'avons pas reçu d'observation, il en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sur les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public solennel sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que ce scrutin s'effectue depuis les terminaux de vote, je vous invite donc, mes chers collègues, à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote. Et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement en l'insérant dans votre terminal de vote. Et en cas de difficultés, vous pouvez vous rapprocher des huissiers qui faciliteront. Je vois que ça suscite à certains moments de contrôle qui démontre que mon annonce n'est pas inutile. Mais avant de passer au vote. Je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote, je rappelle la règle 7 minutes pour chaque groupe, 3 minutes pour un sénateur n'appartenant à aucun groupe et je vais commencer par par donner la parole à Jérôme Durain pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission chers collègues. Permettez-moi de débuter en salant le travail, le travail des deux co-rapporteurs s'il nous arrive encore fréquemment de constater des désaccords, ils sont toujours exprimé avec une cordialité certaines ce constat je l'élargirait Monsieur le Ministre, avec qui nous constatons encore plus fréquemment des désaccords et notre groupe, nous sommes sensibles au fait qu'un ministre prenne le temps de nous répondre, même si nous préférions bien sûr qu'il dise oui à nos amendements, je vais commencer par les éléments dont nous regrettons qu'ils ne soient pas présents dans ce projet de loi. Plusieurs sénateurs de notre groupe ont regretté de ne pas trouver suffisamment de contenus dédiés aux préfectures et à la présence de l'État sur le terrain, en dehors de la sécurité, alors que votre gouvernement communique sur la réouverture bienvenue de sous-préfecture, on aurait pu attendre du ministère de l'Intérieur davantage d'ambition sur l'incarnation de l'État au quotidien. Il y a une autre grande absente ou une quasi absente de ce projet de loi, c'est la réforme de la police judiciaire, les mentions qui en sont faites dans le rapport annexé sont succinctes et même si nous en avons débattu avec passion, mardi dernier, dans cet hémicycle, nous savons tous que le destin de cette réforme ne se joue pas ici la balle est donc dans votre camp, monsieur le Ministre pour réconcilier votre ministère avec ses propres troupes, ainsi qu'avec les représentants du monde judiciaire qui redoutent une atteinte à la séparation des pouvoirs, nous connaissons tous votre revendication d'une certaine fibre sociale, monsieur Darmanin, je pense toutefois que vous ne devriez pas la cultiver au point d'ajouter des manifestations de policiers aux manifestations de salariés pour faire rentrer la PJ dans les commissariats, c'est comme pour faire cesser les blocages dans les dépôts, il faudra négocier. Que j'ai évoqué rapidement le monde de la justice, je crois qu'à droite comme à gauche, nous regrettons de ne pas parvenir à aborder les questions de sécurité et de justice dans un même élan. Nous faisons tous en lien entre les problèmes de sécurité et la réponse pénale. Nous constatons les occasionnels, tensions entre magistrats et policiers, il nous manque la stéréophonie cher au rapporteur Daubresse ce regret d'ailleurs vise tout autant le Parlement que l'exécutif nous regrettons également l'absence de mention du continuum de sécurité, nous considérons que ce silence sur la coopération entre les collectivités et l'État central est étonnant alors que la loi sécurité globale de mai 2021 semblait en faire un tout indépassable, nous craignons que ce silence de soit la traduction de faiblesse que nous avions exprimées à l'époque le continuum de sécurité peut en effet vite ressembler à un marché de dupes, si elle ne consacre pas suffisamment vite des moyens, la sécurité, que ce soit en raison d'un contexte budgétaire ou d'une croissance démographique locale exigeante, une mairie, c'est arrivé récemment pourra être pointée du doigt, si elle le fait, elle prendra la lumière médiatique et donc les coûts en lieu et place du gouvernement et on lui en demandera toujours plus nous considérons pour notre part que la sécurité doit rester d'abord la prérogative de l'État central. Mais j'ai assez parlé de ce qui n'est pas dans le texte, le vôtre de notre groupe repose bien évidemment sur les 3 aspects principaux de ce projet de loi concernant le rapport annexé il y a une certaine cohérence dans le rapport annexé qui nous est fournie, on comprend la filiation avec le livre blanc de la sécurité et le bureau de la sécurité, la place octroyée au numérique, même si nous comprenons les inquiétudes de certains agents, échaudés par les échecs récents nous semble légitime, nous vous remercions d'avoir bien voulu prendre en considération plusieurs améliorations portées par notre groupe à travers de mes amendements de mes collègues Laurence Harribey. Gisèle Jourda ou Patrick Kanner, ainsi en va-t-il de l'accessibilité des locaux et des démarches dématérialisées pour les personnes en situation de handicap et de la meilleure projection des moyens de sécurité civile sur tout le territoire, les modifications apportées au texte qui permettront de s'assurer de l'objectivité du choix d'implantation des 200 brigades de gendarmerie annoncé ou encore d'étudier la création d'une seconde base pour les Canadair constituent de bonnes nouvelles. En ce qui concerne la partie budgétaire, le groupe socialiste fait il se félicite des moyens accordés au ministère de l'Intérieur. Nous en profitons pour exprimer à nouveau un soutien sans réserve à nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, police municipale, qui ne comptent bien souvent ni leurs heures, ni leurs efforts pour assurer la tranquillité de nos citoyens partout sur le territoire. La plupart des candidats à l'élection présidentielle, de gauche comme de droite, s'était engagé à accorder davantage de moyens à la lutte contre l'insécurité, les 15 milliards annoncés dans le texte constitue donc une bonne nouvelle que nous approuvons sans réserve, même si nous serons vigilants sur l'application de cette Lopmi budget après budget dans un contexte hein que économique incertain que nous traversons. Sur les questions de sécurité, j'ai connu la partie droite de l'hémicycle plus discrète. Merci. Pour finir. Les articles normatif on peut évoluer après l'examen, dans l'hémicycle, malgré l'apport bienvenu de mes collègues Rémi Cardon ou Catherine Conconne. Le dépôt de plainte par visioconférence me semble mieux encadrer le projet de radio du futur sera sans doute mieux assurée sans ordonnance, tout comme l'adaptation aux collectivités ultramarines. Nous approuvons l'alignement sur le régime des autres personnes dépositaires de l'autorité publique des peines encourues pour les agressions sur les élus. Nous déplorons le rejet des propositions de mes collègues, Laurence Rossignol et Marie-Pierre de La Gontrie, pour mieux lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales sur les refus d'obtempérer, il est dommage que nous ne soyons pas aller plus loin dans la discussion de l'amendement socialiste qui proposait de revenir au dispositif gouvernemental initial de 2016. Bien sûr nous ne soutenons pas l'extension des amendes forfaitaires. Même c'est les limites voulues par les rapporteurs sont bienvenues. Nous n'approuvons pas davantage les nouvelles modalités d'accès à l'examen d'OPJ ou l'Arctique, le nouveau qui vise les violences dites gratuites. Alors je ne travaillerai pas de secret en disant que nous le sommes arracher les cheveux sur la loi anti-casseurs que nous avions de très profonde opposition sur la loi sécurité globale. Et que tout ne nous plaît pas, et c'est un euphémisme dans cet autre mis. Nous avons envisagé l'abstention sur ses désaccords. Mais notre groupe a choisi de prendre ses responsabilités, la demande de sécurité exprimés par nos concitoyens. Relayée partout par les élus locaux nous a convaincus de voter en faveur de ce texte et des moyens supplémentaires qu'il a qui la loue à nos forces de l'ordre. Je vais donner la parole à Madame, la présidente : Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Madame la présidente de la parole. Monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. être policier c'était au sens de la vie en société, c'est atroce, Centre des choses, écrivait Albert Camus dans les Justes, un policier doit être en contact permanent avec la population, il doit être le garant de la confiance que doivent inspirer les pouvoirs publics, aux citoyens, il s'agit d'un lien de confiance que permet une police de proximité, une conception de la police, défendue par le groupe CRCE mais pas par ce projet de l'autre mis en effet La Lopmi présente, à l'issue de cette première lecture, une conception des métiers de la sécurité intérieure, qui est toujours bien éloignée de la nôtre, et ce malgré l'exercice de notre droit d'amendement au cours de nos débats, nous avons été cohérent avec avec nos interventions passées sur la loi dite de sécurité globale, nous le répétons une autre voie est possible une police, une police qui ouvrent des vocations éveille les jeunes donnent envie de s'engager, ce n'est pas une police trop souvent coupés du citoyen mais une police de proximité exemplaire et digne, tels que de tels que nous le soulignons déjà dans notre proposition de loi visant à réhabiliter cette vision de la sécurité reposant sur le triptyque : prévention, dissuasion, répression, en date du 11 septembre 2017 aujourd'hui cette Lopmi mais à distance les victimes le numérique se présente comme un faux ami vecteur de simplification, être dans la modernité et l'efficacité ne doit pas être synonyme de 7 éloigne La Lopmi ne peut qu'accentuer le fossé entre police et victime le temps passé sur la voie publique dans des actions de sanction ou de répression sera la règle et le temps au commissariat ou à la brigade l'exception aussi je tiens à souligner que la modification de la procédure pénale et du droit pénal induite en particulier par cette distanciation relève de la compétence propre du ministère de la justice et n'aurait pas dû avoir sa place dans une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, vous l'avez reconnu vous-même lorsque vous avez écarté des amendements reprochant au parlementaire d'empiéter sur ce périmètre de compétence pourtant vous n'avez pas su être critique envers votre projet en maintenant votre défense de la simplification de la procédure pénale, or la procédure pénale doit continuer à préserver un équilibre entre l'objectif de recherche la poursuite des infractions et la garantie de la liberté et des droits des citoyens, une simplification de la procédure pénale ne permet aucunement une amélioration de la qualité des enquêtes face à cela, nous avons défendu que la procédure pénale est une garantie indispensable en matière de liberté et de droits fondamentaux pour tous les justiciables qui n'aurait pas fallu simplifié de plus en matière de droit pénal, nous avons mis en relief que l'amende forfaitaire délictuelle représenter un risque d'arbitraire et de disparités de traitement, contraire au principe d'égalité devant la justice, nous dénonçons donc le mec le maintien d'une amende forfaitaire, faisant fi du principe d'opportunité de la peine et nous rappelons qu'il s'agit d'une procédure de masse systématiser qui ne fonctionnent déjà pas en terme de régularisation des délits, nous regrettons également que la question de la formation approfondie des policiers et gendarmes à la procédure pénale n'ait pas été élevé au rang de priorité par ce texte, en effet, la suppression des 3 ans d'ancienneté requise pour passer le concours d'OPJ est un abaissement des exigences en terme de recrutement qui n'est pas souhaitable la responsabilité nécessite la formation, l'expérience et le recul une prise de poste immédiate à la sortie d'école ne permet pas de satisfaire de telles exigences bien que cela soit le cas d'autres écoles de la fonction publique telle que l'École nationale de la magistrature, il est déjà difficile d'être jugé par un juge de 25 ans, alors il sera de même difficile pour un prévenu d'être perquisitionné par un OPJ novice ou par des policiers, être managée par un OPJ sans expérience, ce projet de loi est une loi de chiffres, d'effectifs et ne se penche pas sur l'humain, sur le rapport entre citoyens et police citoyen et services publics, la modernisation du ministère de l'intérieur de l'intérieur se paie au prix de la déshumanisation de la police, on est là dans une rupture le ministère impose sa vision, il ne prend pas en compte, par exemple, la popularité de la police dans les quartiers populaires, mais également les difficultés structurelles de la police, vous devez accepter, Monsieur le Ministre, le constat de cette défiance d'une partie de notre jeunesse à l'égard d'une police qui met la pression, sans s'atteler avec d'autres services publics à resserrer les Liens distendus, c'est une évidence, le tout répressif ne ne fonctionne pas, n'a jamais porté ses fruits, bien au contraire, il faut donc repenser l'action de notre police, mais aussi de la justice dans le domaine du maintien de l'ordre, ce projet de l'consacre également une police de la répression contre ce qui est des nommés dans le rapport annexe la subversion, nous défendons une doctrine selon laquelle les dispositifs de maintien de l'or doivent reposer le plus souvent possible sur la négociation, le dialogue et la pédagogie, une doctrine que nous défendions déjà dans notre proposition de loi visant à interdire les lanceurs de balles de défense et à modifier la doctrine dans ce domaine en date du 22 janvier 2019 il faut enfin tirer les leçons des méthodes d'encadrement des manifestations depuis la loi El Khomri jusqu'au gilet jaune et mouvements lycéens, par exemple, il y a aujourd'hui urgence à tirer les leçons de l'escalade de la violence et de l'usage disproportionné de la force publique par les autorités, un travail d'ampleur doit être engagé pour mettre en oeuvre des stratégies de désescalade efficace et celui-ci doit commencer par une étude sérieuse, complète, détaillée et documentée des avantages et des inconvénients de chaque type de d'autres le groupe CRCE refuse, monsieur le ministre, de stigmatiser les forces de l'ordre, je l'ai dit à plusieurs occasions, et c'est justement, c'est justement parce que nous sommes soucieux des conditions de travail de nos policiers et de nos gendarmes mais également du sens des professions de la sécurité publique, que nous votons contre ce projet de ni il s'agit d'un projet contraire au rapprochement de la police, avec les citoyens, mais également de l'idée que nous nous faisons du métier de policier d'autres peuples expriment souvent une grande inquiétude face aux questions de sécurité, nous ne pensons pas, contrairement à vous, que la fuite en avant sécuritaire répondent à ces préoccupations, les six Monsieur le Ministre, sont là pour le prouver, c'est dans le cadre d'un projet de société qui met le service public au coeur de l'épanouissement collectif que nous concevons une action de la police renouvelée restaurer et efficace. La parole est à un autre collègue Loïc Hervé là pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, co-rapporteur le texte portant loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur va franchir une nouvelle étape cet après-midi devant le Sénat. Et si le texte a été Simunic Fika hâtivement réduit entre son 1er et son second dépôt la discussion parlementaire qui, une fois n'est pas coutume a débuté au Sénat aura permis des échanges qualitatif dans la haute assemblée a le secret, et désormais l'exclusivité cette ambiance tient autant que vous avez consacré personnellement Monsieur le Ministre, pour répondre à chacun de nos collègues quand ils déposaient des amendements et ça s'est vu au cours des 3 jours où nous avons siégé. Le texte qui a connu des évolutions significatives au stade de l'examen en commission comme au au niveau de la séance publique les propositions d'amélioration sont devenus de tous les bancs de l'hémicycle et un certain nombre d'entre elles sur tous les bancs de l'hémicycle, ont été retenus par le Sénat. Ainsi à l'article 1er l'économie générale du rapport annexé n'a pas été bouleversé mais plutôt conforté. Le rapport a été amendé ponctuellement pour être enrichi par les travaux de la haute assemblée et la connaissance empirique des sénateurs dans leur département, à cet égard comme certains collègues, ils viennent de le dire, je pense, ou 200 nouvelles brigades de gendarmerie mais je pense aussi à leurs modalités de construction et au rôle que les collectivités territoriales vont jouer aux côtés de l'État pour rendre ces brigades réalité. Je pense également à l'amendement porté par notre collègue Dominique Derrien sur les maisons de la confiance dans chacun de nos départements. Le sur de la cybersécurité a été longuement évoquée dans nos échanges et c'est bien nécessaire, tant les attaques numériques et les demandes de rançons sont entrés dans la vie de nos entreprises. Contraindre au dépôt de plainte dans un délai rapide, c'est permettre à nos cyber policiers et à nos cyber gendarmes d'intervenir au plus vite, en plus de la modernisation numérique de votre ministère, l'essentiel : la moitié de l'effort prévu dans cette Lopmi nous avons inscrit dans le dur de la loi, le réseau radio du futur et grâce à vous Monsieur j'étais rendu témoin que les industriels français retenus sont déjà à l'oeuvre notre pays pourra donner à nos forces de sécurité comme aux services de secours, des moyens de communication modernes est résiliant en cas de crise. Je tiens ici à dire que sur proposition de mon collègue co-rapporteurs Marc-Philippe Daubresse, le Sénat a renforcé une fois encore notre arsenal pénal contre les violences contre les élus, les refus d'obtempérer et les rodéos urbains, l'actualité nous rappelle combien il est nécessaire que les moyens de terrain puis suivre la sévérité renforcée de la loi que nous avons au coûts dans le reste du texte, des mesures d'améliorations ont été apportées pour simplifier la procédure pénale, nous avons permis le recours à la visioconférence pour la prise de plainte, comme pour la déposition permettant une fois de plus, de prendre en compte des réalités nouvelles réalités vécues par nos concitoyens par des justiciables, parfois très très éloignés des commissaires de police et des brigades de gendarmerie, ça n'est qu'une faculté proposer évidemment à nos compatriotes et pas une obligation mais dans ce texte, c'est bien la création des assistants d'enquête auprès des officiers de police judiciaire qui devra être de nature à améliorer significativement le quotidien des enquêteurs en lice sous sous l'agent d'une charge administrative bien trop lourde. Dès l'entrée en vigueur du texte, il faudra embaucher et former ces 5500 personnels dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale, c'est finalement l'enjeu majeur qui sera désormais votre Challenge Monsieur le Ministre, celui de votre ministère, une fois que le texte sera promulgué. Le Sénat a fait le choix d'accompagner la déjudiciarisation de nombre d'affaires en privilégiant le recours aux amendes forfaitaires délictuelles, nous n'avons pas emprunter le chemin périlleux de leur généralisation qui aurait conduit à aboutir à quatre mille CAF de figure où les AFD aurait été possible. Il y a actuellement dans le droit positif, dit délit pour lequel l'AFD est possible avec le texte que le Sénat s'apprête à adopter, il y en aura 24 14 de plus, nous pourrons ainsi évaluer leur mise en oeuvre infraction par infraction, nous savons que certaines AFD fonctionnent bien, voire très bien d'autres fonctionnent plus difficilement et ce sera tout l'intérêt du contrôle parlementaire de faire cela, nous avons renforcé l'outrage sexiste et sa répression, nous avons même renforcé le la la répression contre l'outrage sexiste aggravé qui devient désormais un délit, c'est quelque chose d'extrêmement important : le lien avec le texte n'est pas aussi évident que cela, mais l'actualité, encore une fois, nous rappelle l'importance d'avancer sur ce terrain, nous avons aussi j'y viens à ma chère collègue, nous avons aussi renforcer le pouvoir des préfets dans le département, fort de l'expérience qui a été celle de la crise Covid et des travaux du Sénat en la matière, de mettre aussi les agences régionales de santé à disposition des préfets, comme toutes les administrations de l'État quand il s'agira de prendre des décisions de terrain rapide et d'être efficace est résiliant parfois notre discussion du texte, mes chers collègues, a permis de mettre en lumière d'autres débats. qui sera nécessaire de poursuivent dans des textes plus approprié si sur la réforme judiciaire, la commission des lois du Sénat a confié à 2 de nos collègues, le soin de conduire une mission d'information, je je dois rappeler ici que nous avons eu des débats sur la question des violences conjugales et intrafamiliales, nous avons eu des débats aussi sur le, la question du droit des images, notamment dans la perspective de l'organisation des Jeux olympiques, nous avons eu des débats sur la question de l'accueil des gens du voyage. Monsieur le ministre, il appartient au gouvernement maintenant de donner les textes qui permettront de débattre de ces sujets-là, en tout cas le Sonia s'y emploiera pour ce qui le concerne, monsieur le Ministre, ce texte donne des moyens significatifs aux missions régaliennes de votre ministère, il est fortement attendu par le terrain par des actes, des acteurs qui le mérite, oh combien nos auditions l'ont montré, l'adoption de ce texte devra devrait réunir un consensus assez large : OK, le groupe de l'Union centriste apportera son soutien, je vous remercie. Je vais m'maintenant donner la parole à notre collègue Jean Louis Masson qui n'appartient sur la liste d'aucun groupe.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce texte est vraiment un excellent texte et disons, il faut se réjouir de ce que nous soyons amenés à examiner des propositions aussi aussi positive et porteuse de remise en ordre au niveau de l'Ordre public de la délinquance et d'un certain nombre de dossiers, c'est donc pourquoi, la raison pour laquelle, à titre personnel j'avais initialement décidé de voter pour ce texte Cependant, quand on prend en compte ce type de texte, on se rend compte de ce que son application va dépendre aussi de l'ensemble de ce qui l'entoure et des mesures qui sont prises, or il y a dans votre politique qui vient d'être annoncée, qui est depuis un certain temps, il y a une mesure qui me qui m'inquiète profondément et qui m'amène à vous dire que tout ce qu'on peut faire pour renforcer, je dirais les les structures cocktail que vous le faites dans ce texte de loi, hé bien, risquent d'être menacés par certaines réformes que vous envisagez par ailleurs et je pense notamment à la mise sous tutelle de la police judiciaire sous l'Ordre sous les ordres des préfets et sous les ordres des pouvoirs locaux, moi, je crois, Monsieur le Ministre, qu'on ne peut pas donner beaucoup de pouvoirs à la police s'il n'y a pas à côté, un lien avec la le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire et ce qui accompagne le pouvoir judiciaire en l'espèce, la police judiciaire et tous ceux, tous ceux qui sont depuis un certain temps dans la vie publique savent très bien que dans les grandes villes, il y a toujours des microcosmes avec des relations entre le préfet, on entre, on finit par entretenir des Liens entre le préfet, le un certain nombre de de structure, que ce soit politique, économique ou autre et ce qui faisait la force qui fait la force de la police judiciaire, c'est que la police judiciaire n'est pas actuellement impliqué comme le reste de l'administration de la police dans les rapports locaux avec les, les risques d'influence et même plus des risques, hein, parce que dans certaines villes, ben, on se rend bien compte que c'est c'est plus ils, ce sont des réalités avec certaines certains réseaux d'influence, et je crois que tout ce que vous faites là est gâchée par à côté des des actions Paul des choix politiques qui sont complètement aberrants et qui sont mais profondément inquiétant du point de vue du respect d'une certaine indépendance de la justice d'une, de la justice et des organes qui travaillent pour la justice que la tels que la police judiciaire et je crois qu'il y a là quelque chose qui est vraiment qu'on ne peut pas accepter, je ne sais pas si ça compte tenu des rapports entre fin de la de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, je ne sais pas si ce cette réforme de la police judiciaire passera au Parlement, et c'est la raison pour laquelle je profite de cette, de cette séance pour vous faire part de ma totale réprobation de ce qui est envisagé, et je crois que cela rassurerait tout le monde que disons cette réforme soit abandonné au niveau de la police judiciaire, merci. Je vais donner la parole madame la présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la présidente. Monsieur le président, Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au terme de l'examen de ce projet de loi je voudrais partager le constat que ce texte tant dans ses propositions initiales, mais aussi par les apports conséquents du Sénat, que cela soit au regard de ces dispositions programmatique mais également normative va dans la bonne direction, de saluer ici le travail de nos co-rapporteur et votre investissement Monsieur le Ministre, dans vos explications. Sans refaire le sommaire du rapport, il comporte un certain nombre de sujets pour lesquels nos forces de sécurité publique, attendez un développement et un soutien notamment matériels techniques numériques et juridiques, notre assemblée a supporter d'autres sujets, et notre groupe, celui par exemple de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et je me réjouis que nous ayons adopté plusieurs amendements apportés par notre collègue Maryse Carrère, de se féliciter de la perspective budgétaire pour laquelle l'augmentation annoncée semble à la hauteur des enjeux de sécurité publique auxquels notre pays est et sera confronté, pour autant, il faut que ces moyens soient déployés à bon escient, je pense notamment à la formation, les carences en matière de formation ne sont plus à démontrer, surtout s'agissant de la formation continue, le rapport annexe qu'il s'agisse du numérique ou des métiers de terrain j'espère donc il sera suivi d'effet, d'autant plus au moment où l'article 9 supprime les 3 années de pratique pour devenir au de revenir également sur l'implantation de nouvelles casernes de gendarmerie pour assurer le maintien de l'or dans les territoires ruraux chacun, c'est la nécessité d'implanter de nouvelles brigades notamment dans les territoires qui connaissent une poussée démographique et cela touche la Gironde, Monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion de vous le dire durant nos échanges, c'est donc un point sur lequel je serai attentive et je sais que je ne ferais pas la seule, vous vous en doutez, au cours de ces travaux, nous avons pu aborder longuement certains aspects, je pense en particulier à la réforme de la police nationale et plus spécifiquement aux problématiques liées à la police judiciaire, nous avons été quelques-uns à relayer les inquiétudes provenant des acteurs de terrain et des magistrats notre assemblée a pu faire inscrire dans le dur, que la réforme devra tenir compte des spécificités de la police judiciaire, vous avez eu Monsieur le Ministre des propos rassurants, notamment quant à la question de l'indépendance des magistrats dans la direction de l'instruction, nous espérons que ces engagements permettront de réformer sereinement notre police car oui les Vosges dilution de cette dernière est nécessaire je pense également que les travaux menés pour cadrer l'usage de l'amende forfaitaire étaient les bienvenus le projet initial soulever des inquiétudes par sa généralité, la rédaction de l'article 14 par nos rapporteurs qui limitent strictement le Champ d'application du dispositif est de nature à nous rassurer l'amendement du gouvernement adopté en séance à compléter le dispositif, je pense que cette solution est plus sage au regard des principes qui gouvernent notre justice, l'une des innovations de ce texte reste aussi l'objet d'interrogations, je pense à la création de la nouvelle fonction d'assistant d'enquête, l'analogie avec les greffiers séduisante, mais elle présente aussi son lot de questionnements, comment seront-ils formés, encadrés, comment seront-ils rémunérés, comment seront-ils répartis comment seront-ils contrôler des échanges ont eu lieu en séance, je ne crois pas qu'il faille renoncer à l'institution de ces nouveaux personnels mais il faudra veiller à la manière dont ils seront institués. Monsieur le Ministre, il reste cependant en terme de nos échanges quelques interrogations, voire quelques regrets, notre collègue Roger Karoutchi là évoqué très justement des la discussion générale, la police et la justice se plaignent souvent l'une de l'autre, au point de s'opposer parfois alors qu'il y aurait lieu de les penser ensemble, de ce point de vue ce texte donne le sentiment d'une occasion manquée, sentiment largement renforcés par la manière dont les irrecevabilité ont été prononcées, j'en veux pour exemple un amendement que j'avais déposée et qui reprenait les dispositions de la proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un idylle victimes d'agressions. Cet amendement a été déclarée recevable car ne s'inscrivant pas dans le périmètre de la loi, je comprends évidemment le raisonnement qui a conduit à cette décision dès lors que nous n'aime Sami, non pas un texte qui touche à la question du procès mais nous voyons aussi la limite de l'exercice qu'aura représenté cette loi de programmation, d'un côté nous adoptons un article 7 bis qui vise à renforcer la protection pénale des élus quand d'un autre, nous ne pouvons pas examiné d'autres dispositifs qui participent à cette même finalité au motif qu'il y serait question de l'organisation du procès et donc du ministère de la justice, plutôt que de l'intérieur ce cloisonnement d'ordre quasi-administratifs et regrettable, il a parfois d'ailleurs mené à des confusions sur d'autres débats également important mais il est vrai qu'une partie conséquente des articles du projet initial du mois de mars n'a pas été retenue dans l'affaire Sion finales présentées notamment un volet justice important cette loi de programmation n'est qu'une première étape, nous attendons beaucoup des prochains textes qui devrait nous être présenté et nous l'espérons rapidement dans cette attente, notre groupe dans sa grande majorité se prononcera en faveur de ce texte, je vous remercie. Donner la parole à monsieur Marc Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des lois, mais chers collègues. Monsieur le Ministre, la réponse est oui, mais quelle était la question. Si la question qui nous est posée, consiste à savoir si nous nous réjouissons de trouver dans un texte, une renforce un renforcement significatif des moyens du ministère de l'Intérieur pour faire face à l'augmentation de la violence et aux nouveaux circuits de délinquance organisée, nul doute que nous allons soutenir avec beaucoup de ferveur texte mais s'il s'agit. De répondre à la vraie question que se posent tous nos compatriotes mais quand donc va-t-on rétablir l'autorité de l'État dans nos villes et dans nos campagnes, quand donc va-t-on, comme le dit le président Retailleau réarmer l'État sur le plan migratoire et sécuritaire, vous ne recueillerait que notre scepticisme car le droit à la sécurité n'est pas qu'une question de police, c'est d'abord et surtout le problème d'une réponse pénale inadapté à la violence de notre société, la genèse du projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui monsieur le monsieur le ministre est longue, il fait suite, on l'a dit à la publication du Livre blanc qui qui s'est concrétisé par le bobo de la sécurité qui a été suivi avec beaucoup de compétences et d'appuyer par notre collègue Henri Leroy et finalement vous nous avait présenté un projet plus resserrée que vous avez déposé sur le bureau du Sénat le 7 septembre nous vous remercions de cette marque de considération. Mais en retour, vous pouvez nous donner acte des nombreuses améliorations qui ont été apportées par la commission des lois dans un climat serein, comme l'a dit mon excellent ami Loïc Hervé avec un débat approfondi qui a été enrichi par les très nombreuses réponses pédagogiques que vous avez fait, monsieur le Ministre, et nous vous en sommes reconnaissants de voler manque cruellement aux dispositions qui relève de votre compétence, celui sur l'immigration qui est enfin reconnue comme une des causes principales de l'augmentation de la délinquance de notre pays et celui sur l'utilisation. Des techniques de l'image et de l'Intelligence artificielle de la reconnaissance faciale qu'il est plus que temps que mettre en oeuvre si on veut aborder, vous le savez bien sereinement les grands événements comme la Coupe du monde de rugby ou les Jeux olympiques. qui manque cruellement à votre dispositif et qui a frustré de nombreux collègues qui n'ont pas pu présenter leurs amendements comme Madame Delatte, qui avait un excellent amendement mais qui n'a pas pu le présenter, c'est justement l'amélioration de la réponse pénale qui la qui demeure la principale cause de l'inefficacité de vos politiques, comme l'a justement dit notre excellent collègue Roger Karoutchi la sûreté. La Sûreté. N'est pas aujourd'hui un droit fondamental pour chaque citoyen, pour cela, il faudrait une objet une loi d'orientation et de programmation de la justice, justice qui est. C'est comme lente inefficace et inéquitable cette loi, nous l'attendons depuis plusieurs années et comme soeur Anne, nous ne voyons rien venir présenter une loi d'orientation de la police, sans y ajouter une telle réforme, c'est se condamner à l'impuissance publique que dénonce jour après jour, nos compatriotes au total si je reviens à votre texte monsieur le Ministre, 15 milliards d'euros supplémentaires, dont 7 milliards consacrés aux nouvelles technologies au numérique. 2 fois plus de présence, vous nous avez expliqué comment de forces de sécurité intérieure, sur le terrain équitablement répartis 8500 postes entre gendarmes et policiers et la capacité de mieux faire face aux nouvelles frontières digital et de mieux prévenir les menaces et les crises du futur pour l'essentiel, évidemment nous serons favorables à ces dispositifs, et d'ailleurs ils reprennent beaucoup de propositions que nous avions fait antérieurement. Vous avez un Monsieur le Ministre dans votre loi. Un rapport d'orientation très intéressant et les rapporteurs avec le président Buffet nous avons voulu que ce débat ait lieu complètement sur ce rapport et vous également. Et finalement, ce rapport, quand on l'écoute quand on le lit et il dresse un réquisitoire assez implacable de l'augmentation de la violence dans notre pays depuis 5 ans. Et elle explique qu'il faut de nouveaux moyens, c'est ce que vous faites aujourd'hui, Monsieur le Ministre. Mais il y a un certain nombre de sujets qui peuvent fâcher : d'abord la réforme. De départementalisation de la police nationale, notamment sur les questions de la police judiciaire nous avons fait inscrire dans la loi qu'il fallait tenir compte des spécificités de la police judiciaire dans le débat, monsieur le ministre et je vous en donne acte devant la Haute Assemblée, vous vous êtes engagé, vous avez dit que s'agissant de la nécessité impérative que la pèserait sur l'autorité du procureur de la République s'agissant du fait que tout ce qui est affaire Censier manquements devoir de probité devait rester exclusivement du ressort de la PJ, s'agissant du fait que pour la délinquance organisée, qui n'a pas de frontières, il faudrait une réflexion zonal et non pas une réflexion étriqué dans le carcan départemental, vous en étiez d'accord. Cela va sans dire, ça ira mieux en l'écrivant et donc au moment de la CMP, comme je vous l'ai dit, nous déposerons un amendement pour que ce soit écrit dans votre rapport d'orientation. Par ailleurs. Vous avez présenté un certain nombre de choses sur la question de la nécessité de travailler mon collègue et sur les plaintes en ligne, je pense, nous avons singulièrement améliorée, ce dispositif, dont je rappelle qu'il ait une faculté et pas une obligation et qui au contraire va rapprocher le citoyen de sa police, enfin, à l'initiative de notre groupe, les auditions ont montré l'urgence et l'importance d'améliorer la réponse pénale face aux violences sur la voie publique, c'était bien le périmètre qui était défini dans la loi sur 3 enjeux essentiels : les violences faites aux élus les refus d'obtempérer et les rodéos urbains, j'ai donc proposé un article 7 bis qui a été votée, une fois n'est pas coutume pas ici de temps en temps, à l'Assemblée, beaucoup moins à une très large majorité pour qu'on renforce significativement les sanctions correspondantes pour mieux protéger tous ceux qui se mettent au service de la société, je rappelle ici que les atteintes compte les dépositaires de l'autorité publique, c'est plus 35 % que l'année dernière les atteintes et les violences faites aux élus, c'est plus 47 % que nous sommes dans une société où il est grand temps donne le même statut aux élus locaux que les représentants des forces de l'ordre qu'il soit enfin complètement. S'agissant du Christ feuilleton des refus d'obtempérer, là encore, un refus d'obtempérer, tous les vingt minutes dans notre pays, mes chers collègues, et contrairement à ce qu'ont dit certains collègues sur d'autres bancs ce n'est pas avec une augmentation des tirs de policiers depuis 5 ans, les tirs de policiers face au refus d'obtempérer, sont en recul, c'est donc pas uniquement avec des mesures de prévention mais bien que des mesures de répression que nous pourrons traiter ce triste feuilleton des refus d'obtempérer. En conclusion. Notre vote positif sur ce projet, Monsieur le Ministre, est un vote lucides et vigilants, évidemment nous le maintiendrons CMP avec tout ce que je viens de vous dire telle de Candide de Voltaire, finalement, vous avez bien cultiver le jardin de la police, mais il reste beaucoup à défricher sur les jardins de la justice et de la procédure pénale avant que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au cours de la semaine précédente, nous avons débattu d'un texte très attendu par nos concitoyens, tous constatent une augmentation de l'insécurité dans notre pays, les violences contre les personnes vulnérables sont devenues quotidiennes, certaines zones du territoire tentent à se soustraire de l'autorité publique à l'autorité publique faisant vivre un véritable calvaire à nos concitoyens, il est temps que cela change l'ensemble de nos concitoyens ont besoin d'ordre et de tranquillité publique, nos entreprises aussi ce texte constitue une première réponse à la dégradation du climat sécuritaire que notre pays connaît depuis plusieurs années, des augmentations de budget prévu jusqu'en 2027 sont importantes : sept heures est nécessaire car les défis auxquels notre pays devra faire face le sont aussi résurgence du terrorisme islamiste, criminalité organisée mais aussi accueil de grands événements sportifs et bien d'autres. Ces Budgets serviront à moderniser le ministère de l'Intérieur, bien sûr, mais ils seront également employé à recruter davantage d'effectifs, c'est ainsi que 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront créés 8500 agents rejoindront les rangs de la police et de la gendarmerie pour renforcer leur présence dans la rue, les agents des forces de l'ordre doivent être plus nombreux mais ils doivent également pouvoir se consacrer pleinement à leur mission, certaines recrues deviendront ainsi des assistants d'enquête cette nouvelle fonction parfois de celle de greffier doit permettre aux policiers, de gendarmes, d'accentuer leur présence sur le terrain des assistants d'enquête se chargeront de la myriade de tâches administratives qui submerge actuellement les agents au cours des débats, nous avons eu l'occasion de dénoncer la complexification de la procédure pénale, à force de réformes sectorielles, le code est devenue impraticable pour les policiers et les gendarmes pizza encore le rapport des états généraux de la justice estime que cette complexité et l'une des raisons majeures de l'allongement des délais, même les juges peinait à s'y retrouver. Cet allongement n'est bon pour personne, ni pour les victimes qui doivent attendre longtemps avant que la justice ne leur soit rendue, ni pour les mises en cause, qu'il n'est pas bon de tenir longuement éloigné du bras de la justice, le-ci doit être rendu avec efficacité, clarté et célérité pour cela, il faudra s'attaquer à la simplification de la procédure pénale et sans doute fusionner les régimes de l'enquête préliminaire et de l'enquête de flagrance. Grâce aux travaux réalisés en commission et en séance, le texte a été enrichi. 2 sujets majeurs me semble devoir être mis en lumière le 1er est celui des rodéos urbains piètre divertissements de ce qui devrait avoir mieux à faire lorsqu'elle met en danger la vie de nos concitoyens, les peines de 7 infractions ont été sensiblement alourdi 5 ans et 75000 euros d'amende, il est hors de question que la vie de nos concitoyens soit menacée, le second et celui des violences contre les élus, les Français sont scandalisés à juste titre, que leurs élus soient pris à partie ou agressé l'élu local ou national est un représentant du peuple, il représente ses électeurs mais il représente aussi la République dans son ensemble, l'élu Anne est une composante essentielle leur porter atteinte revient porter atteinte à la République, il était temps de renforcer les sanctions contre ces agressions inacceptables le seront désormais punis au même titre que celle commise ou contre les policiers, nos concitoyens l'attendaient davantage de fermeté dans les sections dans les sanctions, s'il a été enrichi par les débats, le texte n'a, n'est pas deviner devenu pour autant un catalogue, c'est ainsi que la procédure de l'amende forfaitaire, elle n'a pas été généralisé mais étendu cette procédure se justifie pleinement pour certaines infractions, mais elle ne n'a pas vocation à devenir la norme, la commission et le gouvernement se sont accordés pour y inclure 14 nouvelles infractions actuellement, certaines d'entre elles ne donne bien souvent lieu qu'à un simple rappel à la loi, c'est le cas de l'atteinte à la circulation des trains ou de la filouterie de carburant, gageons qu'à présent l'amende forfaitaire permettra aux contrevenants de ne pas oublier la leçon, cela permettra non seulement une réponse pénale plus rapide et plus certaines mais cela évitera également des procédures longues et chronophage pour les infractions du quotidien, l'objectif de cette loi et de renforcer la présence des policiers, des gendarmes dans la rue pour cela le texte, les décharges de bons nombres de tâches administratives, nous l'avons dit il leur permet également de recourir à des procédures simplifiées pour renforcer les effectifs, le texte supprime aussi la condition d'ancienneté nécessaires pour se présenter à l'examen d'OPJ d'officiers de police judiciaire, si cette mesure ne réduit en rien les compétences requises pour réussir cet examen, il nous semble important que les jeunes recrues bénéficient d'un encadrement suffisant, ces jeunes sont souvent affectés dans les zones les plus difficiles dans notre pays, là où la tension est la plus forte, c'est dans ces zones que l'encadrement est le plus nécessaire, nos forces de l'ordre ont font face à des situations délicates souvent dangereuses, je veux saluer le travail qu'ils accomplissent dans une ville comme ruralité le sont une composante essentielle de notre République, par ce texte, nous ne faisons pas que leur témoigner notre respect, nous leur donnons des moyens supplémentaires pour remplir leur mission, ces augmentations initie une nouvelle dynamique que nous l'espérons, durable, car elle est nécessaire pour nos forces de l'ordre, l'ensemble de notre groupe votera en faveur de l'adoption de ce projet de loi. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue Guy Bénard Roche pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Vous avez la parole. après des heures de débats plus ou moins construite. Six plus ou moins cohérent dans leur argumentaire, plus ou moins mesurés. Nous devant valider approuvé la lampe, ce texte avait une particularité de nous présenter au travers du rapport annexé à son article 1er une vision portée par le gouvernement de la sécurité de la tranquillité publique pour les prochaines années. Cette loi est bel et bien une loi d'orientation mais lacunaire ne présentant pas le projet sur l'ensemble des politiques du ministère certains aspects sont effectivement développé de façon claire et lisible, dont 13 dans une pénombre préoccupante nos prises de pas. Moins nombreuses, certes il notre engagement lors de ces longues séances. Profondément dans la volonté de dans le groupe de présenter et de défendre son projet pour la sécurité de notre pays un projet cohérent, nous avons bien perçu, par contre, la continuité d'une politique qui se veut plus répressive que protectrice qui obère les Liens avec les citoyens, causant ou aggravant une rupture de confiance mais aussi en même temps une immense souffrance au travail de nos forces de l'ordre, nous partageons tous l'objectif police bénéficiant de meilleures conditions d'une meilleure formation, avec des moyens humains mobilier. Mobilier satisfaisant dans le but d'exercer ses missions auprès de la population auprès de la population, avec la population pour la population, c'est bien là le coeur des propositions que nous avons. Supporter Monsieur le Ministre, oui nous devons soutenir l'action de la police républicain dans ces cas, au service de la population toute la peau. Assure les Français à l'aide avec le numérique, comme les 13 millions d'ailleurs qui souffrent d'électronique. Que dire du la doctrine du maintien de l'ordre, pas des choses sur la justification de l'utilisation de tactique plus de discutable, nous ne voulons pas Des BD des drônes de lacrymo de la tactique de la DASS ou d'autres techniques d'interpellation dangereuses oui dans le groupe, cherché à entamer un vrai dialogue avec le gouvernement, avec la majorité de cette assemblée, dialogue sur les attentes des citoyens qui de police à leur service, nous sommes déçus de d'avoir vu aucune de nos propositions sur la réforme de l'IGPN par exemple étudier de manière sérieuse, cette réforme est plus des Césaire et plus attendu par nos concitoyens que celle dite de la police judiciaire qui est à l'avance à marche forcée, contre l'avis de beaucoup en ayant déjà fait c'est. Premières victimes dans le directeur de la PJ Sud monsieur le besoin de sécurité des citoyens portent sur la transparence de l'action de la police, une meilleure gestion de dérive une nouvelle vision de l'IGPN mais aussi sur la transparence des données de la police de leur publication de leur transmission entrante aux élus locaux. Notre groupe, s'est étonné à plusieurs reprises de la position de la majorité, c'est La Touriale de la position changeantes de ses rapporteurs sur ce qui devait faire partie du débat, rejetant un certain donc d'un amendement précisant que ces derniers sur des sujets en cours d'étude par des mission sénatoriale préconisant des modifications législatives ultérieures où se retranchant derrière le fait que les débats ont déjà eu lieu précédemment pour refuser toute discussion nous refusant toute proposition d'adaptation fonction d'impacts de mesures déjà votées d'Andrew pas tenté de manière parfois inaudible, semblerait-il de présenter sa vision des moyens dans le ministère a besoin, nous avons soutenu l'augmentation du budget à l'article de nous aurions aimé pouvoir être plus entendu dans nos propositions d'amélioration des conditions de travail des forces de l'ordre de l'amélioration de leurs relations avec leurs usagers qui en découlent, notre groupe a voulu que la formation initiale et continue, bénéficient réellement d'une pluralité d'intervenants et soient plus protectrices des agents, y compris en augmentant et sanctuarisant le travail duel au au La prise en compte des droits de la défense que nous portions alimentée par les rapports de la Cncdh, du syndicat de la magistrature ou des avocats n'a hélas pas trouvé une oreille attentive, comme par exemple dans l'inscription de l'interdiction de la reconnaissance faciale, nous avons aussi de nouveau voulu engager une discussion réaliste sur les caméras piétons qui jusqu'à présent, se sont avérés assez inutile pour le citoyen, comme pour les agents des forces de l'ordre nos inquiétudes sur les droits des justiciables n'ont pas été dissipé par nos discussions relatives à l'amende forfaitaire, le déploiement de l'amende forfaitaire est un signal fort, un mauvais signal pour nous un outil cyniquement utile comptablement pour le ministère, mais dans l'efficacité sur la réponse pénale n'est que peu étudié les problématiques de contestation sans réels et pour l'instant sans réponse l'opportunité de poursuivre, qui revient d'habitude au juge et nié de nouveau et n'y voyez pas un reproche à nos forces de l'ordre, son utilisation semble très très variable selon les territoires. Les territoires justement je salue l'adoption de l'amendement de mon collègue Thomas Dossus sur le dialogue nécessaire avec les maires, sur la gestion des fermetures des commissariats le continueront de sécurité dans le gouvernement s'est fait grand défenseur ne pourra faire l'économie de dialogues là encore apaisé mais surtout chiffrés avec les élus et les décideurs locaux. Alors mis quand il y a quelques éléments sur les besoins de lien entre le ministère de l'Intérieur et la recherche, mais aucune des 2 modes de notre groupe permettant tel suivie n'a été adoptée et là encore nous le regrettons, pourtant, nous avons été agréablement surpris du soutien par le gouvernement dans ce que nous avons proposé des avancées pour généraliser des mécanismes ayant fait leurs preuves, par exemple, les agents de liaison LGBT plus ou pour exploiter au mieux les formations nécessaires par exemple les agents formés au cyber harcèlement ces propositions n'ont pas trouvé grâce auprès des rapporteurs, pour des raisons qui m'apparaissent encore obscurs nous saluant l'adoption de l'amendement de notre collègue Monique de Marco, sur les besoins de base supplémentaires pour faire face aux incendies, nouveau plus fréquents plus fort auquel les pompiers sont confrontés, nous aurions aimé pouvoir discuter d'autres mesures ou vision tout aussi importante, la gestion des frontières, particulièrement avec les drônes, le maintien de la possibilité ou pas du port d'armes hors service dans les établissements recevant du public, des fois, la discussion a été refusé car elle avait déjà eu lieu d'autrefois, car elle ferait l'objet de débats ultérieurs en conclusion, j'ai pu à mettre aux prises avec les collègues rappeler combien les forces de l'ordre sont au coeur de notre pacte républicain, ce sont elles qui endosse le rôle de protection de notre population, il s'agit donc de leur donner les moyens de travailler dignement correctement, mais aussi de permettre à notre population, d'avoir confiance dans leur formation dans la préservation des droits de la défense dans leur organisation et dans leur fonctionnement, les craintes que nous avions exprimées au début de l'étude de ce texte, or malheureusement été nos prises de paroles, nos propositions, nos amendements ont défini une vision équilibrée vers laquelle vous n'avez pas jugé bon d'avancer, ne serait-ce que très partiellement l'orientation définie par cette loi du ministère de l'Intérieur ne nous paraît Nick convaincante ni justifiée : nous ne pouvons donc pas nous y associer et nous voterons contre ce projet de loi. Merci. Je vais maintenant donner la parole au président Alain Richard pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole monsieur le président, messieurs. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'adoption du projet de loi telle qu'il ressort des débats du Sénat nous paraît naturel, et je me dispenserait de la sortir comme d'autres orateurs d'une collection de critiques à l'encontre du gouvernement, je voudrais donner les 3 raisons principales de notre soutien, la première, la plus consistante, si j'ose dire, réside dans la partie programmatique de ce projet de loi et précisément son article 2 qui encadre de façon précise l'attribution de moyens aux différentes composantes du ministère. Qui est pas par nature, celui de la sécurité des Français et de la protection quotidienne de leur liberté. Cette injection de moyens fait suite à une remontée de capacité déjà réalisés au cours des dernières années, avec la création des 10000 postes de policiers et de gendarmes qui se conclut cette année conformément aux engagements pris en 2017 avec aussi un renforcement de la formation des personnels de terrain et une remontée plus récente mais sensible des crédits d'équipement dont nous commençons à voir les signes dans les locaux d'actifs, il l'accueil des brigades et des commissariats et parfois aussi sur leur véhicule, le projet sur lequel nous allons voter organise ce nouveau renforcement en ne laissant sur tous les éléments du tableau de bord, si j'ose dire, du ministère de l'Intérieur, d'abord les effectifs 8500 policiers et gendarmes créés au cours des 5 années à venir et nous souhaitons, c'est bien l'esprit du projet et les termes de son de son rapport d'orientation, nous souhaitons veiller bien sûr à la bonne répartition territoriale de ses nouveaux nouveaux effectifs en regardant particulièrement les attentes et les besoins des secteurs périurbains et aussi bien sûr du monde rural. L'annonce des 200 brigade et donc certainement quelque chose que nous allons suivre positivement et je veux souligner aussi, ça n'a pas encore été évoqué le développement de la réserve qui augmentera là aussi les capacités humaines du ministère, il y a également un relèvement important des moyens de fonctionnement n'y assiste pas et puis toute la transformation numérique et sur ce point, je voudrais souligner que c'est à mon avis, de mal regardé le sujet que de parler de déshumanisation, c'est au contraire le développement numérique la démultiplication des capacités d'action de chaque personnel de police et de gendarmerie, qu'il s'agisse des démarches dématérialisées des outils de travail disponible en plus en pleine efficacité dans chaque véhicule ou sur la voie publique avec l'accélération des moyens numérisé de police technique et scientifique et on pourrait multiplier les exemples : le ministère et ses personnels seront donc plus en phase avec les attentes des citoyens et sera aussi outillés. Pour répondre à des formes de délinquance qui exploitent de plus en plus eux aussi l'espace numérique. Cette programmation apporte donc un une une réponse au bon niveau défi qu'apporte quelque affronte aussi nos forces de sécurité civile. Et principalement les services d'incendie et de secours, le programme de renouvellement des flottes d'hélicoptères et d'aéronefs anti-incendie de forêt et bien sûr une des pierres angulaires de l'ensemble du plan et ce sera une satisfaction et un encouragement pour tous les personnels des services si souvent mobilisés. les dans les améliorations de moyens, je veux souligner la volonté de la d'améliorer le l'accueil de chaque victime la priorité particulière pour recevoir et soutenir comme il se doit, les victimes de violences intrafamiliales et les dispositions importantes qui sont prévues en terme de moyens d'accueil et d'accompagnement et de formation des personnels. La 2ème grande raison d'approuver ce projet c'est qu'il offre un cadre de cohérence et une méthode de travail pour l'ensemble des services, il prévoit, et c'est l'intérêt particulier du rapport de présentation qui encadrent le projet d'organiser mieux les services de l'État face aux crises et aux crises institutionnelles de toute nature, en s'appuyant sur nos expériences récentes, nous aurons aussi à intensifier notre coopération internationale sur les sujets de sécurité, de prévention et de renseignements et particulièrement notre coopération européenne sur tous les enjeux de sécurité la démarche affirmé par le rapport que nous allons approuver fait aussi la part nécessaire à la modernisation des méthodes de ressources humaines, il s'agit d'un ensemble de plus de 250000 personnels et il faut veiller à leur bien-être au travail et à leurs perspectives de de carrière à leur temps de travail de de formation encore améliorer, très heureux des pistes d'accompagnement des personnels, en particulier des jeunes entrant dans les services, qui affronte des mobilités souvent difficile. Ce travail de mise en cohérence de planification au sens concret du terme a bénéficié des temps de confrontation de de propositions, d'une particulière intensité que ce soit d'abord le livre blanc sur la sécurité intérieure et le Beauvau, la sécurité, ça nous permet, mes chers collègues, d'être sûr, au moment d'approuver ce projet que toutes les contributions constructives de tous les partenaires, inspiré par la sécurité et les libertés, les Français ont été entendus et ont pu être intégré à ce grand projet, c'est donc une programmation au sens plein complète et cohérence et sont suivis sera facilitée par le la profondeur du travail qu'il a préparé. C'est d'ailleurs cette qualité de réforme de méthode, pardon, qui a conduit un travail collaboratif d'excellente qualité, entre le Sénat et vous-même, Monsieur le Ministre, sous la conduite de nos rapporteurs qui sont allés au fond des sujets et ont su réunir un consentement large parfois presque unanime sur les dispositions que nous approuvons, enfin 3ème motif de soutenir ce projet de loi, il comporte un ensemble de dispositions législatives dont l'objet commun et de rendre plus efficace la lutte contre la délinquance, en donnant des outils et des marges d'action aux forces de la loi.

Nous étions nombreux. Ah, approuvé le diplôme, le développement des amendes forfaitaires délictuelles qui permet d'appliquer une sanction concrète et immédiate au délit trop fréquents qui contribue à dégrader la vie en société. La proposition du gouvernement était très large, nous avons trouvé, me semble-t-il, un bon accord sur les cas qui sont maintenant donc 24, comme l'a rappelé, lui avait auquel ces amendes seront applicables et ça nous permettra de suivre efficacement cette innovation pour apprécier les projets qu'elle permettra dans le recul de certaines délinquance, nous devons aussi soutenir les modifications justifié justifié à certaines règles de procédure pénale du quotidien qui pèsent sur la charge la trop lourde ne nos enquêteurs et qui allonge les opérations sans bénéfice pour l'équité du projet Et je veux souligner, sur ce point que on peut être vraiment en désaccord avec l'idée que tout le code de procédure pénale, telle qu'il est alors que c'est une accumulation de de modification partielle qui n'ont pas forcément été harmonisées, que l'ensemble serait absolument nécessaire pour garantir les droits il y a au contraire un travail de rationalisation. à faire pour que ce code soit vraiment efficace, c'est ce qui me conduit à exprimer par notre vote positif le soutien et l'admiration que nous voulons adresser à l'occasion de cette loi qui leur est dédié à tous les personnels du ministère qui veillent jour et nuit sur les droits des citoyens merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il va être procédé maintenant dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. N'ouvrira le scrutin dans quelques instants. Le scrutin est ouvert et je vous invite à insérer votre carte de vote dans le terminal.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin, numéro 3 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote Nombre de votants : 336 Nombre de suffrages exprimés 334 pour l'adoption 307 contre 27. Le Sénat a donc allô. Vous avez la parole monsieur le ministre. au Sénat pour son sa contribution et monsieur les rapporteurs, monsieur le président de la commission des lois de l'esprit avec lequel je croyais que tous les groupes, nous avons travaillé dans un esprit monsieur le Président, constructif, me semble-t-il, comme l'a très bien dit, comme l'a très bien dit, les rapporteurs des amendements de tous les groupes ont été adoptés, je me suis engagé envers le président de la commission des lois, ça tombe de choses, notamment en ce qui concerne la réforme de la police nationale, mais aussi les décrets et règlements que je soumettrai à sa sagacité, celle de l'ensemble des commissaires aux lois et à travers lui, bien sûr, à l'ensemble des sénateurs, vous dire que c'est avec le même esprit et porteur de ce compromis républicain, merci également au groupe socialiste de l'encouragement à faire mieux, mais un encouragement positif pour porter à l'Assemblée Nationale le texte qui va effectivement donner 15 milliards de plus à nos forces de sécurité et des moyens à la police, la gendarmerie, je veux dire au rapporteur de Bresse et comme à tous ceux qui sont intervenus que nous n'oublions pas que pour qu'il y ait une bonne sécurité, il faut qu'il y ait une bonne justice et d'autres politiques publiques notamment la loi immigration que ne porteront au mois de janvier prochain, le gouvernement n'esquisse pas un une absence de réponse en vous le disant mais découpe les débats dans des politiques publiques qui, j'espère, ont montré leur efficacité et l'esprit de Concorde que nous avons porté ici, je veux dire à chacune et à chacun que c'est avec le même esprit que nous reviendrons en CMP pour j'espère faire adopter ce texte, merci à l'ensemble de nos collaborateurs également ce la séance monsieur le président, et à l'ensemble de ceux qui ont pu contribuer en amont et en aval de l'adoption et de ce beau score si j'ose dire, pour le bien-être de nos policiers, de nos gendarmes de nos pompiers et de nos agents préfecture. Merci. Merci à nos deux rapporteurs. Et au président de la commission, je vais maintenant suspendre la séance, elle sera reprise à 16 On me dit à 15 heures 45, ce qui laisse un temps très bref, pour l'examen de la proposition de loi visant la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale afin de lutter contre les déserts médicaux. La séance est suspendue pour cinq minutes.

Bien, chers collègues, la séance est reprise. La parole est à monsieur saumon pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, pour une rectification de vote effectivement c'était marqué : je n'ai pas pris part au vote, mais en fait j'ai voté pour, parce qu'il n'y a pas eu une bonne transmission dans le scrutin numéro 3 précédentes. a acte et donnez-nous votre mise au point Monsieur saumon, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale afin de lutter contre les déserts médicaux présenté par Monsieur Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues demande du groupe, les républicains. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais saluer bien sûr, la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche et puis l'excellente rapporteure Corinne Imbert qui a fait un excellent travail, monsieur le Ministre, la France est aujourd'hui le pays des pénuries et des rationnements. Pas seulement pour le carburant ou l'électricité, pas seulement sur un certain nombre de produits alimentaires, cher Laurent Duplomb mais aussi sur des médicaments et, malheureusement, sur l'accès aux soins, cette situation, c'est plus qu'un problème cette situation, c'est une formidable injustice pour des millions de nos compatriotes 6 1000000 300000 Françaises et Français, mais c'est même plus qu'une injustice, c'est un scandale, c'est un scandale quand on met ce chiffre de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant. Ah la dépense que nous avons pour la santé dans notre pays et qu'on la compare ces dépenses, notamment aux pays de l'OCDE, parce qu'il est très élevé, d'où vient, si j'ose dire ce ce scandale, certainement pas des médecins. ça n'est pas leur faute, cette situation procède de choix qui ont été des choix technocratiques et des choix idéologiques d'abord des choix technocratiques, puisque on a abandonné la médecine et la santé, aux mains de comptable et on a pensé à l'époque, il suffirait pour ralentir les dépenses de santé de rationner l'accès aux médecins et de former, de moins en moins de médecin. Le choix idéologique c'est d'avoir tout misé sur une organisation très hospitalo-centrée de notre système de santé, ce qui fait que la médecine libérale, a été mise à mal et ce qui fait qu'aussi la formation de nos jeunes médecins a été très orienté dans justement les facultés de médecine sur autre chose que leur installation en médecine générale, la médecine générale en réalité a subi ces 2 influences qui l'ont finalement extrêmement fragilisé, hé bien le moment, il est venu Monsieur Monsieur Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues, d'y remédier d'y remédier parce que cette conséquence c'est les Français qui la supporte, mais c'est aussi les élus locaux. Ce que je suis venu dire à cette tribune, c'est que beaucoup de merde entre flux parce que, évidemment, ils sont en première ligne et la population leur population dans un village dans une petite ville dans une grande ville, la population rend les maires responsables. Alors que ils ont rivalisé d'un certain nombre de propositions, allant même jusqu'à salarier des médecins ouvrir bien sûr des maisons de santé, nous avons fait aussi avec votre appui du reste des centres de soins non programmés, la situation n'est plus possible, nous ne voulons plus désormais laisser les mères laisser nos compatriotes seul avec ce problème où nous agissons où nous n'agissons pas. C'est ce que propose justement cette PPL pourquoi on en est arrivé là et pourquoi les solutions qui sont actuellement mises en place, il y en a d'ailleurs je pense que il n'y a pas de panacée et qu'on arrivera pas à trouver la seule unique et bonne solution, j'en suis certain, il y a un bouquet de solution mais pardon, les solutions qui sont aujourd'hui en place, ce sont des solutions insuffisante, de déblocage du numerus clausus pardon beaucoup de facultés quand on parle des des doyens n'ont pas les moyens en réalité de former ces nouveaux médecins et puis ensuite ça met 10 ans plus combien d'années d'installation, alors on va attendre, on va tendre, mes chers collègues, 10 ans, 15 ans, non, on ne peut plus attendre, c'est pas possible, il y a d'autres solutions, des aides, y compris des aides des que des collectivités, des aides bien sûr de l'État, mais ces aides, elles viennent trop tardivement, c'est pas d'ailleurs ce que demandent des médecins, c'est pas. C'est juste une rustine et c'est pas une réponse fondamentalement satisfaisante, alors je sais qu'entre un certains nombres de 2 collègues, y compris au sein d'un certain nombres de groupes, certains voudraient la coercition, je me souviens d'un excellent rapport d'un collègue de l'Union centriste Jean Marie Wallenberg, qui nous avait fait un point sur ce que donnait sur les résultats de la coercition sélective du conventionnement sélectif, notamment en Allemagne, je j'invite les uns les autres à à pouvoir en relire les conclusions les conclusions, c'était que, en réalité, avez réguler un petit peu et encore les zones sur-denses et ça n'avait rien fait en zone sous-dense, échec et mat et je crois que, on en conviendra donc, me semble-t-il, la solution n'est pas celle de la coercition, ça n'est pas non plus la solution de palliatives telle que je l'expliquais sur les aides qui existent déjà, parce que elle ne produise pas suffisamment de résultats, la solution elle est quelque part curatif, c'est ce que nous essayons de creuser, nous avons essayé de faire des propositions pour ne pas rester les bras ballants, pour ne pas laisser encore une fois, ni nos compatriotes ni les maires de France, seul face à ce problème, cette solution, elle nous a été aussi inspiré par le fait que le gouvernement puisque dans la loi Buzyn dit en 2019 nous avions voté, vous savez, chers collègues, les six mois de dernière année du 3ème cycle de médecine générale comme étant six mois que les jeunes médecins devaient faire sur le terrain, jamais, jamais, de gauche et de droite, vous pourrez je parle sous votre contrôle, mais le décret n'a été pris, pourquoi jamais le décret d'a été pris, parce qu'on nous a expliqué ben, il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce que il faut laisser les internes dans l'hôpital, donc si vous voulez, nous on a creusé, on a creusé encore une fois, nous voulions des propositions et nous vous proposons cette proposition ce texte là qui est un texte qui est important pour nous, puisqu'il s'agit de créer une 4ème année de consolidation de professionnalisation au 3ème cycle de médecine générale, ça permet un d'installer provisoirement, certes, mais 3500 à 4000 jeunes médecins généralistes sur l'ensemble du territoire en ville ou en rural parce que désormais, c'est la France entière, qui est un vaste désert me médical, ça leur permet d'être rémunérés de façon attractive et nous tenons beaucoup à les rémunérer comme de vrais médecins, avec un paiement à l'acte, ça permettrait aussi aux collectivités de s'engager beaucoup de collectivités ne demanderait pas de mieux que de leur mettre à disposition, par exemple, un logement parce que la question se posera quand on est pendant une année, sur un territoire, c'est, c'est une évidence et ça permettrait surtout aussi de faire en sorte que on puisse faciliter l'installation dans nos territoires urbains ou ruraux pour ces jeunes médecins parce qu'on pense que la formation actuelle ne les prédispose pas ne les incite pas à s'installer quand on lit d'ailleurs les auditions il rapport l'excellent rapport de notre rapporteur oui de ce, je vous le fais pas dire je, on constate d'ailleurs que, il y a peut-être pas l'unanimité, mais il y a quand même un consensus qui s'est établi, j'avais moi-même rencontré l'Ordre national j'avais rencontré les 2 grands syndicats des médecins généralistes et de grands syndicat des des internes, franchement j'avais pas senti une franche opposition donc je pense que la médecine générale, les internes sont les seuls à ne pas avoir cette 4ème année de consolidation depuis que cette médecine générale est devenue une spécialité on pense que là il y a un problème et que cette année de consolidation permettrait d'avoir une meilleure préparation une meilleure incitation à l'installation de ces jeunes médecins à condition qu'on les accompagne, je dis bien entendu qu'il faut un médecin référent, c'est un point que il disait : il est important, en tout cas de de souligner et puis ensuite de mettre effectivement en oeuvre ce que je voudrais dire pour terminer, c'est une proposition qui est importante, j'ai vu que et nous avons vu, vous m'aviez d'ailleurs appelé que vous l'avez en quelque sorte, reprise dans le PLFSS je pense que vous l'avez fait de façon précipitée, sans beaucoup de concertation et sans en définir les modalités, ce qui a pu je pense raidir un certain nombre de syndicats notamment d'internes, je pense aussi que la façon dont elle a été rédigée vous fait courir le risque d'une disposition anti-constitutionnelle dans la mesure où elle n'importe pas vraiment les finances de la Sécurité sociale, peu importe en quelque sorte cette proposition de loi d'une séance de rattrapage et je suis très heureux de pouvoir y contribuer utilement je pense mes chers collègues, que quand on choisit et je sais qu'un certain nombre ont choisi parmi vous ce métier quand on choisit de devenir médecin, on fait plus que choisir un métier, Monsieur le Ministre, vous êtes médecin ont choisi, non pas seulement une vocation mais une mission de service public et je pense que c'est aussi au regard de cette mission de service public que nous devons examiner cette proposition de loi, j'y crois beaucoup et je pense que ça nous oblige nous à parlementaire à bouger, à voter, à faire des propositions, ça vous oblige vous l'exécutif aussi consolider ses propositions et ça oblige quelque part les jeunes médecins quand ils s'investissent dans ce beau métier à considérer que on ne peut pas laisser des millions de Français vraiment sans médecin traitant, c'est une prise de responsabilité, nous la prenons aujourd'hui nous la prenons je pense avec une forme de courage avec beaucoup de sincérité, vous devez la prendre aussi et le monde, le évidemment doit l'apprendre, je pense que c'est fondamental, il y a cette réforme, elle est à la fois elle est nécessaire et je crois aussi qu'elle est urgente, merci de votre attention. Merci monsieur le Président Retailleau et la parole est maintenant à Corinne Imbert, rapporteure de la commission des affaires sociales. monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la président, l'excellent président Bruno Retailleau est inscrite à l'ordre du jour, à la demande du groupe, les républicains, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, poursuit 2 objectifs auxquels la commission des affaires sociales a pleinement souscrit. Le texte vise d'abord à améliorer la formation des médecins généralistes en allongeant d'un an, le troisième cycle de cette spécialité, cette nouvelle année voulu professionnalisante doit permettre de mieux accompagner les étudiants dans la découverte de l'autonomie et de l'exercice ambulatoire mais ce faisant, le texte vise également à trouver un moyen d'action nouveaux pour s'attaquer à la problématique de l'accès aux soins et j'y reviendrai. L'article unique de la proposition de loi porte sur la durée du 3ème cycle des études de médecine générale, elle le porte à 4 ans et affecte la quatrième année à la réalisation d'un stage en ambulatoire et en autonomie superviser cette mesure est envisagée depuis plusieurs années, la durée du 3ème cycle de médecine générale rester fixé à trois, en fait en effet figure d'exception, ceux des 43 autres spécialités s'étendent tous sur 4 à 6 années, elle empêche la médecine générale de bénéficier de l'ensemble des avancées de la réforme du 3ème cycle des études de médecine, intervenue en 2017 et l'isole des autres spécialités ainsi les futurs médecins généralistes sont les seuls à ne pas bénéficier de la 3ème phase d'internat, dite de consolidation visant à consolider les connaissances et compétences acquises jusque-là par les étudiants, ils ne bénéficient pas non plus du statut de Docteur junior associés à cette dernière phase et permettant aux étudiants de réaliser pendant une année entière des stages en autonomie progressive et superviser tout en bénéficiant d'une meilleure rémunération enfin alors que la soutenance de la thèse d'exercice constitue désormais l'une des conditions d'accès à la phase de consolidation et donc souvent réalisés dans les délais, les étudiants de médecine générale ne bénéficie pas de cette incitation : les retards de soutenance sont fréquents et reporte d'autant l'installation des jeunes médecins généralistes. La durée du 3ème cycle de médecine générale est établi sur le minimum fixé par l'Union européenne et s'avère plus courte que celle retenue dans de nombreux autres pays les médecins généralistes suivent par exemple la 3ème cycle de 5 ans au Danemark, en Suède ou en Norvège, les enseignants et médecins que nous avons auditionnés sont majoritairement très favorable à cette mesure, plusieurs d'entre eux nous ont indiqué, il travaillait depuis plusieurs années, ils ont insisté sur l'opportunité d'enrichir les référentiels de formation la maquette actuelle ne comprend pas suffisamment de stages en ambulatoire, alors que ce mode d'exercice constitue un débouché naturel pour la médecine générale, seuls de dépistage prévus sont obligatoirement réaliser en ville sont pourtant ces stages qui prépare le mieux les étudiants l'exercice libéral en leur donnant une expérience concrète du fonctionnement d'un cabinet ou d'une structure d'exercice coordonné. La mise à jour de la mafia devrait aussi permettre aux étudiants qui le souhaitent d'approfondir plus facilement des compétences spécifiques commune à plusieurs spécialités. En améliorant la professionnalisation des internes de médecine générale, la proposition de loi vise ainsi à favoriser leur installation rapide, l'ajout d'une phase de consolidation encouragera les étudiants à soutenir leur thèse des déçus de la troisième année, ne pourront plus comme aujourd'hui la reporté jusqu'à 3 ans après la fin de leur internat surtout la réalisation d'une année entière de stages en ambulatoire et en autonomie, supervisée par mettra d'améliorer largement la professionnalisation des étudiants et de mieux les préparer à l'exercice en ville en elle-même d'extension du 3ème cycle portées par le texte devrait donc être favorable à l'amélioration de l'offre de soin toutefois la proposition de loi ne s'arrête pas là, afin de répondre plus directement aux problèmes d'accès aux soins dans de nombreux territoires dont de très nombreux territoires, elle prévoit que les stages en ambulatoire de quatrième année seront prioritairement réalisées dans les zones sous-denses, identifié par les agences je régionales de santé. Cette mesure a concentré ces dernières semaines, les inquiétudes des organisations représentatives des internes qui ont craint que la formation soit instrumentalisée pour régler les difficultés d'accès aux soins, je tiens donc à lever toute ambiguïté président Retailleau vient aussi de le rappeler, le texte que nous examinons aujourd'hui n'entend pas sacrifier la qualité de l'encadrement des étudiants ni celle de leur formation, au contraire, il prévoit que les stages de quatrième année seront comme les autres, supervisé par des maîtres de stage formés et agréés par l'université, ils devront permettent de mieux accompagner les étudiants dans la découverte de l'exercice ambulatoire et la préemption progressive de l'autonomie. Afin de tenir compte des inquiétudes manifestées par les organisations d'étudiants et parce que l'expression désert médical ne lui a pas paru décrire fidèlement la réalité contrastée, il est vrai, et des zones sous-denses, la Commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi afin de mettre en valeur son objectif 1er, l'amélioration de la formation des internes en médecine générale, malgré tout je crois évidemment qu'il n'est pas possible d'ignorer entièrement les besoins de santé ne d'autres territoires dans l'affectation des internes en stage, l'accès à un médecin généraliste, constitue un enjeu majeur pour nos concitoyens, or la démographie de la profession est particulièrement sinistré, la France a perdu en 10 ans, environ 5000 généralistes, la diminution de la densité médicale aggrave les inégalités. Territoriales d'accès aux soins, la suppression du numerus clausus et l'augmentation du recrutement d'étudiants ne mère ne permettront pas de résoudre cette situation avant plusieurs années. C'est pourquoi je crois au contraire que les affectations doivent être cohérente avec les besoins de santé des territoires, chaque fois que cela est possible sans perte sur la qualité de l'encadrement des étudiants. Afin d'assurer la pleine efficacité de cette mesure, les efforts devront être poursuivis pour augmenter encore le nombre de maître de stage, universitaires et s'assurer que ceux-ci mailles suffisamment le territoire, il s'agit d'un enjeu central hé bien identifié à ce titre des collectivités territoriales sont déjà employé à favoriser l'augmentation du nombre de mettre du maître de stage, ces dernières années en facilitant en accord avec les facultés de médecine, l'organisation des formations de maîtrise de stage au plus près du lieu d'exercice des médecins généralistes, c'est-à-dire la condition de concilier ces 2 impératifs : amélioration de la formation des étudiants, d'une part et amélioration du service rendu à la population dans les territoires, d'autre part que la réforme sera un succès, ce texte est un pas indispensable en faveur d'une meilleure réponse aux attentes de soins de nos concitoyens, il a deux mérites celui de démystifier l'installation en favorisant une meilleure connaissance de l'exercice en cabinet mais également celui de démystifier la notion de zone sous-dense, il y a une vie dans ces territoires, mes chers collègues, et vous le savez tous un 2ème motif d'inquiétude réside dans la situation matérielle des étudiants dont l'affectation serait éloigné de leur domicile. Les collectivités territoriales font déjà beaucoup d'efforts dans ce domaine, je constate, par ailleurs, Monsieur le Ministre, que le gouvernement a souhaité ouvrir une concertation dans le cas d'une mission interministérielle et n'est pas fermé à l'idée de modalités de rémunération spécifique à la médecine générale, je crois même que c'est indispensable, les docteurs juniors, quand bien même ils exercent en autonomie progressive sont aujourd'hui rémunérés forfaitairement et il faut le dire. Assez faiblement au regard du travail qu'ils accomplissent, je souhaite, comme le président Retailleau que des solutions puissent être trouvées pour étirer buée justement les étudiants de médecine générale qui suivront cette année supplémentaire et leur permettent de réaliser leur stage sans difficulté s'agit une condition essentielle à la réussite de cette réforme. Enfin, les organisations que nous avons entendu nous ont tous confirmé que l'ajout d'une 4ème année ne devraient pas s'appliquer aux étudiants actuels du 3ème cycle de médecine générale pour ne pas nuire à la cohérence de leur formation, la commission a donc adopté un amendement en ce sens, prévoyant que le dispositif ne s'appliquera qu'aux étudiants qui, à la date de la publication du texte n'auront pas encore débuté le troisième cycle se ce délai doit également permettre, monsieur le ministre, de prendre le temps nécessaire avec les parties prenantes pour établir le nouveau référentiel de formation, j'ai pu constater lors de mes auditions que la plupart d'entre elles, il avait déjà beaucoup travaillé Dray maintenant m'attarder sur le contexte dans lequel intervient l'examen de ce texte, votre gouvernement a repris, Monsieur le Ministre, l'essentiel de son dispositif pour l'inclure au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre dernier alors même que la proposition de loi que nous examinons cet après-midi était dépose au Sénat depuis janvier et inscrite à son ordre du jour, elle s'inspire, vous le reconnaîtrez d'ailleurs de nos travaux et comme l'a rappelé le le président Retailleau, en effet, nous avons adopté dès 2019 les chers collègues, un dispositif qui prévoyait que les étudiants de médecine générale réalise lors de leur 3ème année d'internat, un stage d'une année en pratique en bu là. En autonomie superviser en priorité dans les zones sous-denses stage qui a été ramené à au moins un semestre à l'issu de la CMP, cette disposition n'a jamais été appliquée par le gouvernement qui n'a pas pris les décrets nécessaires, malgré les promesses données dans cet hémicycle, la proposition de loi reprend aussi une recommandation du rapport de la commission d'enquête relative à la situation de l'hôpital qui proposait, je cite. De renforcer la formation en médecine générale par une 4ème année d'internat en priorité dans une zone sous- dense je je crois enfin que la proposition de loi du président Bruno Retailleau constitue Monsieur le Ministre, le véhicule le plus sûr pour adopter cette mesure non pas seulement parce qu'elle est antérieure au projet de loi de financement de la Sécurité sociale est issue de nos travaux, mais aussi parce que l'article 23 du PLFSS qui porte cette réforme n'est pas conforme à la loi organique en effet l'absence l'absence d'incidence financière de la mesure sur les régimes obligatoires de base est mise en évidence par l'étude d'impact, établi par le gouvernement lui-même, c'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter cette proposition de loi, elle constitue. Que le meilleur moyen de mettre en oeuvre cette 4ème année qui permettra d'améliorer à la fois la formation des étudiants de médecine générale et surtout l'accès aux soins dans nos territoires, je vous remercie. Merci madame la rapporteure et maintenant la parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la prévention. Merci. Monsieur le président, madame la présidente de la commission madame la rapporteure mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui pour l'examen d'une proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale. Cette proposition de loi porte sur un sujet qui me tient, vous le savez très à coeur, à savoir la qualité de formation de nos futurs médecins généralistes, d'une part et la lutte pour l'accès à la santé dans l'ensemble du territoire, d'autre part. Cette proposition qui fait écho à l'article 23 du Plfss pour 2023 actuellement en cours d'examen répondent donc à 2 enjeux distincts. Je parle bien d'enjeux distincts, car la proposition gouvernementale qui fait suite à un engagement de campagne du président de la République ne vise en aucun cas envoyer des internes en médecine, faire des stages dans des territoires pour boucher les trous, et ce sans encadrement. Elle vise au contraire par l'accession au statut de Docteur junior pour les futurs médecins généralistes à renforcer la formation des internes pour leur permettent d'être en sortie de diplôme autonome et plus à même de gérer une installation, un cabinet médical. C'est bien, et j'insiste là-dessus l'objectif 1er de cette proposition. Et si pour aider nos territoires, nous souhaitons en priorité envoyer ces jeunes médecins vers les zones sous-denses, cela ne se fera aucunement au prix de la qualité de l'encadrement, à ce titre-cette séance d'examen législatif qui nous réunit aujourd'hui est un moment bienvenue pour nous permettre, à quelques jours du début de l'examen du PLFSS en séance publique de rappeler dans quel cadre de la proposition gouvernementale s'inscrit. Je remercie donc le président Bruno Retailleau, ainsi que l'ensemble des sénatrices et sénateurs, cosignataire de cette proposition de loi de nous permettre de débattre et d'échanger sur cet enjeu crucial. La quatrième année d'internat de médecine générale, part d'un constat ancien et partagé. Sans la phase de consolidation qui définit le statut de Docteur junior l'installation immédiate en sortie de cursus n'est pas facile, elle devient même rarissime, l'objectif de la mesure gouvernementale et de la vôtre s'inscrit dans le même état d'esprit si j'en juge l'amendement, de modification du titre de la proposition de loi adoptée en commission et donc d'améliorer la formation des jeunes médecins tout en facilitant leur installation à l'issue de leurs études. Non pas pour envoyer au front des jeunes recrues mais pour parfaire une formation polyvalente et exigeante. J'y tiens beaucoup cette 4ème année de formation et de professionnalisation sera assortie d'un projet pédagogique co-construit avec toutes les parties prenantes, dont les internes même. même. Concrétisera par des stages en pratique ambulatoire auprès de maître de stage universitaire expérimenté et capable d'encadrer, de transmettre leur expérience et leur savoir-faire. Je souhaite que cette réforme soit mise en oeuvre dans les meilleures conditions à cette fin, nous avons lancé récemment une mission avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau cette mission permettra, avec l'appui de 4 professionnels de terrain reconnu de conduire la concertation que requiert un tel engagement tant en ce qui concerne les dispositions de leur hébergement, vous en avez parlé mais également les dispositions de leur rémunération. Comme le dispose l'article unique de la proposition de loi, nous souhaitons que ces stages soient effectuées en priorité, sans que cela ne soit une obligation dans les zones sous-denses afin aussi de faire découvrir ce mode d'exercice au futur de médecin qui n'ont pas forcément eu l'occasion d'y exercer dit suivre un enseignement pendant le cours de leurs études. Les inégalités d'accès à la santé sont intolérables et nous devons agir résolument contre elle, aujourd'hui, vous l'avez dit, monsieur le Président, 6 millions de Françaises et de Français restent sans médecin traitant, parmi eux 600000 personnes souffrent d'une affection de longue durée, cela concerne les médicaments également beaucoup de nos concitoyens précaires ou vivant avec un handicap. Cette situation n'est pas acceptable, surtout qu'elle est très inégale selon les territoires. J'étais il y a 2 semaines, dans la Sarthe pour le lancement du Conseil national de la refondation santé qui a vocation à faire, se concerter, l'ensemble des parties prenantes du secteur pour que nous trouvions collectivement des solutions pour qu'il n'y ait plus aucun laissés pour compte en matière d'accès à la santé. Là-bas, pour ne citer que cet exemple, le nombre de médecins généralistes libéraux et de 59 pour 100000 habitants, bien en dessous de la moyenne nationale de 85 pour 100000. Ce déficit de médecins généralistes traitants dans certains territoires et d'autant plus problématique qu'joue un rôle essentiel de suivi de proximité tout au long de la vie. Nos médecins généralistes traitants sont aussi des aiguilleurs de notre système de santé puisqu'ils orientent les patients et assure la nécessaire coordination de leur parcours de soins. Surtout, cette situation a des conséquences sur l'ensemble du système de santé. La situation des urgences que je connais bien, qui sont devenus pour beaucoup un 1er recours le montre, puisque leur fréquentation a augmenté de plus de 50 % en 20 ans. Mais lorsque tout s'organise, ville et hôpital comme avec les mesures prises cet été, elle chute enfin pour la première fois de 5 %. Nous devons par responsabilité à l'égard de nos concitoyens, prendre des mesures fortes, vous l'avez dit. La création d'une 4ème année d'internat de médecine générale s'inscrit ainsi dans tout un arsenal de mesures du PLFSS qui vise à renforcer l'accès à la santé à travers nos territoires. Je pense par exemple la création d'un cas donc plus adapté pour les négociations conventionnelles qui devra nous permettent de mettre en place des engagements réciproques au service des Français dans tous les territoires, notamment les moins dotés, dans une logique de droits et de devoirs. Je pense aussi à la simplification des aides pour l'installation de nos médecins dans les zones sous-denses pour intensifier leur impact, enfin, je tiens à souligner le fait que nous allons pouvoir tirer des des fruits dans les prochaines années des réformes déjà engagées dans le quinquennat précédent, vous l'avez cité la suppression du numerus clausus, mais qui effectivement n'aura d'effet que dans une dizaine d'années. Cette réforme importante et nécessaire. Que nous aurions dû prendre il y a 10 à 15 ans devrait permettre d'inverser la dynamique de la démographie médicale et de renforcer nos bataillons de médecins généralistes comme spécialistes. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je le pense profondément cette 4ème année ne serait pas seulement une chance pour nos territoires sous-dotés, c'est aussi une chance pour nos jeunes médecins et in fine et pour les patients. Oui, cette année supplémentaire leur permettra de bénéficier d'une phase bienvenue de consolidation dans leur formation, à l'instar de ce qui est fait dans les autres spécialistes. C'est à mon sens la clé d'une mise en responsabilité progressive et superviser, vous l'avez dit, pour accompagner le mieux possible, nos jeunes médecins généralistes vers leur installation. Elle traduit la volonté exprimée dès le début de ma prise de fonction des solutions concrètes et pragmatiques pour répondre aux défis auxquels notre système de santé fait face je partage donc avec les auteurs de la proposition de loi, le fond de ce qui est proposé. Cependant, comme vous le savez, le gouvernement a choisi de faire prospérer cette mesure via le Plfss pour 2023. C'est pourquoi le gouvernement apporte un avis de sagesse bienveillante à la proposition de loi du président Retailleau je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi du groupe, les républicains visant la formation des internes en médecine générale permet d'avoir un débat sur les réponses publiques à apporter face aux difficultés d'accès aux soins, merci à la rapporteure Corinne Imbert pour son travail, comment accepter en effet que 30 % de la population française vit dans un désert médical, la difficulté, pour prendre un rendez vous avec un généraliste en secteur 1 n'est plus une situation spécifique aux territoires ruraux, elle concerne désormais également les territoires péri-urbain et urbain ainsi la région Île-de-France et le 1er désert médical de France 62 4 pour 100 de la population francilienne, soit 7,6 millions de personnes ont du mal à accéder à des médecins, trop peu nombreux, les maires sont soumis à rude épreuve pour trouver une solution coûte que coûte, il faut redire que depuis 20 ans, les gouvernements successifs ont refusé de supprimer le numerus clausus, et d'augmenter le nombre d'étudiantes et d'étudiants en médecine, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn reconnaissait elle-même dans une tribune du journal Le Monde que le numerus clausus avait été desserrer de façon trop progressive et que, je cite : on a perdu plus de quinze depuis 2017, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pourtant pas corrigé la tendance puisque le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus n'a pas significativement augmenté le nombre de médecins formés, faute de moyens financiers et humains supplémentaires pour les universités, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en médecine est passé de 9300 en 2020 à seulement 11180 en 2021 alors que les besoins sont plus importants, la population plus nombreuse, les patients plus âgés et souvent atteints de poly-pathologies dans ce contexte, la proposition de loi du groupe, les républicains d'ajouter une 4ème année pour les internes en médecine, non seulement ne résoudra rien, mais au contraire va démotiver et précarité, j'ai les internes tout d'abord sur la méthode, l'ajout d'une dixième année d'études sans avoir ouvert de négociations avec les internes revient à mettre la charrue avant les boeufs, une réforme de la formation des internes nécessiterait de discuter du contenu pédagogique et du rythme des études de réfléchir à la prise en compte de l'épuisement professionnel qui touche les 2 tiers des internes à la revalorisation de leur statut aux mesures pour lutter contre les comportements sexistes lors des stages dénoncée par l'association des étudiants de médecine, je veux rappeler ici qu'un interne environ 3 fois plus de risques de se suicider, jeune du même âge et qu'en 2021 il y avait eu une campagne protège en interne à ajouter une dixième année d'étude prouve bien que cette proposition de loi étant déconnexion totale avec la réalité des internes, d'autant qu'elle ne réglera ni la pénurie des médecins ni l'aspiration des jeunes, des qui souhaitent, à juste titre, pouvoir pratiquer la médecine en conciliant davantage leur vie familiale et personnelle aujourd'hui la majorité des nouveaux médecins aspirent à exercer leur activité, de manière salariés en équipe et dans un territoire muni d'un hôpital de proximité, et non pas en libéral comme le privilégie cette PPL il faudrait donc favoriser la réalisation de stage et l'installation dans les centres de santé, l'incitation effectuer des stages dans les territoires sous-dotés ne va pas entraîner mécaniquement l'arrivée de 3900 interne dans les déserts médicaux, les incitations fiscales à l'installation démontré leurs limites, puisque seulement 400 médecins parents sollicite les 50000 euros proposés pour s'installer dans un territoire sous-doté, les internes qui souhaiteraient effectuer un stage dans un désert médical devront être encadrée par un médecin senior alors que par définition les déserts médicaux sont dépourvues de médecin ou pour le moins manque de médecins disponibles de plus, l'ajout d'une année supplémentaire en stage va créer une année blanche d'installation de nouveaux médecins, enfin les critères d'attractivité pour les jeunes médecins sont cruellement défaut puisque les politiques d'austérité menées ces dernières années, y compris par la droite, mon cher collègue, Bruno Retailleau ont entraîné la fermeture des hôpitaux et maternités de proximité et la disparition des services publics de proximité, selon nous, la réponse politique est multiple, mais dans le temps qui m'est imparti, je vais privilégier 4 propositions qui me semble majeur : l'augmentation des moyens des universités pour former davantage de professionnels de santé, le développement des centres de santé, le rétablissement de la permanence médicale de nuit et le week-end en abrogeant le décret Mattéi et en revalorisation, les gardes de tous les soignants dans le public comme dans le privé, mise en place d'conventionnement sélectif dans les zones surdotées, mes chers collègues, vous êtes loin du compte, avec votre PPL aussi les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen écologistes voteront contre cette proposition de loi, tout comme nous voterons contre l'article 23 du PLFSS. Monsieur le Ministre, qui prévoit le même dispositif, je vous remercie. Bien, merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission madame la rapporteure, mes chers collègues, il y a quelques semaines, nous a été soumis une proposition de loi visant, je cite, à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale afin de lutter contre les déserts médicaux, les démarches qui consisterait à proposer une modification de leur formation uniquement dans le but de lutter contre les déserts médicaux nous semblerait inadaptés, on n'envoie pas les jeunes dans des déserts pour réparer des erreurs dont ils ne sont pas responsables, le poids des mots, ce n'est pas rien, il est grand temps d'en changer certains j'habite moi-même dans une région où l'angoisse des patients et des soignants et grande l'accès aux soins et le problème sans doute l'origine d'un sentiment d'abandon dramatiquement vécu par les habitants et les électeurs, on ne peut ignorer l'attente des territoires, les travaux que nous avons menée avec Hervé Maurey et Jean-François Longeot l'ont démontré, mais ce ne sont pas des déserts de nouvelles manières de travailler, il amène de nouveaux habitants des projets émergent des soignants, ils viennent aussi en nombre insuffisant, hélas, mais de leur plein gré et avec un vrai projet de vie, les jeunes médecins ne construisent pas leur vie pour des primes, ils construisent leur vie en cherchant à s'épanouir professionnellement et personnellement, donc pas de désert, pas de punition en ce et ceux notre commission l'a bien compris puisqu'elle a veillé à présenter en séance une proposition de loi désormais intitulé : proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale, si cette initiative de Bruno Retailleau et nos collègues est une proposition pour orienter la formation des jeunes praticiens vers plus en mille Bulat à Thouars, alors c'est intéressant et ce doit être soutenu les autres spécialités se font dans 4 années il y a une forme de logique à aligner celle-ci considéré que la médecine générale est une spécialité pleine et entière, exigeant une phase longue de pratiques de terrain qui est au fond la meilleure des écoles, une année de Docteur junior qui, pour la rendre pleinement attractif devra être assortie d'une juste rémunération, un peu comme certains d'entre vous l'ont sans doute connu ses mois ou années que faisaient les jeunes médecins généralistes en remplacement, ici et là, le temps d'écrire la thèse avant de se fixer pour de bon, dans un communiqué d'un regroupement de généralistes jeunes installés, remplaçant, voici ce que je lis, nous témoignons tout notre soutien à nos futurs confrères en formation, nous réclamons pour une formation de qualité et une phase de consolidation qui les accompagne réellement de leur la construction de leur projet, oui il est indispensable que cette 4ème année soit une plus-Value dans le groupe Union centriste, les avis sur ce texte sont sont majoritairement favorables, si je le voterai moi même, je sais que certains de mes collègues, émettent des réserves sur le nombre potentiellement insuffisants de maître de stage sur la nécessité d'une plus grande concertation sur le besoin d'enseignants en médecine générale sur le risque d'une coercition déguisé par le passé comme conjoint collaborateur d'un médecin généraliste, j'ai accueilli moi même dans mon foyer de jeunes internes en fin d'études pour des sessions de quelques semaines, je sais combien ces séjours à ce moment-là de leur vie à la découverte d'un territoire au contact de ses habitants peuvent être déterminants, 3 de ses stagiaires, se sont installés près de chez nous une année pleine et entière en autonomie aurait certainement eu des effets encore plus significatif, donc j'y crois, mais avec des réserves, cependant, en effet, quid des maîtres de stage pour connaître les médecins généralistes de la Nièvre, donc mon département et leur charge de travail, je sais que les sessions de formation sur Dijon, 2 heures et demie de route aller sur des journées entières qui reviennent régulièrement c'est très dissuasif si certaines sessions sont depuis la crise sanitaire en distanciel celles qui subsistent en présentiel doivent absolument être organisées au plus près des médecins dans tous les départements, comme cela commence à se pratiquer en de rares endroits ces possibilités doit se généraliser et c'est à ce prix que de nouveau maître de stage universitaire viendront grossir les rangs actuellement l'ambulatoire est déjà au programme du DES de médecine générale, mais il est insuffisamment mis en oeuvre faute parfois de lieu de stage et parfois, hélas, parce que les internes aussi reste dans les CHU, pour pallier les manques de personnel, c'est qu'il est tout à fait inadmissible cette réflexion autour de l'ambulatoire d'être, elle doit être globale, concerner également les spécialistes : ne pas rester théorique s'inscrire, peut-être dans un vaste chantier de refonte des études médicales, en s'inspirant d'autres modèles voisin reste l'épineux sujet du lieu de ces stages puisqu'il est désormais acquis que c'est presque tout le territoire national qui est en zone sous-dotée, les internes, M. les stages intéressants, mais en fin de cursus, ils peuvent aussi avoir des charges de famille et des ancrages que l'on comprend aisément le lieu de vie pendant une année entière, après de longues études, ce n'est pas rien l'idéal sera alors qu'il puisse se diriger vers une région probablement sous-dotés aussi puisqu'elles sont presque toutes où ils ont peut-être déjà une attache, voire même un début de projet quatrième année ne doit pas impliquer territoire inconnu, pas plus que des airs ou punition il faut prévoir de la souplesse dans les affectations, ce qui m'amène à un autre sujet essentiel, celui de l'origine géographique des étudiants pour prendre encore le cas de ma région, si tous ceux qui réussissent le concours de médecine à Dijon sont de jeunes Dijonnais qui ont bénéficié d'une prof X imiter familial et et d'un contexte connu et familier, il semble difficile sauf coercition de venir les voir s'installer en milieu rural, c'est pourquoi il est capital que les formations se délocalise ne se cantonne pas aux grandes villes universitaires et viennent au plus près des territoires, c'est en partie les années pendant lesquelles nous n'avons formé que de jeunes urbains que nous payons actuellement une faculté de médecine est en train de se se mettre en place à Orléans la passe santé premières années d'études de médecine à Nevers, obtenu après de longues années de bataille, a permis à 50 % des étudiants de réussir le concours, voilà une vraie solution et il y en a d'autres en France les déserts médicaux sont tout simplement des déserts de formation, il en faut plus, monsieur le ministre, il faut que le numerus apertus mutant numerus Proximus voilà ce que la proposition de Bruno Retailleau, m'a permis d'exprimer si cette disposition est votée, alors il faudra que les moyens soient là et le décret d'application parce qu'il y a des précédents, Monsieur le Ministre, vous partagez le même objectif, à l'article 23 du PLFSS justifiant que la mesure aurait un impact sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concurrents à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes toutefois au chapitre impact financier global de l'étude d'impact votre dispositif n'a aucun effet sur l'Europe, je ne doute pas, ce que ce que je vois le Conseil constitutionnel le verra aussi aussi je vous invite à vous saisir de ce véhicule législatif je termine en reprenant une réponse du ministère à une question que j'avais posé en 2019 sur les stages des internes en médecine, la ministre des solidarités et de la santé est extrêmement attaché à favoriser le développement de la maîtrise de stage ambulatoire, les débats qui ont eu lieu avant l'adoption de la loi du 24 juillet 2019 ont rappelé combien à la diversification des lieux de stage, constitue une nécessité pour permettre aux étudiants, futurs médecins de se former et de découvrir un large spectre de situation professionnel alors souhaitons que la loi de 2022 puisse mettre en place en mieux ce que la loi de 2019 n'avait pas vu aboutir, je vous remercie.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, et bienvenue en France, le pays qui prétend posséder le meilleur système de santé au monde, mais qui abandonne plus de 10 pour 100 de sa population, soit 8 millions de personnes dans les déserts médicaux, même si, désormais, certaines grandes villes se trouvent sous dotées en raison principalement de l'insécurité qui y règne, comme dans les quartiers nord de Marseille, où la patiente, elle ne manque pourtant pas puisqu'elle vient des 4 coins du monde et même plus précisément du tiers-monde les déserts médicaux se concentre principalement en ruralité le désert n'est pas que médical, il y est, comment voulez-vous qu'un médecin, il s'installer avec sa famille dans un endroit où s'accumulent les problématiques de mobilité, de logement, d'emploi ou dont on disparu, les écoles et les commerces, faute d'une véritable politique d'aménagement du territoire, de plus, une aggravation inéluctable de cet état de fait état venir un généraliste sur 2 est âgé de plus de 60 ans et partira bientôt à la retraite, le vieillissement général de la population va rendre l'abandon plus criant encore les pénuries énergétiques et d'inflation puisqu'il rompt ces phénomènes, car l'assurance maladie rembourse les consultations mais pas les trajets pour s'y rendre, chez moi, dans les Bouches-du-Rhône, la disparition de SOS Médecins dans les communes rurales a pour conséquence moins de visites à domicile, et plus de médecins disponibles et le week-end et les jours fériés, cela engendre une surcharge ambulancière supporté par le SAMU et les SDIS déjà sous tension, les meilleurs sont le dernier influx nerveux d'une ruralité exangue beaucoup débloque des aides incitatives, malgré cela, les maisons de santé pluridisciplinaires se retrouvent souvent sans médecin face à une telle situation, c'est tout un panel de soutien à la ruralité, qu'il faut repenser, mais avant toute chose, il faut réintégrer les soignants non vaccinés leur suspension, qui était déjà un scandale n'est vraiment plus n'a vraiment plus aujourd'hui aucun sens pour en venir au coeur de la PPL les internes en médecine ne peuvent pas être les variables d'ajustement des carences de l'État, ce sont déjà eux qui font tourner l'hôpital en quatrième année d'internat, les étudiants ont entre 27 et 30 ans, certains ont déjà fonder une famille, on ne peut pas leur imposer une année supplémentaire après 10 ans d'études sans qu'ils sachent où ils sont affectés surtout en les payant 8 euros par mois euros pas à l'heure, pardon, c'est c'est déjà peu cette mesure coercitive sur un an, pose également un problème de suivi des patients ou est chers collègue Retailleau président Retailleau. Excellent président Retailleau, comme le veut la formule consacrée, où est la mission de service public que vous évoquiez tout à l'heure pour justifier votre texte, un texte qui relèvent plutôt de la philosophie macroniste un texte que l'on retrouve d'ailleurs, allez savoir pourquoi dans l'article 23 du projet de loi de finance de la Sécurité sociale présenté par le gouvernement pour conclure, je voterai contre cette mesure palliative administrer à un système en état de mort annoncée, je suis pour une une partisan d'une réforme en profondeur en faveur de la ruralité une méthode demandent à être mieux exploiter celle du contrat d'engagement du service public, il aide les médecins à s'installer dans les déserts médicaux à hauteur de 1200 euros par mois, le nombre des CESP recolle évolue chaque année et je conclus, merci Monsieur le Président, faisons en sorte, faisons en sorte que ce dispositif soit plus connu en attendant de reconstruire l'attractivité de notre territoire. Merci, cher collègue, et la parole est désormais à notre collègue Véronique Guillotin, pour le groupe RDSE. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de commission madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi à l'initiative de Bruno Retailleau et d'un certain nombre de ses collègues nous invite à nous saisir de la question essentielle de la formation des médecins, elle doit répondre à la fois à l'acquisition d'une somme importante de connaissance d'un savoir-être et surtout de la préparation des jeunes médecins à leur futur exercice professionnel qui, pour les généralistes se fera majoritairement sur les territoires en libéral, la question n'est pas tant d'aligner le nombre d'années de la spécialité médecine générale sur celle des autres spécialités mais plutôt et surtout de savoir pourquoi on ajoute une trois et une année supplémentaire et une trois au 3ème cycle d'études médicales s'il s'agit de déployer un bataillon de Docteur junior sur des territoires sous dotés, afin d'apporter une réponse politique à la problématique complexe des déserts médicaux, je n'y serai pas favorable car, en effet, le doute persiste sur la finalité de cette PPL du fait du titre initial de la proposition de loi de la commune de la communication qui a été fait autour de cette mesure, des discussions qui ont eu lieu en commission et en audition jusqu'à l'exposé des motifs de la PPL qui commence en évoquant la question des déserts médicaux, alors que la discussion est entamée depuis plusieurs années déjà, sur cette question que les étudiants, professeur et doyen n'y était pas, il n'y sont toujours pas fermement opposé la finalité à peine masquée de cette mesure a suscité beaucoup d'inquiétude, si l'accès aux soins doit mobiliser chacun d'entre nous, je ne crois pas aux mesures de coercitive, même en celle qui se drape près de bonnes intentions et d'autant plus dans un contexte de manque de professionnels, doit-on rappeler qu'en 10 ans, la France a perdu 5000 médecins généralistes qu'en 20 ans leur densité sur les territoires, a baissé 2 fois plus que celle des autres spécialités et que 84 % de notre pays et dissous doté, aucune réforme des crèmes mesure plan non réglées, ne régleront de manière isolée, à elle seule, la problématique de l'accès aux soins, tant le temps que le nombre de médecins généralistes en exercice n'aura pas augmenté de manière significative par une amplification nette du numerus apertus mais, surtout, du nom du % du quota de médecin généraliste dans la sélection vers les spécialités alors si cette année supplémentaire doit voir le jour, ce dont il faut parler, c'est bien de pédagogie de professionnalisation et d'une meilleure adaptation de la formation au coeur de métier de la médecine générale, une 4ème année professionnalisante bien pensé concertée pourrait et devrait mieux préparer les jeunes à la réalité du métier qui se fait pour l'essentiel, je l'ai déjà dit en libéral et, de fait, si elle est bien menée, elle favorisera les installations sur les territoires, je suis convaincu que cette 4ème année avec un stage obligatoire en ville, mais aussi un stage Libre dans un hôpital de proximité par exemple répondrait mieux aux exercices qui sont aujourd'hui plébiscités par les jeunes et au décloisonnement ville hôpital que l'on appelle tous de nos voeux, j'y vois aussi un autre Avantage : les étudiants devront présenter leur thèse en troisième année de troisième cycle et ne pourront plus repousser cette échéance qui les éloigne d'autant d'une installation au cabinet mais cette année supplémentaire doit répondre à plusieurs conditions : la première, et qu'elle ne doit pas être un prétexte pour répondre de manière totalement imparfaite à la problématique des déserts médicaux, la seconde tient l'adhésion des étudiants du Collège national des généralistes enseignants afin de les emmener dans cette réforme et la troisième, et celle de l'encadrement, s'il est bien précisé que ces stages s'effectueront sous un régime d'autonomie supervisée, il devrait être obligatoirement encadré par un maître de stage.

la rémunération, la proposition de loi évoque une rémunération à l'acte, 7 autres sont me semble peu abouti ne risquerait-elle pas en fait de créer des conflits entre stagiaires et référent, ne faudrait-il pas un socle commun salariale avec pourquoi pas une incitation supplémentaire dans le cas de cabinet à forte activité ou dans le cas, par exemple, une pratique en zone sous-dense, de manière générale, n'oublions pas que ce sont les bonnes conditions de travail et ça a été dit par les orateurs précédents un environnement professionnel stimulant des territoires accueillants pour les familles qui sont, je le crois, les critères privilégiés du choix d'installation des jeunes professionnels plutôt que de dire, orienter les docteurs juniors en priorité vers les territoires sous dotés dont la définition reste imparfaite, ne pourrions-nous pas dire orientons les en priorité vers des lieux d'exercice où il existe des dynamiques de santé Des MSP des exercices professionnels coordonnées des équipes de soins primaires à même de leur donner envie de poursuivre l'aventure et faisons en sorte dès le début des études médicales de former des jeunes, des jeunes avec toutes ses réserves, le groupe RDSE n'est a priori pas défavorable à la proposition de loi mais vous l'aurez compris pas hein, n'importe quel prix notre groupe déterminera son vote en fonction de la discussion qui va suivre et du sort qui sera réservé aux amendements, notamment les plus coercitives. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à madame la présidente, Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que cette proposition de loi n'est pas sorti du chapeau le président Retailleau l'dit en effet, nous en parlons depuis plusieurs années avec avec et l'Ordre des médecins et des doyens et lors de l'audition que nous avions fait en début d'année, notre commission associant l'association des étudiants en santé de France et la conférence des doyens cette quatrième année avait été évoquée, recueillant un assentiment notamment de la conférence des doyens je voudrais tout d'abord rapport remercier le rapporteur de la commission des affaires sociales, pour son travail sur ce texte que j'avais bien évidemment co-signé, elle a en effet apporté de clarifications qui me semble indispensable sur l'entrée en vigueur, tout d'abord, il est parfaitement clair que l'allongement de la durée des études ne s'appliquera pas aux étudiants qui ont entamé leur 3ème cycle la réforme suppose d'une part, une révision de la maquette qui ne s'improvise pas et, d'autre part, il ne s'agit pas de prendre au dépourvu des internes déjà bien avancé dans leur cursus 2ème précision nécessaire, il ne s'agit pas de réformer les études de médecine générale pour répondre uniquement à l'accès aux soins dans des territoires sous-denses, il s'agit de réformer les études de médecine générale pour consolider la formation des futurs médecins en leur permettant de se confronter aux caractéristiques de l'exercice en médecine de ville sous un régime d'autonomie superficie la crainte des étudiants, nous l'avons entendu dès 2019 lorsque la Commission a proposé d'aménager à l'époque, la troisième année du cursus pour permettre un an devenu si mois en CMP, 6 mois de stage en autonomie supervisée, il ne se sentait pas prêt à un exercice Othonon craignaient pour la qualité de leur formation et redoutait une affectation forcée dans un lieu non choisi abandonnés à leur solitude dans des territoires dans le terme même de désert usité fait parfois, reconnaissons-le, une description peu engageante, rien de tel dans le texte que nous proposons le mode d'exercice, hé bien, celui de l'autonomie supervisée sur l'autorité de maître de stage universitaires formé avec une formation à l'exercice en ville et très certainement à l'exercice coordonné avec le collectif et la pluri-professionnalité auquel les jeunes médecins Aspire la formation 1er recours en médecine de ville à la gestion de l'entreprise médicale entre guillemets, qui fait actuellement défaut ou à la compréhension des mécanismes des projets territoriaux je pense particulièrement aux ces BTS ou à d'autres projets de ils viendront compléter le cursus, ce seront de vrais apports pédagogiques pour les futurs médecins nous à nous n'allons pas tenter de transformer de jeunes internes, un médecin de famille à ancienne n'mettre un médecin sous chaque clocher ça c'était avant, mais maintenant, il en est ainsi, ce n'est plus la société actuelle, mais en revanche il faut il faut définir pour les populations en difficulté d'accès aux soins, il faut réfléchir à des formes qui peuvent évoluer dans les territoires donnés réfléchir à des zones d'activités médicales permettant un équilibre permettant aux patients et aux médecins un équilibre dans les demandes de recours, la concurrence entre les territoires et délétère et il nous faut plus de coopération quant à l'affectation forcée, même si je conçois bien que c'est le souhaitent certains, elle ne me semble pas envisageable dans le contexte de la démographie médicale actuelle et du vieillissement de la population que nous connaissons, on ne gère pas la pénurie par la coercition et n'existe pas de zones sur-dotées en tout cas pas de zones sur-dotées en secteur 1 et nos collègues là 10 à la fois un phénomène urbain, périurbain ou rural, en revanche, je pense, et c'est ce sera un des rôles de la mission que vous allez mettre en place Monsieur le Ministre, je pense que la mission devra associer les ARS les du, à faire les représentants des internes, les ordres et les URPS et les élus et les élus pour définir les zones et les lieux de cette professionnalisation sur chaque territoire avec ces temps de formation nouveau ce dispositif crée du temps médical supplémentaire, ça c'est majeur en irriguant les territoires chaque année de nouveaux médecins la nouvelle maquette incitera les internes en médecine générale à passer leurs tests échéance qu'ils ont aujourd'hui trop tendance à repousser ce qui est rédhibitoire pour les installations et ce qu'il dément un peu l'idée de de retard à l'installation par cette 4ème année les territoires ont un rôle à jouer pour retourner le pour soutenir le développement des maîtres de stage universitaire, cela a été dit, faire valoir leur dynamique et mettre en place de bonnes conditions n'les collectivités sont déjà très impliqué certaines obtiennent d'excellents résultats, il existe déjà 12000 mètres maître de stage universitaire certes le nombre devra être renforcée pour être maître de stage universitaires pour un docteur junior mais je pense que c'est tout à fait possible bien sûr, cette proposition de loi ne saurait constituer une réponse unique au creux de la démographie médicale auxquels nous serons confrontés pendant encore au moins 10 ans à cette question éminemment complexe les réponses doivent être multiples elles vont de la télémédecine aux dégâts sont tâches en passant par l'organisation de transport d'accompagnement pour les patients, et cetera, la liste n'est pas exhaustif, donc je pense que ce texte propose en effet de préparer les étudiants en médecine générale à la médecine de ville afin qu'ils fassent leur choix de vie et d'exercice en confiance et en pleine connaissance des territoires où ils pourront faire le choix de s'installer ce pari, il faut le prendre sans tarder, dans un esprit gagnant-gagnant, c'est pourquoi, bien évidemment, je voterai ce texte. merci, madame la présidente et la parole est maintenant à Daniel Chassain pour le groupe, les indépendants. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission madame le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi du président, Bruno Retailleau, poursuit un objectif que nous souhaitons tous pour atteindre depuis maintenant une décennie, faire en sorte d'avoir des médecins dans nos villages dans nos bourgs bref lutter contres les zones sous-denses et je sais que la commission des affaires sociales et mobiliser sur le sujet, élu de la Corrèze médecins en milieu rural, je ne peux que constater les problèmes de manque dramatique de médecins généralistes qui suivent rural ou en périphérie des villes, les citoyens doivent pouvoir être soigné et suivi, nous souhaitons avoir un médecin dans nos maisons de santé, j'avais d'ailleurs déposé une PPL à ce sujet, la suppression du numerus clausus est une bonne chose, mais nous allons devoir patienter une dizaine d'années avant d'en ressortir les premiers effets sur nos territoires actuellement nous allons vers une catastrophe, notamment dans les territoires ruraux si nous ne prenons pas rapidement des décisions efficaces avec aussi des urgences encombrées car cela a été dit, beaucoup n'ont pas de médecin traitant la BPL que nous étudions, aujourd'propose une avancée nouvelle c'est aussi une des promesses de campagne du président Macron l'urgence est réelle et je me réjouis que nous ayons ce débat et je félicite Madame la rapporteure Colin Corinne Imbert, j'ai rencontré récemment des étudiants en médecine qui m'ont fait part de leur crainte, ce qui ressort, c'est le sentiment d'être exploitées avec une année supplémentaire en étant payé 2000 euros par mois après 10 ans d'études, ce que je conçois totalement totalement auparavant vous savez des remplacements effectués en 6ème ou 7ème année les étudiants tu dis en médecine, les études de médecine sont déjà très longue ne ne ans et Andres nombreux stages au programme, les étudiants s'inquiètent aussi de cette dernière année d'internat de ne pas être suffisamment seconder mais j'ai répondu qu'ils auront un médecin traitant, et je rappelle que, actuellement, après 3 ans

et qu'il n'aurait pas été adopté de proposer une réécriture de l'article unique et s'inscrivait dans la pensée qui a dominé nos échanges en 2000 19 au moment où la loi relative à l'organisation, la transformation du système de santé à l'époque, je rappelle que c'était un amendement consensuelle de la commission pour que les 6 derniers mois d'internat puisse se réaliser dans les territoires où il y a un manque de médecins, cela a été négocié par le président Alain Millon avec les étudiants, mais le décret n'est pas paru mon amendement proposé que le stage de ça se passe soit subit de notre stage de six mois faisant passer à un an sans une année supplémentaire complète à l'internat en médecine générale bien sûr à la priorité donnée aux zones sous-denses de plus, j'ai proposé une rémunération plus importante de cette année de ça se passe ce qui compléter mon amendement j'ai déposé un deuxième qui lui aussi a été déclarée recevable pour les mêmes raisons que le précédent pour lesquels je conserve un peu mon incompréhension, il portait sur la rémunération des médecins junior dans le cadre d'une 4ème année d'internat, je porte je proposais de placer cette rémunération mensuelle à hauteur de l'équivalent de 10 consultation à à l'acte par jour avec un logement, mais le médecin qui fera appel à un médecin junior mais aura une clientèle bien sûr très importante, je rappelle aussi que les étudiants de dernière année d'internat de professionnalisation ont déjà 9 ans d'études ils sont formés, ils peuvent consulter seul mais bien sûr, avec l'aide, les conseils de médecin référent médecin maître de stage, universitaire, bien sûr, c'est préférable, et c'est dans cette PPL mais Monsieur le Ministre, lorsqu'on a une clientèle débordante, les médecins n'ont pas le temps d'être hein messieurs, voilà la réalité du terrain et le médecin devra devenir M avec plus de proximité dans la formation, enfin mon 3ème amendement porte sur le lieu de la dernière année d'internat, prévu dans la PPL, je pense qu'il est important qu'elle soit faite dans le territoire de CHU où l'étudiant a fait ses études de même aussi que des étudiants en quatrième et cinquième année pourraient aller dans les hôpitaux périphériques, cela participe aussi à la répartition géographique des étudiants et des internes et à la découverte des territoires, ministre, non, mes chers collègues, nous avons l'impérieuse nécessité de proposer l'accès aux soins dans tout n'étaient nos territoires, c'est le rôle de l'État, nous devons, à mon sens davantage écoutez décide, étudiante en ce qui concerne leur rémunération chez Philippe, monsieur le président, le groupe les indépendants votera en faveur de cette PPL qui j'espère apportera en 1000 900 en 2026 des solutions pour les zones sous-denses merci. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Raymonde Poncet moche pour le groupe écologiste.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame la rapporteure, chers collègues, signe de l'impuissance des politiques publiques depuis longtemps les zones sous-denses s'étendent renforçant les inégalités d'accès aux soins selon l'adresse entre 2015 et 2018, la part de la population française vivant en zones sous-dotées en médecins généralistes a augmenté de 50 particulièrement impacté les zones rurales et les zones populaires Tom et des métropoles subissent à la fois les fermetures des hôpitaux de proximité des maternités, des services d'urgence et le non-remplacement des médecins, des infirmiers ou des sages-femmes au domaine de sang dans le domaine de la santé, toujours selon l'adresse 60 pour 100 des personnes en territoires ruraux connaissent des difficultés d'accès à un médecin généraliste, comme souvent, les mesures d'incitation financière ont été privilégiés, des dizaines de millions ont été dépensés avec des résultats plus que décevants, la Cour des comptes en 2014 puis en 2019 constate que ces mesures ont plutôt provoqué des effets d'aubaine pour les médecins, déjà en place cet échec doit nous conduire à reprendre l'analyse des causes pour de nouvelles solutions si certaines études scientifiques disponibles, conclut qu'un stage long en zone rurale, sous-dotées, surtout en fin de cursus peut encourager les nouveaux médecins à s'y installer, beaucoup estiment au contraire l'impact très faible, mais d'autres études pointent des pistes intéressantes structurels qui ont donné d'excellents résultats, notamment à l'étranger et de plus des résultats durables à ce sujet la méta-analyse de l'adresse en 2021 est formel : ils ressortent de toute la littérature scientifique, que le choix de s'installer dans une zone mal desservie est en 1er lieu liée à un ensemble de facteurs personnels, et ce sans méconnaître d'autres conditions, les conditions d'environnement plus intensité des services publics, proximité des centres hospitaliers autres professionnels de de santé installé sur ce même territoire dynamisme des activités économiques ne toutes ces raisons, nous les connaissons mais de façon constante, les travaux de recherches concluent que l'origine rurale du médecin est un facteur essentiel et le meilleur prédicateurs de l'installation en zone rurale, être né en milieu rural, y avoir grandi y avoir fait sa scolarité ressortent dans tous les pays, comme des déterminants majeurs du choix d'exercer dans cet environnement rural aussi, or les territoires ruraux étant majoritairement populaire, les élèves issus de ces territoires se heurte à la sélection du à l'université amplifiée depuis quelques années par Parcoursup véritables machines de reproduction sociale, les études de santé compte parmi les plus clivée socialement si déjà se représenter en en études de médecine, les chances de réussite d'un enfant de cadre métropolitain est 2 fois 5 2 Emmy fois supérieure à celle d'un enfant d'ouvrier, cette absence de diversité sociale a été amplifié par les politiques de déstructuration de l'enseignement supérieur et la concentration des lieux de formation, les fusions des universités vont vont à l'encontre frontale des recommandations de l'OMS préconisant justement la décentralisation des centres de formation dans les tréfonds territoires ruraux et sous-denses de nombreux pays ont entamé une démarche de décentralisation des ressources à des centres satellites ruraux voire ont ouvert de nouvelles écoles de médecine la Norvège, l'Australie, le Canada et, suivant ainsi les recommandations de l'OMS, de la critique des critères de sélection à l'université pour ouvrir la diversification sociale à la décentralisation, autant que possible des lieux de formation certaines solutions durables contre les déserts médicaux réclament des mesures structurelles qui questionnent les politiques tant en matière d'enseignement supérieur que d'aménagement du territoire, aménagement du territoire qui accentue aujourd'hui un phénomène de répartition sociale du territoire entre concentration des cadres, ce que le chercheur Guillaume Faburel appellent les classes créative des cadres au sein des grandes métropoles, d'un côté et les territoires ruraux majoritairement ouvrier de l'autre, qui subissent la dévitalisation économique la fermeture des services publics et des déserts médicaux, il n'est pas étonnant, dans ce cas que le démographe Hervé Lebras et pu dire hier que la France des déserts médicaux étaient celle des gilets jaunes or pour lutter contre ce phénomène, l'OMS recommande des politiques ciblées pour les étudiants d'origine rurale et recommande de décentraliser une partie des campus et des programmes d'internat, cette proposition de loi propose, selon nous, une solution de régulation très partiel et contesté en faisant l'économie d'autres types de régulation de de, du moins de son débat, notamment par l'installation comme des causes que je viens d'évoquer, c'est pourquoi le groupe écologiste votera contre, je vous remercie.

pour président et c'est le ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est l'un des chemins de recherche pour préserver et améliorer notre système de soins sur tous nos territoires, la médecine générale est la seule spécialité à n'avoir que 3 années de formation, un 3ème cycle sans phase de consolidation ni d'accès au statut de Docteur junior. Le dispositif proposé vise à mettre en place une craqueler moi né véritable année de professionnalisation, les internes réaliseront plusieurs stages un autonomie superviser et un ambulatoire, tout en préparant mieux leur installation longtemps mentionné comme une piste de réflexion pertinente cette 4ème année permettrait l'arrivée chaque année de plusieurs milliers de médecins junior. En priorité, dans des zones où l'offre des soins est faible. Ce serait aussi l'opportunité pour ces jeunes professionnels de découvrir et apprécier d'autres lieux d'autres modes de vie. Plusieurs véhicules législatifs nous permettront de débattre davantage de cette mesure, le gouvernement les a inscrit dans le projet de de loi de financement de la Sécurité sociale et je m'en félicite, nous sommes tous à la recherche de solutions pour consolider la formation de nos médecins faciliter leur l'installation est également permettre à chaque citoyen d'obtenir les soins qu'nécessite sans inégalités, la mesure s'inscrit ainsi dans une logique plus globale et effective d'amélioration de la santé pour tous, en complément d'autres dispositifs déjà mis en oeuvre par l'État et nos collectivités, elle nécessitera d'assurer nombre suffisant de maître de stage, grâce à l'effort engagé le nombre des praticiens habilité à était en hausse de 9 6 % entre 2000 19 et 2021 il faut inciter davantage les médecins à candidater faciliter les procédures ainsi ciblant les territoires où l'offre des soins est très insuffisante,

Qu'il faut prendre en compte, si l'on souhaite assurer le revenu sur le territoire et leur installation dans la durée, profession du conjoint, éducation des enfants, service public, sécurité, mais aussi l'organisation du travail en lui-même existence d'un réseau de paramédicaux et des spécialistes, c'est là suppose d'ailleurs. Augmenter aussi le nombres de maître de stage universitaires dans les autres spécialités tout et n'a, semble, en fait, j'en suis d'autant plus persuadé que je viens d'un territoire non pas non sous-dotées mais. Sous sous. Doté, je dis bien sous sous-et j'aimerais d'ailleurs souligné le travail réalisé par mes collègues de la commission des affaires sociales sur les systèmes de Saint-à Mayotte l'offrent des soeurs en médecine de ville en particulier et balbutiante 27 médecins généralistes libéraux dans cette maître de stage, quasiment aucun spécialiste pour 300000 habitants à la Réunion. Le département voisin, je viens collègue de la réunion qui était là. Où la population est presque 3 fois supérieure, il y a 1200 médecins généraux et plus de 160 mettre 160 maître de stage Mayotte n'a pas de CHU. Son centre hospitalier doit pallier les lacunes d'accès aux soins primaires. Il est constamment sous tension et multiplie les évacuations sanitaires vers la Réunion, les Mahorais qui en ont les moyens vont se soigner hors du département, soit la Réunion ou ici en métropole. Les autres renoncent souvent aux soins même essentiel, l'état de santé de la population est très en-deçà de la moyenne nationale, la sécurité sociale est toujours régi par des dispositions spécifiques mais je suis heureux de constater que la convergence progresse avec notamment la le projet de loi de finances. Pour la sécurité sociale. l'année prochaine l'extension à Mayotte de la complémentaire santé solidaire c'est oh, vous savez que les médecins libéraux, souvent, n'ont pas signé de convention avec la sécurité sociale, beaucoup de problèmes pour certains malades parce qu'ils ne sont pas remboursés, donc il reste à la maison, comme je l'ai dit un peu plus haut cette 4ème One aide hein Thomas apprendrez beaucoup aux internes qui l'affaire est chez nous et serait une opportunité pour Lille je vais souligner ici la création à l'initiative du hospitalier de Mayotte, d'une agence TT territoriale de recrutement qui a reçu cette année un Grand Prix de l'innovation et elle vise l'ensemble des des acteurs de santé du territoire centralisé le recrutement accompagner les candidats renforcer la l'attractivité fidéliser, là, je fais la campagne de l'hôpital, je ne les obstacles sont nombreux dans nos territoires et ils le sont de façon d'autant plus intense et urgente à Mayotte, cette proposition de loi contribue en partie à le lever, le groupe des pays votera positivement cette mesure merci. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant à Bernard Jomier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues. Notre monde vit assez de malheurs actuellement pour qu'on essaye au moins Lyon en épargnés, hein, c'est de mal nommer les choses. Or, cette proposition de loi et je l'entends depuis la présentation par son auteur, je crois qu'il n'est plus là. Installe cette confusion. Elle a été déposée au mois de janvier dernier avec un titre qui porte sur la formation des internes en médecine générale et la lutte contre les déserts médicaux. 8 mois après, alors qu'elle a inscrite en séance publique la partie lutte contre les déserts médicaux a été effacée du titre mais omniprésente dans les propos de l'initiateur de la proposition de loi lui-même et des collègues qui, à tour de rôle, se sont exprimés sur cette PPL alors si ça n'est pas de la confusion dans le débat, il faut m'expliquer ce que ça signifie. Et ça n'est pas parce que le titre a été expurgée que cette proposition porte bien sur la formation des internes de médecine générale et je je voudrais vraiment insister sur ce point parce que je pense que c'était un des problèmes actuels du débat public dans notre pays, c'est de masquer les objectifs et de ne pas le dire clairement à ceux qui sont les premiers concernés, en l'occurrence les jeunes médecins qui sont visés par ce dispositif. Nous, nous préférons le langage des intentions qui sont clairement affirmé et à cette aune, c'est un texte qui est maladroit, notre vie publique et beaucoup trop encombré de propos qui sont euphémisé nous le voyons tous les jours maintenant dans notre pays quand on parle de concertation, ça veut dire en gros : cause toujours et quand on parle de co-construction, ça veut dire on fait comme j'ai prévu. Et c'est ce qui est en train de se passer sur ce dossier là, le président, Bruno Retailleau, nous connaissons ses capacités d'analyse, de clarté et de synthèse, je ne veux pas croire une minute qu'il les a perdu tout récemment Et donc il faut clarifier, il faut clarifier la véritable question qui se pose à nous, c'est est-ce que l'on peut conjuguer dans un dispositif unique l'objectif d'une meilleure professionnalisation des études de médecine générale avec l'apport de temps médical supplémentaires au bénéfice d'une population qui en a besoin, donc en clair : doit-on proposer demander aux jeunes médecins de pas ici IP à une meilleure offre de soins dans les 85 90 % de notre territoire qui en a bien besoin. Et de 2 choses l'une, si ce n'est qu'une question de formation comme le dix-sept, intitulé encore une fois, alors la quatrième année n'a rien à faire ici. Car ce n'est pas le Parlement qui jamais, ce n'est pas la loi qui décide de la longueur des cycles des études de médecine. Mais ce n'est pas le Parlement qui décide des lieux dans lesquels les étudiants doivent effectuer leur stage. Hé oui, alors on peut dire que le gouvernement en inscrivant le dispositif dans le PLFSS prend un risque d'inconstitutionnalité, mais moi je dis qu'en en faisant une proposition de loi on abaisse le niveau de la loi dans un débat d'ordre réglementaire. mais si, comme nous le pensons, on peut proposer ce dispositif, qui porte ces 2 objectifs, alors il faut commencer par tenir un langage de vérité aux premiers concernés, ceux qui sont l'objet les jeunes médecins et d'abord leur dire fortement que nous savons qu'ils ne sont pas responsable de la grave pénurie de médecins que connaît notre pays, nous sommes un pays qui, au mitan des années 70, former 10000 médecins par an nous avons abaissé à 3250 par an, ce nombre est actuellement nous en sortons 8500 par an, comment il y aurait-il pas une pénurie profonde alors que notre pays dans le même temps est passé de 50 millions d'habitants, à plus de soixante-cinq un vieillissement de la population des problématiques d'autonomie et de dépendance et les jeunes ne sont en rien responsables de cet état de fait, ce sont les gouvernements successifs, obsédé par une politique de l'offre, il s'agissait de réduire les dépenses de santé, en réduisant le nombre de médecins formés et à cette décision des gouvernants ont participé activement des syndicats professionnels médicaux. Et l'Ordre des médecins qui, ensemble, hé oui, disait : ah bon, on manque de patients, alors on va réduire le nombre de médecins, c'est ça la vérité et les seuls qui à l'époque et je m'en souviens bien au mitan des années 90 ont pris position pour dire que c'était une erreur funeste c'était les organisations de jeunes, celle que vous n'associez pas la négociation en en en proposant un parlement un dispositif précipité, ils refusent et ils ont raison, une 4ème d'année d'internat, car c'est un dispositif qui ne le reconnaît pas pleinement, c'est un statut sous-rémunérés 5, statut qui fait croire qu'il ne s'agit que de formation et qu'il en est qui, qui cite même pas les objectifs, c'est une décision qui est prise sans eux, vous mettez la charrue avant les boeufs, il faut d'abord négocier, il faut négocier car oui, les étudiants peuvent être mieux préparés à des formes d'exercice qui nécessite des approches qui se sont complexifiées avec la rareté de l'offre, mais aussi avec de nouveaux parcours de soins avec de nouvelles organisations territoriales avec des nouveaux enjeux sociaux qui parfois sont plus prévenant et qui rendent inopérants, une approche qui est purement sanitaire et donc conjugué à une meilleure professionnalisation avec l'apport de temps médical dans nos territoires sous-dotés, mais donc il s'agit bien de reconnaître le quatre pédagogique et l'apport de santé publique. La bonne réponse, ne se situe pas dans la 4ème année d'internat de médecine générale, mais dans une année de professionnalisation et les mots ont un sens qui doit respecter ses jeunes qui doit reconnaître est rémunéré à sa juste valeur la contribution demandée qui doit prendre en compte leurs problématiques de vie qui doit associer aux universités, les collectivités territoriales qui sont mieux à même d'assurer des conditions matérielles de logement, de transport, de vie quotidienne, qui soit adapté, ce texte est précipité et nous avons bien noté d'ailleurs la course qui s'est engagé entre votre proposition de loi et le gouvernement pour le PLFSS oui on a, on a bien noté le calendrier qui a été rapport rapport rappelé par la rapporteure voilà pour porter à toute vitesse, ce dispositif et je ne doute pas, nous avons compris que, au moment du PLFSS se renouera une alliance qu'on a vu lors des textes au mois de juillet, hé oui, on en prend le pari, si vous voulez, chers collègues, c'est ce qui est en train de se préparer, mais là c'est précipité s'est précipité, car il ne doit pas être inscrit aujourd'hui dans la loi la 4ème année de médecine du 3ème cycle de médecine générale, il doit être négocié avec les jeunes médecins avec leurs organisations syndicales, en quoi ils peuvent apporter du temps médical supplémentaires au bénéfice de notre population et de la santé publique, ils y sont prêts, mais pas alors que le Parlement aura délibéré, on négocie d'abord on vote la loi ensuite cette proposition de loi et donc à bien des égards contreproductive, elle ne pose pas un cadre qui soit adapté et le législateur commettrait une erreur s'il venait à prendre la décision de changer ex abrupto la durée du 3ème cycle de médecine générale nous nous appelons volontarisme de la négociation de la responsabilité partagée, oui, d'une meilleure formation et d'un temps médical augmenter oui et sans ces conditions, nous voterons contre cette proposition, je vous remercie. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant à Alain Milon pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission affaires sociales madame la rapporteure chers Corinne en 1947 Jean-François Gravier publié Paris et le désert français, ouvrage qui fit longtemps référence et dans lequel l'auteur démontrer le fort déséquilibre entre Paris et la province et les conséquences qui en résultent 75 ans plus tard, la rhétorique du désert retrouvent une acuité et une actualité particulièrement sensible, notamment en matière médicale depuis quelques dizaines d'années, Bernard depuis quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, peut-être même une quarantaine, une au moins 40 ans les déserts médicaux se répondent, sur l'ensemble du territoire et ne sont plus un phénomène uniquement rurales, les villes et notamment les quartiers périphériques sont concernés, la question est de savoir si ces déserts médicaux sont des phénomènes spécifique ou s'ils ne sont pas davantage la conséquence d'un phénomène global lié à la disparition des services publics dans les territoires ruraux et certains quartiers suburbains peut-on raisonnablement dans ces conditions, espérer l'installation de médecins et de leurs familles dans des lieux sous-équipée en service de qualité, notamment scolaires et culturels stricto sensu, peut-on raisonnablement envisager que la vie et le rythme de travail d'un médecin de campagne des années 1970 1980 correspondent aux attentes des nouvelles générations,

face à cette situation complexe cette situation multi-causal, il est impératif de proposer des solutions permettant de concilier les attentes des jeunes médecins avec celle d'une patiente, elle inquiète de voir son accès aux soins limités la PPL donc déposé par le président bien de Bruno Retailleau, s'inscrit dans cette volonté d'apporter, d'une part des réponses précises à nos concitoyens et aux élus locaux, qui sont souvent en première ligne face aux doléances de leurs administrés et d'améliorer, d'autre part le cursus de formation des étudiants en médecine générale, cette préoccupation n'est pas nouvelle pour le Sénat, car dès 1919 des 2019 nous avions adopté, Monsieur le Ministre, un dispositif presque similaire mais resté lettre morte en l'absence de décrets d'application qui relevait du gouvernement aujourd'hui, le gouvernement a ajouté à la hâte un article dans le PLFSS reprenant quasiment les termes de cette PPL sans y apporter la moindre plus-Value, la méthode est pour le moins discutable car elle traduit une forme de mépris à l'égard du travail parlementaire en se l'appropriant en catimini, au lieu de le valoriser, mais laissons de côté ce problème méthodologique et concentrons-nous sur les dispositions de ce texte, qui ont fait l'objet de débat fort intéressant en commission des affaires sociales, la reporter, tant le sujet rêvé différente dimension sociétale d'aménagement du territoire, et bien il va vaguement de formation de nos étudiants, je sais que les internes aujourd'hui contestent le bien- fondé de cette réforme, en raison de la logement d'un an de la durée du 3ème cycle des études de médecine générale l'obligation de réaliser cette 4ème année en stage ambulatoire en autonomie supervisée et prioritairement dans les zones sous-denses identifiés par les ARS les inquiète parfois aussi, il convient de souligner les apports de ce texte pour la professionnalisation des internes en médecine générale grâce à cette année supplémentaire ils acquerront le statut de Docteur junior dont ils ne bénéficient pas aujourd'hui et seront mieux préparés à l'exercice de la médecine en ville grâce à l'accompagnement d'un médecin superviseur ce texte constitue donc une réelle avancée, même si certains points restent en suspens, c'est le cas notamment des conditions de rémunération de ses étudiants, mais également de leurs conditions d'accueil dans les communes en matière d'hébergement en matière de transport, ça a déjà été dit ces frais seront-ils à la seule charge des collectivités, comment les inciter à aller dans ces zones sous-denses, de même la question de l'encadrement demeure essentielle, le nombre de maître de stage formé sera-t-il suffisant et répartis équitablement sur l'ensemble du territoire, pédagogique des maîtres de stage devront être réglés dans des délais raisonnables et non plusieurs mois après la fin des stages, des internes, contrairement à ce qui se passe actuellement ces retards de paiement pénalisent et démotive ces maîtres des stages qui se sont engagés dans ce processus d'accompagnement et de formation des internes, enfin, il convient de mener une réflexion sur le lien entre la création de postes d'internes et le bassin de vie, des lieux d'implantation des universités en terme de démographie de territoire de situation sanitaire de la sociologie, ceci afin d'éviter des distorsions entre la réalité de terrain et le nombre d'internes formés dans les centres hospitaliers universitaires, un exemple simple, dans les Alpes Maritimes et conclu un 1000000 100 1000 habitants 20 postes d'internes en médecine générale, c'est largement insuffisant, je conclus, monsieur le président, Mesdames et messieurs, mes chers collègues, cette PPL pose les jalons d'une répartition géographique plus équilibrée tout en respectant le libre choix d'installation des futurs médecins principe cardinal de notre médecine. Merci, cher collègue. Et la parole est maintenant à Anne vont allons groupe les républicains pour 4 minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comment la France nation à la médecine réputé et au système de soins généreux et ont envié en était à l'arrivée à cette situation de pénurie aujourd'hui 11 % de la population française serait dépourvu de médecin traitant, cette proportion atteignant parfois le double comme dans mon département de l'Ardèche, sans doute, notre pays a-t-il refusé de considérer la question du nombre de médecins sur le long terme, c'est là une responsabilité partagée, il n'est que de lire les échanges entre le gouvernement et les parlementaires du début des années 90 aux élus qui s'inquiétaient des conséquences des baisses successives du numerus clausus en deuxième année de médecine sur la démographie médicale à venir les gouvernants répondez par des courbes statistiques et des projections lénifiante, il faut donc appréhender le sujet en sachant que, de notre inertie ou de nos actions dépendra l'accès aux soins des temps à venir ces décennies qui seront marqués par le vieillissement et la perte d'autonomie de la génération du baby-boom, nous, de nous savons que nous devons considérer le problème sans tabou, mais que le salut ne viendra ni des slogans ni des Mireille des miracles, mais d'une conjugaison de solutions complémentaires et d'effort collectif étant les représentants au Parlement des collectivités locales, il est de notre devoir de nous emparer du sujet en proposant des solutions concrètes et viable et je salue en cela l'initiative de Bruno Retailleau, car à présent ce sont essentiellement les élus des territoires qui investissent dans des solutions pragmatiques, elles le font, notamment avec la création de maisons de santé pluridisciplinaires le salariat des médecins, le recrutement des personnels les déchargeant des tâches administratives chronophages ou même, comme le fait le département de l'Ardèche en répondant concrètement à la question du logement des internes, la mesure proposée par le groupe Les Républicains, n'a pas la prétention de régler à elle seule la pénurie des médecins généralistes, mais d'en saisir un volet important, celui de la présence médicale, les internes qui en constitue l'un des rouages important ne doivent nullement se sentir montré du doigt et tenu pour futur responsable de la situation, au contraire, nous considérons qu'il constitue une partie de la solution cette année supplémentaire de formation, de consolidation ne résoudra pas à elle seule le problème de la désertification médicale mais elle constitue l'un des leviers à actionner aux côtés d'autres tels que meilleur recours aux infirmiers en pratique avancée aux assistants médicaux à la restructuration de l'offre de soins qui conjointement permettront de restaurer le droit à la santé pour chacun cette 4ème année d'internat et Madame la rapporteure la rappeler permettra d'aligner la formation des futurs généralistes avec le cursus des autres spécialisations en réalisant des stages en en autonomie progressive la superficie de la supervision pardon de médecins expérimentés, ils bénéficieront également d'une rémunération supérieure à celle reçue pendant leurs années d'internat de plus au cours de cette année passée dans les localités sous-dotées ses futurs médecins prendront toute la mesure du délaissement pour ne pas dire de la détresse médicale de certains territoires, notamment ruraux, ce qui, à l'aube de leur carrière, sensibilisera autant ces praticiens qui ont fait de la santé, une vocation qu'elle mobilisera la conscience civique de ces jeunes citoyens je vous remercie. remercie. Merci, chers collègues, la discussion générale est donc Close et nous allons passer à la discussion du texte de la commission et de son article unique, alors j'ai plusieurs demandes de prise de parole sur l'article unique on va commencer avec notre collègue Fabien Genêt. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, je voudrais saluer cette initiative de consolidation et de professionnalisation de la formation des internes en médecine générale contenues dans cet article, Car si cette initiative n'affiche plus pour objectif la lutte contre les déserts médicaux, elle représente tout de même un espoir pour nombre de territoires qui en sont privés, j'ai entendu que certains s'interrogerait sur un dispositif trop précipité qu'on accusera de mettre la charrue avant les boeufs, alors vous permettrez à l'élu charolais que je suis, de vous dire qu'on a plutôt le sentiment, dans nos campagnes qu'on a beaucoup trop tardé, en 2014 comme maire de Digoin, j'ai été confronté au départ de la moitié des médecins généralistes en quelques mois, et à l'angoisse de la population privée de soignants confrontés à l'irresponsabilité totale de notre système de santé, aucune institution ne faisant quoi que ce soit et l'Agence Régionale de Santé finissant par renvoyer les patients vers le maire que j'étais depuis, heureusement, la situation s'est localement améliorer avec la création par exemple d'un centre départemental de santé par le président qui salarie des médecins mais aussi avec la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire, soutenu par l'intercommunalité, porté par une équipe de médecins extrêmement dévoués, dont d'ailleurs une majorité de jeunes médecins, je pourrais bien sûr, vous parlez comme ma collègue Marie Mercier d'autres communes comme Cuisery genou il qui cherchent encore leur médecin, tout cela pour dire, Monsieur le Ministre, que votre tâche n'est pas facile mais elle est vitale, nos concitoyens des territoires ruraux s'adapte de gré ou de force aux délégations de tâches au cabine de télémédecine et demain au médecin stagiaire qui a, ils n'ont pas d'autre choix, mais il ne saurait accepter qu'on finisse par entériner le principe d'une d'une médecine à 2 vitesses, monsieur le Ministre, l'urgence de la situation commande donc des mesures complémentaires et structurelles à cette initiative d'aujourd'hui une vraie mobilisation générale pour ne pas oublier le grand sacrifié de cette situation, le patient. Merci. Merci, cher collègue, donc toujours des interventions de deux minutes maintenant notre collègue Katia pour. Merci monsieur le président, après l'intervention de ma collègue Laurence Cohen, je souhaitais intervenir à mon tour sur cet article unique et ses limites. Il y a quelques années, les études de médecine duré 7 ans. Pensez-vous que les médecins été moins. Pour ma part, je ne le pense pas, je m'en sors pas trop mal, j'avais un médecin qui avait fait 7 ans d'études et donc apparemment ça va. Finalement, je m'en sors mal. Que maintenant au coeur du bassin minier, on a plus de médecin, donc on s'en sort bien plus mal, elles sont aujourd'hui ses études de médecine de 9 ans et avec cette proposition de loi, elle serait 10 ans pensez-vous vraiment que faire une année de plus ça va régler la question des déserts médicaux, en plus, il faudra des médecins seniors pour encadrer ces interne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il en manque partout en urbain : comment ruralité qui donc encadrera ces jeunes internes volontaire car on parle bien sûr de volontariat évidemment à moindres coûts je rappelle quand même qu'on va les payer 2000 à 2500 euros par mois pour 10 ans d'études plus que jamais, je pense qu'il nous faut réfléchir à l'installation, nous ne pouvons pas continuer à laisser s'installer dans les zones de soins à fort excédent des médecins, autrement nous ne régleront pas le problème, bien au contraire, il va s'aggraver, nous sommes favorables plus qu'à une dixième année à la réduction du 1er cycle et du second cycle après discussion et concertation, il nous faut une véritable loi pour rediscuter de la refonte des études de médecine dans son ensemble, avec l'ensemble des partenaires concernés car il n'y a plus de numerus clausus, vous l'avez dit, monsieur le ministre, j'ai bien entendu, vous disiez que les effets ne se verrait que dans 10 ans, malheureusement, les effets ne seront là que dans 10 ans si on desserre l'étau pour former plus de médecins, et si on donne des moyens immédiats en nombre de places dans les facultés, je vous remercie. Cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Pierre Ouzoulias. Merci monsieur le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, on l'a dit, l'hôpital public, il peut pas fonctionner aujourd'hui sans les internes, une une réalité j'aimerais rappeler 2 chiffres : la formation d'un d'un médecin généraliste coûte à l'université, environ 104000 euros par par personne n'est pas et par an et le travail qu'ils fournissent, lui il est estimé à 121000 euros, je rappelle que les internes de médecine Gannon moyenne six euros de l'heure et que 70 % des internes, des le dépasse, pardon le plafond hebdomadaire légal de 48 heures, en travaillant, environ 58 heures par semaine, coût de la formation 104000 euros. Chiffrage du travail qu'ils apportent 121000 euros, les étudiants en médecine sont les seuls étudiants en France qui rapporte de l'argent à l'État, les étudiants. Il faut le répéter, parce qu'ils le vivent comme une profonde injustice, ils ne comprennent pas qu'on reconnaisse ce qu'ils apportent aujourd'hui à la médecine et ce qu'ils ont fait pendant la période du Covid souvenez-vous, vous les avez appuyé applaudi pour six euros de l'heure, c'est ça la réalité aujourd'hui du travail lors de son audition par la commission de la culture du Sénat, le président de France universités Monsieur Manuel Tunon de Lara, ancien président de l'université de Bordeaux et praticien hospitalier déclaré, je le cite les CHU vont dans le mur les hospitalo-universitaires sont noyés sous des tâches cliniques entre 50 et 60, professeur de médecine ont de missionner depuis 2018 est-ce que c'est vraiment la réforme qu'ont besoin aujourd'hui, les études de santé merci monsieur le président. Merci, cher collègue, la parole est maintenant notre collègue Bruno rejouant. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission madame le rapporteur en commission aménagement du territoire et développement durable : nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet de l'accès aux soins dans les territoires qui malheureusement sont très nombreux en France maintenant, je dois dire qu'il est intéressant que la commission aménagement du territoire se soit aussi emparés de ce sujet-là, parce que c'est une manière c'est une vision peut être un peu différente de la commission des affaires sociales, au moins, au moins dans le dans le fait d'aborder ce ce sujet, alors moi je suis très heureux, je me dis enfin une PPL, celle du président Retailleau aujourd'hui qui envoie un message fort vers ces populations délaissées dans les territoires et surtout vers les élus locaux, les élus locaux, chaque fois que nous le déplaçons dans une réunion, irrémédiablement, nous on les maires nous parle de la du problématique de la présence médicale dans leur commune dans leur communauté de communes, donc c'est un message, c'est le 1er message fort envoyé par notre assemblée en direction de ses élus locaux que nous, qui sont nos partenaires numéro un, mais vu la situation désastreuse dans laquelle effectivement et la santé en France, il ne faudra pas s'en arrêter là le Sénat, la représentation des territoires et le lieu même où finalement on doit discuter et je propose bien que finalement cette ce vote qui va avoir lieu tout à l'heure, soit l'étape hein de quelque chose, car il faudra revenir et tous presque vous l'avez dit d'une manière différente, mais il faudra revenir avec ce sujet là, car on ne va pas le régler par cette seule disposition. un ensemble de mesures que suite au travail fait dans la commission, j'ai rédigé au sein d'une PPL et déposé seul cet ensemble de mesures prix à peu près simultanément ou, du moins dans des temps assez raccourci va pouvoir permettre que les Français, les 6 millions de Français, et les autres. Vont pouvoir voir leur situation s'améliorer ainsi, donc je pense que, aujourd'hui, exposé le long point de départ d'une discussion beaucoup plus longue sur l'accès aux soins des Français dans leur territoire, merci. Oui, merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'aimerais tellement que ça marche. Parce que ce n'est pas nouveau, ça fait 10 ans qu'on débat de cette question dans cet hémicycle, et ça fait 10 ans qu'on liste un certain nombre de dispositions pour essayer de répondre à la question des déserts médicaux avec mon collègue Hervé Maurey, en 2011, 2012 on a produit déjà un 1er rapport qui identifie le problème et qui fait des propositions qui sont sans doute des propositions qui, pour la période et sont un peu coercitive un peu dur, mais en tous les cas, elles existaient, et elles n'ont pas réellement changé en termes de nécessité alors qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle proposition, alors moi je ne vais pas évoquer la quatrième année, parce que je pense effectivement que ce n'est pas notre sujet, mais on utilise la quatrième année, sujet de formation pour essayer quand même de manière masquée de répondre à la question des déserts médicaux et qu'est ce qu'on dit on dit voilà. Si vous avez un maître de stage. Si le maire veut bien mettre un logement à votre disposition si il veut bien vous mettre une voiture à disposition et, pourquoi pas, si il veut bien créer un cabinet médical si toutes ces conditions là sont réunis. Vous stagiaire de quatrième année vous pouvez prioritairement faire votre stage dans des lieux Soudan où il n'y a pas de médecin, ça veut dire qu'ils ont dit : il y a un potentiel de 3500 médecins, moi je ne crois pas à ça, je n'y crois pas du tout, parce qu'effectivement on l'a assez bien expliqué ici, les internes ont une autre approche, une autre vision, moi je suis d'accord avec mon collègue Pierre Ouzoulias sur le fait que il faut reconsidérer la manière dont on voit les internes à l'hôpital parce que c'est à la limite de la maltraitance, c'est autre chose que d'autres questions des déserts médicaux, la question des déserts médicaux, c'est comment aujourd'hui l'État réparti l'ensemble des médecins de matières il tape sur le territoire et comment chaque administré un médecin à porter de 30 30 minutes à peu près et je crois que c'est cette question là qu'il faut résoudre mais et la proposition de cet après-midi ne va absolument pas dans ce sens-là, je vous remercie. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant à Stéphane Sautarel. Merci monsieur le président je voulais à mon tour me joindre à la voix d'un certain nombre de collègues pour bien évidemment remettre ce texte et cette proposition dans son dans son contexte, donc d'abord pour dire merci à notre groupe à Bruno Retailleau j'ai moi-même cosigné cette cette PPL parce qu'elle me semble indispensable et et et comme chacun l'a dit non suffisante, bien évidemment, ce n'est qu'une partie de la réponse, mais je dis aussi, enfin parce qu'il y a un signe, il y a une exaspération dans nos territoires qui est telle que si on n'est pas capable de répondre à l'offre de soins, de plus de 6 millions de Français et en particulier dans nos territoires ruraux d'autres questions vont se poser en termes d'accès au service public d'accès aux services les 3 services prioritaire, c'est la sécurité, la santé et l'éducation, si notre pays ici dans cette assemblée, nous ne sommes pas en capacité de répondre et désormais dans l'urgence parce que l'heure est grave leur le temps presse à ce besoin, là, nous ne sommes pas à la hauteur de la confiance que nos administrés que nos concitoyens que nos électeurs que les contribuables plaçant nous bien évidemment qu'il y a des sujets plus globaux, au niveau de la santé, au niveau de la situation des internes et que que c'est pas par les internes que l'on peut résoudre l'ensemble de la question et qu'il convient d'examiner la place des internes et la situation des internes dans dans ce système de santé, c'est bien évident, mais je pense que ce 1er signe qui est envoyé aujourd'hui à des territoires qui sont en désespérance, il faut entendre ça sur l'offre de santé que nous offrons à à à nos concitoyens, comme plusieurs collègues l'ont rappelé, me semble être une une absolue priorité et donc, je veux juste insister sur sur cette nécessité là qui bien sûr n'a pas été anticipé, mais aujourd'hui on peut débattre, on peut continuer à réfléchir, mais il faut qu'on compte, il faut qu'on avance, il faut qu'on agisse et donc merci pour ce débat qui est ouvert aujourd'hui et qui j'espère sera un 1er pas dans cette direction. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Jean-Pierre Sueur. Sur le le président monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre collègue Patrice Joly a présenté 2 amendements dont vient de parler Jean Luc Fichet ces deux amendements portent sur les effets et les conséquences, le rapport entre la formation et la présence médicale et notamment la désertification médicale ces deux amendements ont été retirés de l'ordre du jour, ils ne seront pas présentées en vertu d'une interprétation : Monsieur le Président, par rapport à laquelle je tiens à dire mon profond désaccord de l'article 45 de la Constitution, je vous rappelle que cet article dit que tout amendement en première lecture est recevable dès lors qu'ils pressentent un rapport, même indirect avec le texte, si quelqu'un ici peut m'expliquer que ces deux amendements n'ont aucun rapport indirect avec le texte, je les remercie de le faire, faute de quoi nous sommes dans l'arbitraire, donc je proteste aurait une nouvelle fois, et chaque fois que ça se présentera sur cette interprétation qui est faite ici de l'article 45 de la Constitution. Merci monsieur le questeur et. Maintenant le la parole est à notre collègue Élisabeth Doineau de l'Union centriste. monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues, il faut toujours salué les initiatives qui font parler de sujets qui sont très importants pour notre société et je veux remercier le président Retailleau d'avoir, en tout cas eu cette initiative, je remercie aussi Monsieur le Ministre d'avoir finalement corroborer à travers un article de dans le PLFSS à cette proposition, même si le titre a changé, en réalité, nous avons plus parler aujourd'hui des problèmes de démographie médicale que de la professionnalisation des professionnels de santé et je le regrette, tout simplement, je voudrais dire pourquoi moi j'ai des doutes parce que il y a des écailles, en fait, dans cette proposition de loi et là le 1er recueil, c'est en qu'il y a une non-adhésion des jeunes étudiants en médecine et pour moi il est important que l'on décide d'ici 2 lois qui sont en parfaites accord au moins avec la majorité de ceux qui seront concernés, c'est très important, dans les rues de France la semaine dernière et je tiens compte de leur avis parce qu'ils ne veulent pas être la variable d'ajustement d'un problème qui a été effectivement créés par toutes les précédentes majorité il faut le il faut le dire, nous n'avions pas anticiper le vieillissement de la la population, la population, les polypathologies n'avons pas non plus anticiper les besoins de cette société d'aujourd'hui qui souhaite aussi être soignée et qui consomment en fait de de la santé, il ne faut pas l'oublier non plus, je voudrais dire, donc, c'est le 1er écueil, le deuxième c'est comment peut-on imaginer qu'on aura plus de de médecins qui seront maître de stage, quand on voit simplement les courbes de nombres de médecins généralistes depuis une vingtaine d'années et que ça va continuer puisque de toute façon, il faut regarder tout simplement l'âge de nos médecins généralistes et donc il y en a plein qui partiront, et qui ne pourront pas être maître de stage, on en a même pas 12000 comme il faudrait en avoir aujourd'hui donc comment trouverons-nous ceux qui seront nécessaires pour 7 appliquer cette PPL, donc je vois que Montand est terminé, en tout cas moi je m'abstiendrai sur cette proposition, Merci, cher collègue, et la parole est à Emmanuel Capus du groupe, les indépendants. la proposition de loi qui est présenté aujourd'hui, elle va exactement dans le même sens que celle que j'avais co-signée de mon collègue Daniel Chassain, qui était inscrite à l'ordre du jour de jeudi prochain dans la niche des indépendants et que Daniel Chassain donc retiré puisqu'elle était exactement sur le même sujet et elle proposait exactement le même type de solution que celle d'aujourd'hui, je pense qu'il faut dépasser les groupes politiques et se réunir sur ce sujet, pourquoi, parce que dans nos territoires et cela concerne tous les territoires, dans d'autres circonstances, dans nos circonscriptions, en Maine-et-Loire, il n'y a pas une commune qui n'est pas confronté à cette difficulté, je ne parle pas des, des, des médecins spécialistes pour lesquels les rendez-vous cette ah si, moi je parle des généralistes pour lesquels quand il n'y a pas de médecin, il y a pas de médecins et les rendez-vous sont il y a pas de rendez-vous en fait il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui on répond à la population, y compris à Angers mais pas que dans les zones rurales, on répond si vous n'êtes pas aujourd'hui notre passion, nous ne vous prenons pas, point à la ligne, et c'est la raison pour laquelle nous avons autant de personnes qui ne sont pas suivies, donc il y a urgence il y a pénurie et cette pénurie qui fait face, ce sont les maires qui se débrouille dans certaines communes, certains ingénieux ont salarié leur leur médecin il lui font d'ailleurs souvent une opération financière relativement intéressante dans d'autres ils construisent des maisons de santé à leur frais dans d'autres encore, ils font venir des médecins Roumains ou d'autres pays, partout c'est la débrouille, donc nous devons aider les maires ruraux à trouver des solutions, celle qui est proposée aujourd'hui est une bonne bonne solution, elle passe également parce que Élisabeth Doineau a raison par une solution extrêmement simple et que je pense qu'il est soulevé sur chaque banc, ça passe par l'adhésion évidemment des étudiants internes en médecine et donc par une juste rémunération de l'effort et qu'qui qu'ils font au service, notamment de la ruralité. Merci, cher collègue, la parole à notre collègue Sonia de la Provoté. Oui merci monsieur le président, chers collègues, un médecin généraliste, un médecin de famille, c'est un choix des jeunes qui s'engagent dans cette voie sont les pivots, les piliers de la de et ils ont vraiment à coeur, profondément le service public et l'écoute des autres, pourquoi il s'installe pas, voilà pourquoi il ne s'installe pas une fois qu'ils ont fait leurs études pourquoi il remplace longtemps pourquoi ils sont rémunérer la consultation, moins de la moyenne européenne, pourquoi ils choisissent des exercices particuliers en cours de carrière parce que ils sont, ils ont de telles contraintes d'exercice qu'ils choisissent de faire autre chose que que cet exercice là pourquoi elle se salarie la sécurité sociale salarie des médecins, parce qu'on a des médecins coordinateurs parce qu'on trouve tout un tas de postes pour lesquels on emploie les médecins autre chose qu'aux soins de 1er recours c'est pas mieux, médecin généraliste, qui sont un tiers, un tiers des médecins de promotions reçues à l'internat et parmi eux, au final, on ne retrouvera qu'un cinquième, à être en soins de 1er recours auprès des habitants dans les territoires, alors moi je ne voterai pas cette proposition de loi parce qu'on n'a pas à régler les questions, on n'a pas réglé la question de la la rémunération, on n'a pas régularisé régler la question de la qualité de l'exercice, on n'a pas réglé la question de considérer que, finalement, c'est leur rôle à eux qui est le plus important et le pilier notre médecine je vous remercie. Merci, la parole maintenant à Bruno Belin. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, on va pas revenir, comme l'a fait Bernard Jomier sur ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans, c'était au tournant des années 90 on a baissé les numerus clausus chers collègues uniquement à l'époque, rappelez-vous, parce qu'il fallait faire des économies de sécurité sociale et on a sacrifié des vagues d'étudiants qui ne seraient bien utiles aujourd'hui ah mais Monsieur le Ministre. Notre journée historique je comprenne date tous les deux et vous devant notre assemblée, bien évidemment, parce que, on nous a raconté qu'à la fin du numerus clausus tout allait allait bien et on invente ce que aucun de nous, aurait été capable d'expliquer : il y a 6 mois. Le numerus apertus alors en attendant le numerus Proximus. On a le droit au numerus apertus alors le numerus apertus pardonnez-moi de prendre une minute 10 pour vous l'expliquer, c'est ce sont pardon les universités qui fixent elles-mêmes le numéro nombres d'étudiants quels sont en volonté. Ou en capacité de former et donc des riches font des riches et des pauvres font des pauvres et donc, vous trouverez toujours plus d'étudiants formés à Paris-Ouest que vous pouvez trou en trouver à Clermont-Ferrand ou dans d'autres universités de province et donc moi je prends date, monsieur le Ministre, chers Docteur numerus apertus. On a bien compris que c'est la règle, maintenant il va falloir nous en faire vite l'évaluation c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé concrètement dans toutes les universités françaises catégories de médecins par catégorie de professions de santé, combien de places sont donnés qu'est-ce que ça va donner, êtes-vous prêt à le réévaluer, êtes-vous prêt, elle expliquait qu'elle est la transparence sur le numerus apertus merci Monsieur le Président. Merci, cher collègue, la parole maintenant à Patrice Joly. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, je suis très surpris effectivement que cette PPL au départ qui avait vocation explicitement à traiter des déserts médicaux se trouve avec un intitulé qui est amputé d'une partie du sujet qui est essentiel, je suis surpris parce que l'enjeu aujourd'hui de l'accès à la santé dans les territoires ruraux, notamment mais pas seulement bien sûr et et véritablement majeur, c'est l'égalité aujourd'hui qui est bafouée, avec des conséquences sur la qualité de vie de nos concitoyens avec pire des conséquences sur l'espérance de vie de nos concitoyens des écarts pouvant aller jusqu'à 5 ans comme dans mon département, la Nièvre, il y a donc urgence, urgence sanitaire bien sûr urgence politique aussi dans l'attente de nos concitoyens et grande pour une prise en main par les politiques de l'organisation de la présence sanitaire sur notre territoire pour cela, il faut redéfinir les zones dites surdotées et celles dites sous-dotées, sortir de la théorie de la prise en charge de optimal du nombre de patients du nombre de patients par médecin au regard de la pénurie que nous vivons aujourd'hui les zones Soudan sont des zones dont le nombre de médecins est inférieur à la moyenne nationale et les zones sur-denses sont des zones dans lesquelles le nombre moyen de médecins et supérieur à la moyenne nationale et c'est aussi simple que cela, urgence de cette reprise en main, je le disais, c'est le sens de la PPL qui a bien voulu évoquer notre collègue Jean-Pierre Sueur tout à l'heure PPL que j'avais déposé en août dernier, avec comme principale disposition une régulation en matière de conventionnement, la réduction de la possibilité de faire des intérims pour éviter, sortir de ce scandale, garantir des aides à l'installation pour les employeurs qui embauchent des, des, des médecins, comme pour les libéraux, il y a urgence, urgence, Monsieur le Ministre, les Français sont en souffrance, les Français souffrent, monsieur le Ministre, au secours, au nom des territoires, les habitants des territoires ruraux, agissez concrètement agissez vite. Merci monsieur le président, je suis assez gênée, vraiment gêné de prendre la parole à ce stade, mais je tiens à prendre quand même parce que je suis gêné pourquoi parce qu'il s'agit de parler de la formation des internes en médecine générale et je crois que parler de la formation des ethnies, des internes en médecine générale, ça me pose un problème parce que, préalablement, et ça a été, il il s'agissait de parler des déserts médicaux en même temps, c'était le titre initial en tout cas c'était une partie de l'intitulé sur les territoires d'outre-mer, mais c'est aussi partout en France, il y a de vrais problèmes, on ne parle pas à ce stade et j'ai entendu les différentes prises de parole, la qualité, la qualité des soins, l'aménagement du territoire, c'est vrai, ça été évoqué, mais je crois qu'il y a de vrais problèmes et que cette PPL ne peut pas résoudre intégralement les difficultés que rencontrent nos territoires je crois également que la qualité de vie des étés, hein, parce qu'on parle des internes, quand on regarde la charge de travail qui font, moi j'ai trouvé en milieu hospitalier, ce sont des personnes qui travaillent, qui supplée qui prennent des responsabilités, il y a de vrais sujets et là je vois qu'qui seront exploités, ils ne sauront pas correctement payés, on attend beaucoup de pour nos territoires ça peut apporter une réponse, certes, mais est-ce qu'on parle de ce qui pendant le confinement pendant toute la période sanitaires se sont suicidés, ils ont été à peu près onze il faut parler de ça aussi de la qualité de vie de ces personnes, sur lesquels nous comptons alors aujourd'hui je crois que nous nous trompons quelque part parce que dissocier les problématiques de l'aménagement du territoire de la qualité de vie de ces personnes là la qualité de vie, de la santé dans notre population, hé bien je crois que c'est une grave erreur, merci. Merci bien, chers collègues, nous en avons terminé avec les interventions générales sur Arte sur l'article unique et donc nous allons passer à l'examen des amendements donc le premier amendement l'amendement 9 présenté par Monsieur Merci me ce président donc logiquement découlant des interventions que nous avons fait dans cette première partie d'examen du du texte cet amendement, il vise à à prendre acte du fait qu'une année de professionnalisation doit être mise en place et a renvoyé à la négociation avec les organisations concernées, des conditions et on les a beaucoup entendus les conditions j'ai entendu beaucoup de collègues, dire que la question des rémunérations n'était pas réglé que la question des, des, des, des lieux d'affectation n'était pas réglé que la question des moyens matériels n'était pas réglé, tout ça, tout le dispositif doit être négocié, le problème c'est qu'en créant, encore une fois brutalement la quatrième année d'internat de médecine générale, vous avez l'organisme l'ensemble des internes et de leur organisation syndicale qui sont en grève, qui dénonce à la fois l'article 23 du PLFSS qui effectivement exactement le même et cette proposition de loi parce qu'elle s'assied, elle fait fi de la phase de négociation ce n'est pas l'heure pour nous de figer le dispositif, vous faites une erreur moi je vous appelle à adopter cet amendement qui permettra de poser un principe de renvoyer à l'organisation entre les parties prenantes, et il sera temps, un peu plus tard et pas trop tard, j'en suis bien d'accord, mais un peu plus tard, en fonction du résultat de ces négociations, d'adopter un dispositif définitif. Bien, merci, avis de la commission sur cet amendement. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord en en préambule, je voudrais dire que la proposition de loi n'est pas n'est pas amputé du sujet sur la démographie médicale, bien sûr, elle est en elle est amputée de termes déserts médicaux qui ne correspondent pas à la réalité de nos territoires, il y a des problèmes de démographie médicale, partout en France, 85 % du territoire national et Alain Milon, rappelait le titre d'un livre que je ne connaissais pas Paris et et c'est désert.

simplement le le terme de désert médical d'abord, il le terme de désert médical d'abord, il est, je veux dire il est nocif à l'installation des médecins, il donne une mauvaise image de ce que sont les territoires sous-denses ensuite attendez vous vous vous prendrez la parole après mes chers collègues, mais ensuite, je voulais juste dire à Bernard nous respectons les internes en médecine, nous les respectons, si nous les respectons la preuve en est c'est que avec cette proposition de loi, si elle est adoptée en fin de 3ème indécis hier en début de 4ème année ils seront Docteur junior et nous défendons l'idée c'était dans l'exposé des motifs de la proposition de loi d'une rémunération à l'acte et tout à l'heure et on l'a examiné en commission tout à l'heure, il sera présenté par le Docteur René-Paul Savary, un amendement un amendement justement où nous demandons une dérogation à la rémunération des docteurs juniors en médecine générale parce que l'effort qu'on leur demande ses sites reconnaissance et impose reconnaissance et je vous rejoins parfaitement, il n'est pas tolérable que des médecins en quatrième enfin futurs médecins et des internes en 4ème année de médecine générale avec le le savoir qu'ils ont mérite reconnaissance. Sur cet amendement, moins sa secondes ça va être court mais en en instaurant une année de stage supplémentaires pour les étudiants en médecine générale sans l'inclure dans l'internat, cet amendement ne permet pas de compléter le troisième cycle de de médecine générale en lui rendant applicable les avancées permises par la réforme de 2017, donc l'ajout d'une phase de consolidation 3ème cycle de médecine générale parce qu'elle précipite la soutenance de thèse et d'un accès à des stages en en autonomistes Berbizier est essentielle à cette réforme et à la reconnaissance le, le titre de Docteur junior, donc moi je souhaite comme vous, mon cher collègue que soit défini les modalités. De rémunération adaptée à cette 4ème année il a ses contraintes, l'inclure dans la troisième année de cycle de médecine générale n'empêchera pas le gouvernement et je compte sur vous Monsieur mise de le faire, c'est un avis défavorable de la commission.

madame la rapporteure, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Jomier l'ajout d'une 4ème année au au diplôme au DES de médecine générale a justement pour objectif de doter cette spécialité d'une phase de consolidation de professionnalisation cette phase permet à l'interne d'acquérir de l'autonomie d'un cadre protecteur de la supervision, à l'instar d'ailleurs des autres spécialités médicales. Par ailleurs, je ne suis pas favorable à la réalisation de cette année de façon obligatoire dans une zone sous-dense, je ne crois pas à la concertation, non par dogme, mais parce que la concertation ne fonctionne pas, elle est même contre-productive, je souhaite enfin que les modalités de rémunération puissent être concertés dans le cadre de la mission que nous avons confié avec la ministre. De l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous remercie de vous interroger sur la rémunération des internes en médecine générale, tout en précisant que c'est le même problème avec les internes des autres spécialités pour toutes ces raisons je suis et le gouvernement est défavorable à votre amendement. merci Monsieur le Ministre, donc un double avis défavorable monsieur Ouzoulias. Merci monsieur le président, merci Monsieur le le ministre sur cet amendement, nous avons un doute, un doute fort qui tient aux capacités du législatif, nous sommes tous très attachés à l'autonomie des universités, j'ai cru même comprendre que Madame Pécresse a fait une partie de sa campagne électorale sur ce point, l'autonomie des universités, comme le disait très justement Monsieur Jomier dans son intervention générale pour la première fois le législateur va intervenir dans un cursus universitaire est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire et du changement radical que vous êtes un train d'impulser avec cette loi, dans la relation que le législatif ah avec l'université, comprenez bien que si vous touchez, comme vous le faites aux études, vous touchez aussi au master, c'est-à-dire que vous remettez en question tout le processus de Bologne, alors moi je suis favorable à cette discussion, mais moi je j'avais compris que c'était pas tellement votre position illogique vous en changer, ça serait bien de nous l'expliquer, merci monsieur le président. Monsieur Jomier. je remercie la rapporteure pour la précision de sa ses réponses et de ce dialogue, mais madame la rapporteure, que vous ayez supprimé le terme déserts médicaux, personne n'en est chafouin, par contre vous avez effacé, vous auriez pu parler de dispositifs visant. à développer, à améliorer l'offre, l'offre de soins dans nos territoires, parce qu'on le voit bien, encore une fois, nous ne parlons que de ça que de ça dans cet hémicycle mais on les fasse en même temps, et donc c'est la confusion et ne cherchez pas ailleurs, la raison de la grève des internes, ne cherchez pas ailleurs, la raison de leur manifestation et leur opposition à votre proposition de loi et à l'article 23 telle qu'il est rédigé. Alors quoi, on est là pour décider du mode de rémunération. Eh bien moi je je ne préempte pas la question de savoir si, lors de cette année, ils devront recevoir une part fixe salariale une part à l'acte, un mélange des deux une unicité de l'un ou de l'autre, c'est la négociation qui dit ça, les corps intermédiaires, on les a méprisé pendant tout un quinquennat nous avons tenu le discours les revaloriser et au moment de, de mettre en place un nouveau dispositif, on ne les consulte pas, on vote avant la négociation, hé bien, oui, on met la charrue avant les boeufs, il faut d'abord négocier et après adopté le dispositif et c'est pour ça que nous maintenons cet amendement Madame Goulet. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous avez dit dans votre explication, il y a quelques minutes, que vous n'étiez pas fort pas favorables à la concertation, je pense que c'est à la coercition d'accord on est, on est un peu, on est on est

parce qu'alors à ce moment-là, à quoi servait le CNR, moi je trouve qu'il a pas beaucoup d'utilité, mais enfin bon, voilà, c'est quand même soi-disant un un organisme de concertation, alors nous, au niveau du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste on a, je crois bien exprimé notre désaccord avec cette proposition de loi, en tous cas de manière claire et on ne va pas rentrer dans le jeu des amendements parce qu'on pense que de toute façon c'est mauvais, c'est pas comme ça qu'on redresse les choses, d'abord par rapport à la façon dont on traite les internes et y compris par rapport à ce que l'on vit dans nos territoires, quels qu'ils soient ruraux ou urbains, ça n'est pas comme ça qu'il qu'il faut faire, il faut desserrer l'étau effectivement du numerus apertus et puis, mes chers collègues, j'aimerais quand même attirer attirer votre attention sur une chose : je n'arrive pas à comprendre que la majorité des jeunes médecins sont plutôt attirés par un exercice en équipe, un exercice salarié et que, au travers d'une PPL ou d'amendements, on les encourage à travailler en libérale, là il y a quand même un hiatus, c'est-à-dire que vraiment on ne veut rien entendent de ce qu'est la situation réelle de ces internes et on veut, on alors que on laisse, par exemple, d'autres propositions, je pense notamment aux gardes, etc, pour l'ensemble des médecins qu'ils soient, pas seulement en public, mais aussi en privé, on les laisse faire ce qu'ils veulent, là il y a vraiment 2 poids 2 mesures.

on a des enfants en bas âge. Et il y a énormément de femmes évidemment et le conjoint ou la conjointe sont déjà engagés dans la vie professionnelle. C'est quand même compliqué de leur dire après cet engagement volontaire d'exercer en médecine générale, qui est quand même. Par les temps qui courent, un vrai enfin une vraie volonté à vrai sens aigu du service public et du service rendu à la population, c'est quand même compliqué de leur dire que, à la fin tout à la fin, quand la vie personnelle et lancé quand ça devient compliqué, hé ben non, il va falloir aller dans un désert médical ou l'équivalent dans les airs, médical, en tout cas plus loin de là où on habite, pour pour boucher les trous des carences des politiques publiques en matière d'accès aux soins, ben moi je trouve que ce message-là, il est pas audible et en tout cas, il est pas acceptable et c'est pas un message qu'on doit transmettre à des jeunes qui, demain, sur lesquelles vont reposer demain la responsabilité de la prise en charge dans tous les territoires, je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Président, moi je voudrais recadrer un petit peu les choses, j'ai participé à un certain nombre douze ici on la quatrième année, elle tombe pas du ciel quand même hein, ça fait des années et des années qu'on parle d'une 4ème année à l'identique des 43 autres spécialités à ce que le médecin généraliste soit reconnue comme la que la médecine générale soit reconnue comme une spécialité. Ces revendiqué depuis très longtemps, simplement, ça a été mis un peu sous le tapis, peut-être par manque de courage au fil des années pour annoncer la couleur, là au moins il y a une clarté et d'ailleurs quand il s'agit de formation, les internes savent bien que si c'est pour une formation justement à l'installation, c'est d'autant plus intéressant et puis je voudrais désamorcer un petit peu du côté de ces ces territoires, ils vont aller sur des territoires qui sont plus ou moins attractifs, effectivement, mais qui peuvent être très attractif, mais où il y a un agrément d'un médecin stagiaire universitaires quoi qui va les prendre en main, alors si un territoire rural n'a pas de maître de stage, universitaire, il aura pas d'internes. Attention donc la formation correspond à un agrément un suivi avec un maître de stage, qui peut être sur n'importe quel territoire, hein, c'est la raison pour laquelle il faut faire, être tout à fait attentif à cela, moi je ne crois pas qu'on va les maltraiter quand même. Sûrement pas autant qu'ils le sont peut être déjà à l'hôpital, ils vont bénéficier d'une vie nouvelle découvrent des malades dans des territoires extraordinaires parfois et je suis sûr que ça les convaincre d'aller s'installer et pas forcément en libéral, pas forcément libéral derrière, ils peuvent avoir une activité professionnelle au choix en fonction de leur choix, il n'empêche que c'est une année de profit de professionnalisation tout à fait importante et qui mérite peut être monsieur que le ministre-qu'on se penche sur les 2 cycles précédents, pour faire une année de moins, parce que 10 ans c'est long et on résumerait des 6 cinq tout le monde y gagnerait. Merci, cher collègue, la parole. Ah, ah Monsieur Chassang.

quelle est la portée de cette proposition de de loi et en fait, bon, il exprime à la fin, la nécessité de donc les, les, les étudiants en quatrième année, moi je suis. Favorable, j'ai proposé tout à l'heure, mais ça, ce sera à voir en dans un 2ème temps avec les étudiants, il est évident qu'après 10 ans, on ne peut pas les payer 2000 euros par mois c'est c'est surtout leur leur gros problème quand on parle avec eux, si vous voulez, et puis je pense que, y faut alors j'avais proposé moi dit consultation par par jour parce que lorsque un médecin qui a une clientèle qui où il qui est surbooké, il va faire appel à un jeune médecin bien il pourra lui donner facilement 10 consultations par jour et être là au cas où il y a un problème pour le le conseiller et je voulais également dire que les ne plus parler de déserts médicaux par les 2 zones sous-denses mais il faut quand même que les médecins sont là pour soigner, ils sont là pour aller dans des endroits où on a besoin de c'est leur vocation, ils ont fait médecine pour ça, donc je ne vois pas quel est le le problème de demander un an pour des médecins pour des jeunes médecins à aller dans des zones où il y où il où on a besoin de, je ne vois pas quel est le problème et la plupart sont d'accord, c'est un problème de rémunération. merci, après cette intervention, la présidente Catherine Deroche et ensuite, je pense qu'on passera au vote sur la. Merci monsieur le président, je voulais parler de cette place de de cette PPL dans la loi, mais je rappelle qu'en 2019 on avait mis quelque chose dans la loi pour la 3ème année et demain nous allons voter, proposition de loi pour les sages-femmes sur lequel votre groupe et et en effet moteur et et est très porteur, on touche en effet hein que parfois les ce que la formation des professionnels de santé, demain ce seront des sages-femmes, alors c'est vrai que le cursus est différent de celui des médecins, mais c'est quelque chose que l'on fait que l'on fait régulièrement et puis je voulais dire, bon je, je sais ce qui a été le travail de commissions d'aménagement du territoire depuis des années sur ce sujet, moi quand j'étais conseiller régional, à la demande du président Retailleau j'avais fait le plan santé de la région des Pays de la Loire en 2015 dans le cas de la commission aménagement du territoire de la région, donc on est sur l'aménagement du territoire, mais ce que je veux dire c'est qu'il a pas opposition de la commission des affaires sociales, les autres commissions commission des affaires sociales, nous sommes tous des élus locaux, nous connaissons nos territoires, nous savons en effet ce qui s'y passe et et c'est pas du tout une opposition entre commissions sur ce sujet-là, bon, après, qu'on soit pour ou contre la coercition, c'est un vrai sujet, moi je n'y suis pas favorable parce que je pense que c'est pas une solution est partout, elle a été faite, ça n'a pas marché partout à la défaite, ça n'a pas marché, lisez, lisez le le rapport, c'est le rapport qu'on a eu de benchmarking sur sur ce de pardon. De madame Paul ton sur le sujet, partout on est on on arrive de Suède avec la commission des affaires sociales, je peux vous dire qu'ils ont les mêmes problèmes d'attractivité pour les professionnels de santé, que ce soit les médecins et les ou les paramédicaux, ils ont les mêmes problèmes que nous, donc c'est et avec un système totalement différent, donc je voulais quand même préciser ceci. Bien, merci, nous allons passer au vote, donc sur l'amendement, je rappelle qu'il y a 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement, donc il est pour cet amendement. Qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté ensuite 2 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune le 1er présentée par Madame Gerbaud. Merci monsieur le président, cet amendement propose d'affecter les étudiants de 4ème année en priorité dans une zone de sous-densité médicale situé dans la région à laquelle appartient la subdivision territoriale de leur faculté de formation, le but de ce fléchage et d'éviter un phénomène d'appel d'air, incitant les étudiants d'un territoire régional à délaisser ce territoire au profit d'autres zones sous-denses malgré tout plus attractive, à leurs yeux, en d'autres termes, nous souhaitons éviter que les territoires de rattachement naturel des stagiaires ne se trouve spolié du maintien sur place de leurs étudiants par l'attraction relative de textes secteur objectivement moins défavorisées. bon. Président, mes chers collègues, c'est un peu dans la même philosophie, cet amendement propose que les étudiants en dernière année d'internat qui effectuent leur stage dans le territoire où ils ont réalisé leurs études, il paraît normal que le territoire qui forme des médecins puissent bénéficier des forces vives parce que, effectivement, dans ce territoire, ben les étudiants viennent de des fois de territoire très éloignées et je pense que, ils doivent rester pour leurs dernières années dans le territoire, cela permettra également une meilleure répartition des internes sur les territoires de plus c'est une réponse supplémentaire, donc à l'objectif initial de la proposition de loi savoir lutter contres les zones sous-denses. donc madame la rapporteure, avis de la commission sur ces deux amendements. dont il relèvent je comprends l'intention des auteurs qui est d'éviter que les internes qui étudie dans une faculté de médecine délaissent le territoire où ils sont étudiants, cela pouvait présenter au départ des des difficultés parce que si le nombre de maître de stage n'est pas toujours proportionnée localement à la population des internes, il fallait pouvoir que ces étudiants exercent dans une autre région, à défaut de pouvoir le faire dans dans la leur, les amendements trois huit qui ont tous les 2 été rectifiée par leurs auteurs pour tenir compte de cette difficulté permettent désormais des exceptions, il n'exclut aucun territoire en conséquence, la commission a émis un devis favorable sur ces deux amendements. Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Goulet je vous remercie d'avoir corrigé mon lapsus non révélateur, bien entendu. Je suis un inconditionnel de la concertation et je suis fermement opposé à la coercition. l'affectation des internes se fait déjà dans la supplier dans la subdivision territoriale de leur faculté inscrire ces dispositions dans la loi, c'est par ailleurs se priver d'une éventuelle souplesse pour autoriser des exceptions utile à certains territoires, en particulier des territoires qui sont limitrophes entre 2 territoires de faculté, enfin, la répartition des postes d'internes n'est pas décidé seulement par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche mais conjointement avec le ministère de la Santé et de la prévention en tenant compte des besoins de santé des territoires. Pour toutes ces raisons je suis défavorable à votre amendement car déjà satisfait par les textes existent. donc nous allons passer au vote, si j'ai pas de demande d'intervention avec un avis défavorable de, du gouvernement et un avis favorable de la commission, donc il est pour l'adoption de ces deux amendements. Qui est contre. Qui s'abstient ils sont adoptés ensuite l'amendement 13 rectifié Monsieur Savary. Oui, merci, on a déjà abordé ce ce problème de la rémunération de cette 4ème année, donc je vous propose là de faire une dérogation au décret existant parce que tout le monde la la la, souligné, il faut trouver une rémunération à la hauteur de la formation de ces jeunes, il ne faut pas mettre à mal non plus : la rémunération actuelle des médecins spécialistes, c'est pour ça que, au départ il était préconisé de rémunération à l'acte, mais ça engendre des effets dominos difficilement maîtrisable, tandis que là, en faisant une dérogation par rapport au décret qui a été pris, ça permet d'avoir une rémunération auteur en, je trouve ça extraordinaire de pouvoir proposer ça sans avoir l'article 40,

une des années des des 2 premiers cycles. Pour que cette 4ème année de troisième cycle reste. 9 ans en tout pour pas allonger une année qu'elle soit pas contre-productif, mais là j'ai été, article 40. Une année de moi ça génère des dépenses supplémentaires mais une réponse supplémentaire, ça ne semble pas poser de problème, donc je soutiens bien sûr cet amendement et je vous invite, je vous invite à en faire autant. Non mais c'est pas la commission des affaires sociales qui s'auto-on est d'accord quand même des des contraintes pour revenir sur, sur l'amendement qui demande en fait qu'un décret soit publié, des contraintes spécifiques s'appliquant aux étudiants de de 4ème année de médecine générale auquel il est demandé de de faire un effort de réaliser des stages en exercice ambulatoire en zone sous-dense, il est normal que leurs conditions de rémunération puisse être adapté les étudiants devront être justement rétribué au regard du travail qu'ils fourniront et de la contribution qu'ils apporteront à l'accès aux soins de nos concitoyens gouvernement doit avancer sur ce sujet ces prochains mois en concertation avec l'ensemble et j'ai bien dit en concertation avec l'ensemble des parties prenantes, la commission donc formuler un avis favorable sur cet amendement. Avis du gouvernement. c'est justement l'un des objets de la mission que nous avons mis en place avec madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont les conclusions sont attendues pour le 1er trimestre 2023, je souhaite que ce sujet puis être travailler dans la concertation avec l'ensemble des parties prenantes, en prenant le temps nécessaire à son instruction en particulier vu l'incidence cela pourrait avoir sur les autres spécialités médicales pour toutes ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement. Bien Monsieur Savary, l'amendement est maintenu, j'imagine. Vous maintenez l'amendement parce que il y a une demande de retrait du gouvernement donc je vous pose la question, vous maintenez l'amendement. Bon, allez-y, allez-y. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, j'ai je ça ne m'a pas échappé, Monsieur le Ministre, que vous lanciez une concertation il n'empêche que, quel que soit le résultat de la concertation, vous serez amené à prendre une dérogation par rapport au décret, donc autant être concret autant montrer votre ouverture à une rémunération décente de ces interne en en quatrième année de de de derniers cycles, c'est la raison pour laquelle monsieur le Président, je maintiens, bien entendu, cet amendement. C'est entendu c'est noté monsieur Richard. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je voterai naturellement cet amendement parce que je l'ai cosigné et parce qu'il est apparu très clairement tout au long du débat que c'était une condition vraiment essentiels au fonctionnement de de cette démarche, présenté par la proposition de loi du président Retailleau mais permettez-moi juste de revenir sur l'article, je sais bien que c'est pas de la compétence de la commission des affaires sociales, comme l'a fait tout à l'heure monsieur Sueur sur l'article 45, il y a dans cette maison, un vrai problème avec ces limitations au droit d'amendement, là on a quand même René-Paul on a quand même là l'illustration claire des dérives liées à l'utilisation de cet article quarante lorsque j'ai cosigné cet amendement chez René-Paul je, je me suis dit je vais le signé mais attention à l'article quarante je me suis dit il a aucune chance de passer, ils passent, ils passent, mais l'autre, mais l'autre amendement que j'avais cosigné aussi et là aussi il y avait l'article 40 donc, franchement je sais j'ai déjà demandé ça ici dans cette salle, plusieurs fois on m'a envoyé un fascicule extraordinairement long, complexe élaboré par la commission des finances sur l'article 40, j'avoue que j'y comprends toujours rien, mais là, ça vaut vraiment le cas, ça vaut la peine de regarder très clairement comment on a pu à la fois appliquer ce ce fascicule hein, encore une fois et puis arriver à ces aberrations signalé par René-Paul Savary, vraiment je le redemande une nouvelle fois, examinons ce qui cette à faire des, des, des, des articles limitant clairement

prouve s'il en était la limite de la proposition de loi qui nous est proposé, on nous propose donc, on propose de mettre une dixième année sans avoir consulté sur la rémunération, on nous parle d'une rémunération à l'acte, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire, ces jeunes vont être volontaire pour aller dans une zone sous-dense, il y en a qui toucheront 5 actes. Par jour, d'autres en toucheront 10 d'Autrans toucheront 15, d'autres 25 il n'y a pas de cadre et donc on va créer des inégalités entre les jeunes eux- mêmes, vous dites non, mais si parce que ils seront payés à l'acte, donc ça veut dire qu'on va créer pour un même boulot des jeunes qu'on envoie en sous-denses qui ne toucheront pas la même chose, je trouve ça complètement scandaleux et c'est en ça qu'on voit la limite de votre proposition de loi. Merci Monsieur le Président, simplement je voulais apporter une réponse à notre collègue concernant la rémunération dans le texte dans la proposition qui est faite c'est une dérogation, donc ça laisse le temps à la fois de la concertation entre les étudiants et gouvernement de façon à ce que, à la fois on réponde aux attentes porté par ce texte de loi mais en même temps, hé bien aux attentes, porté par les étudiants, voilà, donc on a le temps de discuter et d'avoir quelque chose de cohérent sur le territoire national.

Je vais répondre à ma ma collègue en libéral, moi j'avais proposé qu'on puisse donner au aux internes de quatrième année dit. Consultation minimum mais il est évident que, vous savez quand on est en libéral, moi il y a des jours, on fait beaucoup plus de consultations, d'autres moins, c'est comme ça, hein, ce ce qu'on est un libéral,

bien sûr parce que si il n'en a pas besoin, il en prendra pas, il aura une besoins d'une clientèle, il aura besoin de médecins junior, parce qu'il a une clientèle où il est complètement débordé et avec le médecin junior il pourra arriver à la fois ah le conseiller et à la fois de faire du monde travaille et voilà et je pense que c'est une proposition, je pense que 10 consultations par jour lorsqu'ou travailler 5 jours par semaine, ben ça fait 5000 euros par mois voilà. Alors, nous allons passer au vote avec une un avis défavorable du gouvernement, un avis favorable de la commission sur cet amendement, qui est pour. est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté avant de passer à l'examen du dernière amendement, je veux juste signaler que nous sommes, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et par le groupe Les Républicains donc chacun peut se préparer dans les groupes à ce vote de scrutin public sur l'Arctique oui demande de scrutin public sur l'article donc dernière amendement sur cet article, madame. Merci. Six, président d'abord je voudrais remercier mes collègues ont cosigné cet amendement, vous avez dit monsieur le Ministre que vous souhaitez des solutions concrètes et pragmatiques, hé bien, cet amendement va pouvoir vous combler, en effet, cet amendement a pour objet de de dire quoi de dire que des médecins retraités puissent être médecin référent, pourquoi, parce que cela a été dit, il y aura une difficulté d'avoir des médecins référents en nombre et puis il y a dans nos territoires et dans beaucoup de nos communes, plus de médecins dans des communes, moi j'ai été élu en 2014, maire d'une commune de 2000 habitants Reuilly dans l'Indre, j'avais de médecins généralistes et et un chirurgien dentiste, aujourd'hui il n'y en a plus aucun demain si nous ne prévoyons pas la possibilité pour que ses médecins viennent accompagner ces étudiants et c'est tout à fait normal qu'il puisse être supervisé et accompagné, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'expérience de ces hommes est née ces femmes qui sont dans beaucoup de nos communes, toujours présent, et qui sont prêts à aider à l'installation,

mais c'est pas de chance, vous n'avez plus de médecin, alors vous n'aurez personne, il faut que demain et je sais que ça, ça relève du domaine réglementaire, j'en suis bien consciente mais vous savez comme moi que les débats sont là aussi pour éclairer la rédaction des décrets pour éventuellement aussi éclairer les contentieux possible, mais je souhaite monsieur avec cet amendement d'appel, je vous fais donc un appel, dites-moi, Monsieur le Ministre, que, il sera possible à des médecins retraités demain d'être des référents dans ce cadre-là, il faut l'organiser, ça peut être des médecins qui sont à la retraite depuis moins d'un an d'un an depuis moins de 5 ans, je veux dire, ou dix ans, je ne sais pas, mais en tout cas, il nous faut aujourd'hui le prévoit, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y a un avis de la commission sur cet amendement. Merci monsieur le président, monsieur Ministre, mes chers collègues, la réforme ne pourra réussir que si elle garantit un véritable accompagnement aux internes et améliore leur formation je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point, elle doit permettre aux étudiants de médecine générale de découvrir l'exercice ambulatoire en cabinet ou en structure d'exercice coordonné aux côté de praticiens en mesure de les accompagner dans l'appréhension de l'autonomie sur ce point à l'ouverture de la maîtrise de stage à des médecins retraités, je parle bien de médecins retraités qui n'exercerait plus risquerait d'envoyer un mauvais signal aux étudiants, la maîtrise de stage est déjà ouverte aux médecins en cumul emploi-retraite, je tenais à le rappeler, le gouvernement doit pouvoir accélérer le recrutement de maître de stage en exercice, ils sont aujourd'hui à peu près douze mille y compris et surtout en zone sous-dense pour permettre la pleine réussite de cette réforme, leur nombre a déjà beaucoup augmenté ces dernières années et de nombreuses collectivités s'emploie à favoriser la formation des maîtres de stage dans tous les territoires, je pense particulièrement au au conseil départemental de la. Maritime qui a, avec accord de la faculté de médecine de Poitiers, favoriser l'organisation des formations pour les maîtres de stage au plus près de leur lieu d'exercice dans les départements où il y a pas la faculté de médecine, je pense que c'est un on en a discuté avec notre collègue pour ces raisons, ma chère collègue, je vous demande de retirer votre votre amendement j'ai bien compris que c'était un amendement d'appel, à défaut, la commission a émis un avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis monsieur le président. Mais madame Bellion, vous avez une double demande de retrait. après, si vous le reprenez-vous l'. Prenez mais ce que je veux dire c'est que, concrètement, je sais qu'il y a un cumul emploi-retraite et que l'on peut à ce moment-là, mais il faut que on comprenait bien que, au moment de la rédaction des décrets et c'est une chose que je connais un peu, très vite on va évacuer ceux-là et ce n'est pas possible, vous n'arriverez pas cette réforme et nous n'aurons pas de médecin junior dans nos territoires, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'expérience de ces hommes et ces femmes qui sont prêts à venir aider dans des communes, il n'y a plus de médecin, donc il faut vraiment qu'il soit possible qu'il soit agréé qui soit agréé parce que demain, il ne faut pas venir nous dire ah écoutez, c'est dommage, on ne peut pas les agréer parce qu'ils sont plus médecin, ça fait un petit peu longtemps, voilà, je comprends que les jeunes puissent se dire qu'il faut peut-être des actifs, mais moi je peux vous dire que j'ai des hommes et des femmes qui ont été médecin dans ma commune, qui sont hyper compétents qui sauront parfaitement guidé, en plus, la patiente, elle, ils la connaissent et ils sont de bonne volonté, et ils sont compétents et ils peuvent encore aider, c'est ce que nous avons besoin, il s'agit de la vie d'hommes et de femmes aujourd'hui, et de leur santé, donc je veux bien le retirer mais je mets

donc nous allons passer maintenant au vote sur l'article, je rappelle que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes CRCE et les républicains sur cet article unique et qu'il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Bien, le scrutin est clos. Nombre de votants 344 les exprimer 328 pour 233 contre 95 l'amendement est adopté l'article est adopté, il nous reste un amendement. Après l'article unique, monsieur sol. Vous présenter. monsieur le président, mes chers collègues, dans un contexte de crise cet amendement André à inscrire le fait que le rapport de la part des étudiants se destinant à la médecine générale en 3ème cycle devrait être inversé, je propose donc que la part des étudiants en médecine générale en 3ème cycle soient supérieures à la part dédiée aux spécialités. Dans une proportion de 70 pour 130 % une telle mesure, je pense à lutter contre la pénurie médicale et rejoindrait l'objet de la proposition de loi, je vous remercie. La médecine générale est, et de loin, la spécialité recrutons le plus des. étudiant en médecine, elle concentre environ 40 % des étudiants accédant au 3ème cycle son recrutement augmente chaque année plus de 100 étudiants par exemple supplémentaire en 2022 par rapport à l'année précédente en prévoyant que la médecine générale devra concentrer à compter du 1er janvier 2025 au plus tard 70 pour 100 des postes ouverts aux étudiants de 3ème cycle cet amendement risque de placer les autres spécialités dans la difficulté, la médecine d'urgence, la réanimation ou la gynécologie obstétrique par exemple ne sont la pédiatrie bien sûr madame la présidente, ne sont pas moins essentiel à l'accès, ce soit de nos concitoyens, c'est pourquoi la commission a formulé sur cet amendement, un avis défavorable. Même avis monsieur le mieux disant même avis défavorable. Mais ma vie, donc un double avis défavorable, vous maintenez l'amendement monsieur sol. J'y crois, donc je le maintiens, merci. Qui donc nous allons passer au vote sur cet amendement. Madame de la Provoté excusez-moi je vous savez pas. Oui je je suis défavorable, parce que là on parle des médecins généralistes. Mais on ne Chicken gynécologie obstétrique, je vous signale juste que c'est juste. Un problème alors ça concerne les femmes, on est d'accord, mais quand même, c'est un vrai sujet en ophtalmologie c'est un sujet en anesthésie-réanimation, c'est un sujet aussi dans certains types de chirurgies, on est aussi en déficit de présence dans les territoires, donc on peut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre, on a besoin de tous les types de médecins, on a besoin de grossir globalement les promos de faire les choses plus vite et mieux dire, une complicité, je peux le dire comme ça, collectif pour avoir pendant des années, pas formé assez de médecins et puis remettons les CES parce qu'après tout, les médecins généralistes qui sont bons dans plein de domaines qui sont polyvalents, qu'il redevienne gynécologues médicaux qu'il redevienne cardiologues de ville, enfin bref, on a tout fait pour moquer et de spécialistes et manquer de généralistes, donc je pense que sur la portion congrue, qui nous est proposé dans les effectifs de l'internat ne mangeaient pas là 2 mangeons pas la part des autres, je vous remercie. nous allons passer au vote sur l'amendement donc avec 2 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient l'amendement n'est pas adopté, donc on va passer aux demandes d'explications de vote sur l'ensemble de la proposition de loi je je signale je suis également saisi d'une demande de scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi, donc vous pouvez également vous préparez donc je passe la parole à notre collègue Alain Houpert. Monsieur le président, monsieur le Ministre Mesdames les rapporteurs. Cette proposition de loi. Pose une bonne question sur la démographie médicale, mais apporte-t-elle une bonne réponse. Je ne pense pas que ce soit une bonne réponse. Parce que, en médecine, on traite toujours la cause et on ne traite pas la cause est la cause des déserts médicaux, dont on ne veut pas parler. C'est l'aménagement du territoire qui a toujours été un voeu pieux, on en a beaucoup parlé, mais on n'a, n'a jamais fait. Il n'y aurait pas de déserts médicaux. Si les territoires était plus attractif et si les banlieue était plus sûr. Un étudiant pour un stage de quatrième année dans un territoire défavorisé c'est délocalisé déplacer une famille pendant un an, s'est déplacé, le conjoint, c'est trouver des logements, trouver des écoles, trouver des garderies, trouver des collèges, trouver des lycées et trouver des moyens de culture à des gens qui ont été pendant 10 années dans l'université l'université en milieu urbain, souvent, on explique que les étudiants en médecine sont favorisés parce que l'État leur a payé leur médecine mais le sénateur aux Zulia, ça fait de l'archéologie est un merveilleux aisément expliquer que les médecins rembourser leurs dettes en renforçant l'hôpital et l'ont remboursé largement donc choisir un maître de stage, c'est difficile de choisir un maître de stage, les médecins spécialistes peuvent choisir un maître de stage, les médecins généralistes ne peuvent pas renforçons la très vite d'attractivité des territoires et ne faisons pas un service médical, à l'instar du service militaire, que certains ont connu et arrêtons d'embêter les étudiants en médecine, merci. Merci, cher collègue, la parole est a Hervé Maurey. Merci monsieur le président, monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voterai cette proposition de loi qui est une des 16 propositions qui figurait dans le rapport que nous avons commis et que Jean Luc fiché, il y a 10 ans et qui s'appelait déserts médicaux agir vraiment, c'était il y a 10 ans et, malheureusement, depuis, on n'a pas vraiment agi et les choses n'ont pas beaucoup bougé et je me souviens de de Madame Bachelot à ce banc au moment de la discussion sur la loi qui porte son nom, qui nous expliquait que c'était un mauvais moment à passer et que dans 10 ans tout ça serait arrangé, malheureusement on est 10 ans après et les choses n'ont fait que sa grand-mère ce que s'aggraver, donc je voterai ce cette proposition de loi, elle sera certainement adoptée mais sera-t-elle appliquée, il y a nous, de nombreux exemples de dispositifs qui ont été votées en la matière, à commencer par le dispositif dont on a parlé tout à l'heure de la loi de 2019 qui prévoyaient un stage obligatoire à partir d'octobre 2021, le décret n'ont jamais été pris donc à quoi ça sert de voter des dispositifs si ensuite ils ne sont pas appliquées, mais je suis aussi convaincu et je ne surprendrai pas grand monde dans cet hémicycle, que l'on ne réglera pas le problème avec ce seul dispositif et je demeure convaincu qu'il faudra, je le disais déjà il y a plus de 10 ans un jour installé une régulation à l'installation et la régulation, ça n'est pas la coercition, nous l'avons fait en France avec un certain nombre de professions de santé, notamment pour les kinésithérapeutes avec des, des, des succès qui ont été reconnus, ça se fait dans de nombreux pays, je ne vais pas développer, parce que je vois que le temps est extrêmement compté mais je crois que face à l'échec parce que personne ne peut contester l'échec des politiques mises en place depuis bientôt 30 ans, qui repose uniquement sur l'incitatif, hé bien il faudra un jour que l'on ait des gouvernements courageux pour oser déplaire au médecin parce que je comprends tout à fait, ce qui a été dit sur les médecins sur la difficulté de leurs études, j'ai moi-même une fille médecin mais je crois, quelque chose d'encore plus important que le confort des médecins, c'est l'accès des patients à une médecine de qualité. La parole à Nathalie Goulet. il a fallu qu'Alain Vasselle, quelques mois après, dépose une proposition de loi pour supprimer, c'est l'article qui était un peu coercitif, au motif que ça avait provoqué une bronca chez chez les médecins, donc moi je voterai aussi, évidemment, c'est cette proposition parce que le le sujet est évidemment plus qu'un irritant dans les territoires ruraux et dans les zones évidemment dépourvue de de médecins et que ce soit les les banlieues des grandes villes où les territoires ruraux que cet accès est extrêmement important, mais je trouve qu'il est est dommage que le débat se limite à la 4ème année, que ce soit seulement le 15 novembre qu'on ait un débat sur Parcoursup parce qu'en réalité la filière, elle est aussi bloqués à l'entrée, c'est aussi un échec de Parcoursup de, de, de démobiliser un certain nombre d'étudiants qui voudraient être médecins qui ne fonctionne pas, donc je crois qu'on a saucissonné le débat sur la quatrième année sur le sujet qui nous importe aujourd'hui mais j'ai quand même le sentiment, madame la présidente des roches le débat qui aura lieu ici le 15 novembre sur Parcoursup, répondra en partie si on arrivait à débloquer cette situation pour avoir plus d'étudiants en médecine, sachant que l'ensemble de nos territoires et c'est pas mon collègue Vincent Seguin à qui n'est plus là qui me démentira ah il a changé de place, voilà que le département de l'Orne, comme d'autres départements se sont mis à salarier les les médecins pour essayer de, de pallier les les manques et donc tout le monde fait beaucoup d'efforts, c'est un sujet éminemment important pour chacun d'entre nous, encore faut-il le prendre dans le bon sens, certes, la proposition de monsieur Retailleau est intéressante mais je crois que tant qu'on n'aura pas régler aussi le problème de l'entrée dans la filière et donc Parcoursup on aura des problèmes, donc rendez-vous le 15 novembre sur le débat sur Parcoursup. Merci, la parole à Alain Milon. Oui merci Monsieur prison je voulais moi, revenir sur la loi ma santé 2022, qui avait été proposé à l'époque par Agnès Buzyn et dont j'étais rapporteur, et je me souviens d'un amendement qui avait été présentées par Corinne Imbert qui qui proposé que la troisième année de spécialisation soit une année justement qui permettait aux étudiants de partir à l'extérieur et de se former dans les cabinets médicaux, les étudiants à l'époque nous avait dit une chose assez extraordinaire ce qu'ils estimaient que cette troisième année, il ne pouvait pas le faire à l'extérieur parce qu'ils étaient insuffisamment formés, j'ai été témoin ici qui ont assisté à cette réunion, dans la mesure où ils étaient insuffisamment formés, on a décidé de passer à 6 mois ce qui a été voté en CMP par l'Assemblée nationale et par le Sénat et une jamais appliquée par le gouvernement, cette fois-ci, donc on leur permet de faire une formation complète pendant 3 ans, puisqu'il souhaitait cette formation complète, ils la feront, mais ils font une formation en milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'ils apprennent à soigner les maladies, le diabète, hypertension, et cetera, et cetera, mais ce qui est intéressant dans la proposition qui est faite par Bruno Retailleau, c'est qu'en plus on leur propose d'aller travailler avec des médecins sur le terrain et d'entrer en contact, non pas avec les maladies mais avec des patients, ce qui est pas du tout la même chose, soigner quelqu'un en cabinet en individuel ou soigner quelqu'un sur un lit avec un chef de clinique en interne un patron, ça n'est pas du tout la même chose donc il était extrêmement intéressant que nos étudiants puissent faire cette 4ème année d'autant plus que lorsqu'ils ont été jusqu'à présent lorsqu'ils ont terminé leur 3ème année, seuls 30 30 % s'installer définitivement et immédiatement les autres attendaient faisait des remplacements et caetera, cette fois-ci, on aura l'intégralité des étudiants en médecine générale qui iront chez un médecin généraliste qui termineront leur formation au contact Direct de patients et pendant ce temps,-là préparons le dos dans le doctorat, donc c'est une c'est un une proposition de loi qui est extrêmement intéressante et que je vous appelle à voter. Il reste encore deux, explications de vote, ensuite, je vous propose qu'on passe au vote sur l'ensemble du texte donc Daniel Chassain. monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma je voterai mon groupe votera aussi cette proposition de loi, d'abord je voudrais dire que dans les dans la ruralité, il y a aussi de la culture, il y a aussi des écoles, il y a aussi des des collèges même des lycées, pas très loin, bon c'est vrai que, il y a pas d'université, mais surtout il y a souvent pas d'emploi pour le conjoint et ça, c'est vrai que c'est difficile, parce que maintenant il y a quand même une grande féminisation de la médecine et mais les jeunes jeunes hommes aussi ne souhaite pas travailler bah 24 heures sur 24 et mais maintenant ça complètement évolué, il y a beaucoup moins de garde et maintenant la vie en rural et tout à fait compatible avec la vie que souhaite avoir les jeunes donc nous avions voté avec président Millon une hein. Projet de loi qui allait dans ce sens en 2019, n'a, il y a pas eu décret mais actuellement ça c'est encore beaucoup aggravée et les maires nous demande absolument, dans nos départements, dans nos cantons de d'avoir quelque chose d'efficace, non pas pour, on ne va pas punir les les internes, on leur demande : mais bien sûr et ça a été dit, il faudra qu'ils aient un salaire décent, parce qu'ils ont fait 10 ans et c'est normal que, au bout, hé bien il puisse avoir salaires des pour faire pour faire vivre leur famille mais on leur demande simplement pendant pendant cette 4ème année d'apporter ce qui est souhaitable, c'est-à-dire apporter la médecine dans tous les secteurs de notre pays et je pense que c'est ce qu'il faut faire, je, je pense que cette loi va permettre une amélioration donc je suis entré à cette loi. La parole à Daniel Breuiller. Cher collègue, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, un mot pour dire que si cette PPL évoque des sujets importants, elle passe à côté d'un examen en profondeur des mesures qui seraient nécessaires, pour à la fois améliorer la formation des jeunes des jeunes médecins et également répondre aux enjeux difficiles du manque de couverture médicale dans beaucoup de territoires au fond cette PPL contourne contourne les sujets essentiels de la nécessité ou pas de mesures de coercition de la question des formations initiales de la nécessité de concertation avant de légiférer notre groupe est favorable sur ces sujets comme sur d'autres, à ce que la concertation, pressé de la loi et parce qu'elle la suivent, c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette proposition de loi. Merci madame la rapporteure. Après le vote bien, donc nous allons passer au au vote, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi donc je j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les Républicains, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Bien, le scrutin est clos. Votants : 345 328 pour 232 contre 96, la proposition de loi a été adoptée. Je vais suspendre la séance. Pardon, pardon, excusez-moi, avant de suspendre la séance la parole à la rapporteure Corinne Imbert. merci monsieur le président, merci Monsieur le Ministre, merci pour votre écoute et pour votre avis de sagesse sur cette proposition de loi merci, mes chers collègues, pour la qualité de de nos échanges et merci à à l'administrateur pour m'avoir accompagné sur ce texte, cette proposition de loi du président Retailleau n'avait pas, n'a pas la prétention de de tout régler mais il était important qu'elle soit votée aujourd'hui, la situation actuelle en matière d'accès aux soins est insupportable. Pour un grand nombre de patients tu son portable pour les élus et il fallait apporter une première réponse, c'est un pas, ça n'enlève pas d'interne à l'hôpital public, bien au contraire, peut-être que le renfort et l'arrivée de Docteur junior dans les territoires évitera évitera l'arrivée aux urgences, de passion, parce qu'ils auraient été prises par un médecin en ville, on parle toujours du lien ville hôpital, l'hôpital ira mieux si la médecine de ville va mieux, c'est un pas, un pas demander aux internes en médecine générale, bien évidemment, hein, pas demander au ministère en terme en terme de reconnaissance hein hein pas demander au médecin généraliste installé pour demander qu'il devienne maître de stage, pas demander à la faculté pour faciliter la maîtrise de stage au plus haut au plus près de de lieux d'exercice, je pense que c'est tout l'intérêt de ces propositions de loi, donc merci à vous de l'avoir voté.

s'il vous plaît, faisons le changement dans le plus rapidement possible.

la séance est reprise, la parole est à Jean Michel Arnaud, pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, monsieur le président, je souhaite apporter une rectification de vote pour mes collègues Amel Gacquerre et Anne-Catherine Loisier concernant le vote en début d'après-midi, le scrutin, numéro 3 sur l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation du ministre, du ministre de l'Intérieur mesdames et Loisier souhaiteraient voter pour. Bien là acte est donné de cette mise au point, elles seront publiés au Journal officiel et figurant dans l'analyse politique du scrutin hein je oui la parole à Madame Frédérique Puissat pardon pour une mise au point au sujet d'un vote également. Merci monsieur le président, c'est sur le même scrutin public numéro 3 vous informer que mes collègues, Charles Guené, Gérard Longuet, Albéric de Montgolfier et Damien Régnard soit aussi voté contre ce pour pardon ce scrutin public. Bien, merci encore mes excuses donc acte et donner de ces mises au point, nous passons donc à l'ordre du jour qui appelle le débat sur les finances locales, une demande de la commission des finances, la parole et tout d'abord aux orateurs de la commission qui a demandé ce débat en commençant par monsieur Vincent Eblé, vice-président de la commission des finances. Je serai un peu intransigeant sur les temps de parole de ce débat parce que nous avons pris un peu de retard et il faut respecter la les conditions du débat de la séance de ce soir, donc nous serons de tenir dans les temps et je serai strict sur les temps de parole. Donc, Monsieur le Président, nous sommes contraints, avant et après, merci monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la loi organique relative à la gestion des finances publiques nous permet aujourd'hui en amont de la discussion du projet de loi de finances 2, consacrer l'organisation d'un débat à la situation des finances locales, nous sommes tous d'accord pour dire que cet exercice et bienvenue, Madame la Ministre, vous souhaitez supprimer la CVAE sur 2 ans pour soi-disant améliorer la compétitivité de nos entreprises industrielles pour autant cette suppression ne bénéficierait qu'à hauteur de 40 % à ces dernières et bénéficierait par contre à nombres de sociétés du secteur tertiaire, avec la suppression de la CVAE vous ne ciblait pas les les entreprises industrielles, tant qu'à vouloir soutenir la compétitivité de notre industrie, ne faudrait-il pas mieux conserver ses moyens pour faire face à la crise énergétique. Qui la touche de plein fouet. Par ailleurs, la compensation proposée inclut 2 années de crise sanitaire où nous avons observé une contraction du produit de la CVAE pourtant l'État déjà perçu le montant de la CVAE 2023 qui lui est dynamique, est dynamique, la ficelle est assez grossière pour ne pas fâcher les bénéficiaires ainsi lésés. La première ministre s'est certes engagé à abonder ponctuellement le nouveau Fonds Vert du montant de cette dynamique de 2023, mais il ne l'affecte pas le socle de la compensation de la CVAE cela revient donc à diminuer la somme fixée pour cette compensation, les incidences du schéma de compensation sur les indicateurs financiers des collectivités qui n'interviendrait certes qu'à compter de 2024, non pas à ce jour été évalué ni leurs conséquences, le cas échéant, corriger sur ce point à l'heure actuelle, le projet de loi de finances pour 2023, se borne à un renvoi bien trop large au pouvoir réglementaire, cela me rappelle la suppression de la taxe d'habitation ou des problèmes de compensation subsistent, notamment sur la réforme des indicateurs financiers, vous vous attaquez au sujet de la CBE alors que celui de la TH n'est pas clos. Auparavant, avec les contrats de Cahors aujourd'hui avec le nouveau pacte de confiance, vous souhaitez opéré le mouvement visant à recentraliser le fonctionnement des collectivités d'ailleurs, je note que cet article a été supprimé à l'Assemblée nationale, pourquoi a-t-il été supprimé parce qu'il était irréaliste, il établissait le plafonnement de la progression des dépenses de fonctionnement, à un niveau inférieur d'un demi-point au niveau de l'inflation des sanctions était même prévue en cas de dépassement, cela ne me semble pas acceptable, surtout que l'on ne connaît ni les critères, ni l'organisation précise de ce nouveau dispositif coercitif, Madame la Ministre votre copie est à revoir, il convient de sortir de l'ère du soupçon vis-à-vis de nos élus locaux d'autant plus qu'ils sont contraints par des règles budgétaires bien plus exigeantes que celles qui s'appliquent à l'État et au gouvernement, et Madame la Ministre, je voudrais le dire, cela se voit, tout respecter vos engagements européens, vous souhaitez faire des économies sur le dos des collectivités qui sont plus vertueuses que vous face à la hausse des coûts de l'énergie, de nombreuses collectivités même celles en bonne santé financière se voit dans l'obligation de décaler des travaux importants ou des projets d'investissement, en particulier ceux en faveur de la transition énergétique Madame la Ministre votre seul souci devrait être de permettre aux collectivités de conserver une épargne brute significative afin de couvrir des investissements nouveaux, surtout que la facture énergétique pour les collectivités est estimé à 11 milliards d'euros, selon le rapport de notre collègue, Gatel le bouclier tarifaire, ainsi que le plafonnement des prix de l'électricité à cent quatre-vingts euros le méga-watts sont certes utiles mais ne répondront que de manière insatisfaisante à l'augmentation des charges des collectivités Ces collectivités peuvent participer à l'effort de redressement de nos comptes publics, mais il doit d'abord y avoir un échange constructif avec les associations d'élus, souvenons-nous que les comptes des collectivités territoriales ne peuvent être en déséquilibre. Actuellement, les finances locales connaissent un effet ciseau du fait d'une forte progression des dépenses non compensées par une augmentation équivalente de leurs recettes, Madame la Ministre, le processus de mitage fiscal organisé méthodiquement transforme peu à peu les principaux impôts Directs locaux en compensation, puis en dotation compensation et dotations sur lesquels les élus locaux n'exerce ni pouvoir de taux ni pouvoir d'assiettes au regard du contexte actuel, l'enjeu majeur aujourd'hui est une meilleure coordination des finances locales, sociales et étatiques plutôt que laisser s'engager un retour vers un nid idéal d'État central qui ne peut et ne doit plus être merci. Merci monsieur le président, et la parole est maintenant à Madame Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Pour 100 minutes également. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues j'intervient donc au nom du rapporteur général Jean-François Husson qui ne pouvait être présent ce soir dans l'hémicycle ce débat sur la situation des finances des collectivités territoriale représente une avancée importante permise par la réforme de la LOLF et à laquelle le rapporteur général tenait particulièrement pour cadrer ce débat un 1er constat s'impose : il faut d'emblée dissiper l'illusion d'une situation financière favorable pour les collectivités territoriales, au delà de leur grande hétérogénéité raisonner à partir de moyenne globale n'a pas grand sens, quelle est donc cette réalité tout d'abord, fin 2021 près de 46 % des communes disposer d'une épargne brute encore inférieurs à leur niveau de 2019 la crise sanitaire a laissé des traces budgétaire pour de très nombreuses collectivités désormais par les conséquences de la guerre en Ukraine, une première réponse a été apportée cet été avec l'adoption en loi de finances rectificative d'un filet de sécurité pour le bloc communal et de mesures spécifiques pour les départements et les régions, ce filet de sécurité, le fruit d'un travail entre les différents groupes de l'Assemblée nationale que le Sénat a renforcé de façon significative en y incluant les charges liées au relèvement du point d'indice de la fonction publique à la hausse du prix de l'énergie mais aussi à la forte inflation sur les produits alimentaires, ce dispositif a le mérite d'exister, pour préserver les collectivités qui auront été le plus en difficulté en 2022 pour autant sa portée n'est plus adapté, en effet, la situation continue de se dégrader depuis la rentrée de nombreuses collectivités voit se dresser un mur lors du renouvellement de leur contrat de fourniture d'électricité et de gaz, et ne savent pas à ce stade, comment équilibrer leur budget pour l'année prochaine des mesures puissantes et efficaces doivent être prises dans le projet de loi de finances pour protéger les collectivités qui en ont besoin, le gouvernement doit comprendre qu'en les laissant dans cette impasse financière nous agissons contre notre propre intérêt, en effet, ce sont les collectivités qui ont la capacité de mener dans nos territoires, les projets d'investissements indispensable, en particulier ceux qui permettront de mettre en oeuvre et de réussir au plus près des besoins la transition écologique indispensable à notre pays, mais ce débat budgétaire ne doit pas se limiter aux épreuves de l'année à venir, l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027 nous donne également l'occasion de nous prononcer globalement sur la stratégie de redressement des comptes publics et en particulier sur la juste part que doivent prendre les collectivités territoriales dans cet effort, bien que leur solde soit excédentaire de près de 5 milliards d'euros en 2021 et que leur d'être présente moins de 9 pour 100 de la dette publique totale, le gouvernement fait le choix de demander aux collectivités territoriales, un effort très substantielle de baisse de leurs dépenses de fonctionnement de 0,5 pour 100 par an en volume dans le même temps, si l'on neutralise l'effet des dépenses du plan d'urgence du plan de relance et, plus globalement, les dépenses de crise, il apparaît que l'État ne réaliserait pas le moindre effort sur ses dépenses et que, même celle-ci progressé sur la période de programmation sans aucun doute notre assemblée comme les élus locaux ne saurait accepter sans réagir les méthodes d'un État qui entend réduire la dette publique, tout en continuant d'aggraver la sienne ou encore baisser les impôts en supprimant ceux des autres, la proposition de suppression de la CVAE et à cet égard une nouvelle illustration en conclusion de son propos, le rapporteur général souhaité évoquer le prétendu pacte de confiance on nous affirme que les mesures prévues n'ont rien à voir avec les contrats de Cahors, il faut donc croire que c'est par étourderie, que le gouvernement a laissé dans l'article 23 du projet de LPFP qui nous est présenté plusieurs paragraphes entièrement copier-coller depuis l'article 29 de la précédente loi de programmation qui instituer des contrats de Cahors, alors certes une première année de liberté surveillée est accordé avant la mise en oeuvre d'un mécanisme de correction extrêmement contraignant appliquée au terme d'un raisonnement par strates de collectivités pour le mois d'août, de nouvelles sanctions ont par ailleurs été imaginé avec notamment l'exclusion des dotations d'investissement de l'État, nous sommes vous le voyez bien bien loin de la nouvelle méthode qui nous avait été annoncé, les collectivités territoriales savent pourtant pertinemment qu'il existe entre elle et l'état une communauté de destin et que la réussite de notre pays passe par le redressement de ses finances publiques, elles ont consenti de très importants efforts par le passé pour maîtriser leurs dépenses et sont prêtes à continuer à le faire sous réserve de réciprocité de la part de l'État, c'est une question de justice, au-delà des mots, nous attendons donc plus que des actes, mais des actes de confiance bien sûr. merci, et la parole est maintenant à Madame Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales pour dix minutes maximum. Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission des finances, madame la vice-présidente de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est un plaisir et un honneur de prendre part avec vous à ce 1er débat consacré aux finances locales ce nouvel outil démocratique a été rendue possible par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, il constitue selon moi une avancée pour notre pays, pour nos collectivités en introduisant de manière inédite, un temps dédié aux finances locales dans le cours de l'examen des projets de loi de finances, j'ai déjà pu me livrer à cet exercice, vendredi dernier à l'Assemblée nationale, avec mon collègue Gabriel Attal et comme le veut le fonctionnement de nos institutions, c'est aujourd'hui au Sénat, chambre des territoires que j'ai l'opportunité de me livrer à nouveau dans des modalités légèrement différente, nous avons bien suivi une méthode renouvelée avec Gabriel Attal et Christophe Béchu dans l'élaboration du volet territorial de ce projet de loi de finances, conformément d'ailleurs à la volonté du président de la République et à la première ministre notre démarche a été celle d'un échange continu en amont avec les associations d'élus pour co-construire ensemble des mesures qui répondent aux besoins des territoires et aux attentes de nos concitoyens, nous les avons toutes reçu à plusieurs reprises jusqu'à la présentation du PLF au comité des finances locales, le 26 septembre quelques heures après sa présentation en conseil des ministres après le temps de la concertation, nous sommes désormais entrés dans le temps de la construction, la construction d'un d'un budget protecteur, bien sûr, mais aussi un budget qui prennent en compte l'impératif de maîtrise de nos finances publiques et la participation indispensable de chacun à cet effort, cet esprit de responsabilité et cet impératif d'actions ont été nos 2 guides dans la conception de ce projet de loi de finances pour 2023 et je le sais, ce sont les 2 principes qui animeront également votre examen. Face à la progression inédite de l'inflation et à l'envolée des coûts de l'énergie, les défis auxquels les collectivités territoriales doivent faire face, impose un soutien accru de l'État dès cet été, je voudrais rappeler que notre gouvernement a proposé des mesures fortes dans la loi de finances rectificative que vous avez d'ailleurs ici au Sénat enrichi et voté avec notamment la mise en place d'un filet de sécurité de 430 millions d'euros pour aider les communes et les intercommunalités les plus fragiles à faire face à la hausse du point d'indice à la hausse du coût de l'alimentation et de l'énergie, nous savons que certaines collectivités ont besoin de cette aide au plus vite, c'est pourquoi, comme l'a annoncé : Gabriel Attal dès la parution du décret du 13 octobre et jusqu'au 15 novembre les collectivités pourront déposer leurs demandes qui leur permettra d'obtenir un acompte de 50 pour versé avant le 15 décembre nous avons par ailleurs louer 120 millions d'euros aux départements qui versent le revenu de solidarité active pour compenser intégralement la hausse de 4 % de cette prestation prévue par l'État et nous avons instauré le recouvrement total par l'état auprès des régions de la hausse de 4 % des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Cet accompagnement de l'État est encore accentuée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 avec d'abord un amendement du rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale de prolongation du filet de sécurité pour les dépenses énergétiques de 2023 avec aussi la prolongation du bouclier tarifaire, une mesure qui permettra de limiter à 15 % la hausse des prix de l'électricité pour 80 % des communes. et j'ajouterai le quintuplement de l'enveloppe à destination des communes en grande difficulté qui atteint lui 10 millions d'euros, et puis surtout le non-plafonnement des bases fiscales afin de laisser toute l'autonomie aux collectivités sur leur dynamique fiscale, ces mesures permettront aux collectivités de faire face au surcoût financier dans l'immédiat, mais il nous faudra agir aussi à d'autres échelles à l'échelle européenne, d'abord en cherchant au niveau du marché européen de l'énergie à réguler les prix et à capter les super profits engendrés chez les grands groupes énergétiques par cette situation de tension. Et aussi, chacun à notre échelle, en suivant les recommandations formulées par la première ministre dans le plan de sobriété mais résoudre durablement la crise que nous connaissons impose aussi d'opérer des changements profonds de notre modèle, en favorisant la transition écologique et la transition énergétique dans tous les territoires. C'est pourquoi le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d'augmenter d'un tiers les moyens consacrés à la dotation biodiversité pour 2023 qui avait déjà été doublés en 2022 pour atteindre un montant de 30 millions d'euros et puis de mettre en oeuvre un fond Vert, d'un montant inédit de près de 2 milliards d'euros pour la méthode d'attribution de ce fonds, le financement se fera selon des règles simples décentralisé et sans appel à projets tout partira des initiatives des élus selon une méthode lisible et reconnu celle du dialogue entre les élus et leur préfet de département ou de région la première ministre a par ailleurs eu l'occasion d'annoncer vendredi dernier que 200 millions d'euros seront spécifiquement alloués au département, accompagner les collectivités territoriales, c'est avant tout leur donner les moyens d'agir en sécurisant leurs financement pour leur donner de la visibilité sur le long terme ainsi avec la première ministre et nous avons souhaité porter une hausse de la DGF, d'un montant de 320 millions d'euros de la DSU et de la DSR qui serait financé par l'État et non par écrêtement des autres communes, cette augmentation est inédite depuis 3 13 ans et je considère que c'est un acte fort du gouvernement, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises quant à elle, permettra à notre pays de gagner en compétitivité, sans amoindrir les ressources des collectivités, elle sera en effet intégralement compensée et territorialisées par l'attribution d'une part supplémentaire de TVA, mais aussi de sa dynamique dès 2023 la compensation l'année prochaine, correspondra aux sommes que l'État aurait dû reverser aux collectivités en 2000 23 au titre de la CVAE il n'y aura pas d'année blanche, rien ne sera conservée par l'État, j'ai dit-elle qu'elle serait territorialisée ceux qui accueillent davantage d'activités seront davantage compenser sur la base de critères précisés dans un décret en Conseil d'État, un travail et d'ailleurs en cours à ce sujet avec les associations d'élus et ce sujet comme sur les autres, l'écoute et la concertation devront primer notre souci de protéger les marges de manoeuvre des collectivités transparaît enfin dans le maintien de leur dotation d'investissement à un montant de près de 2 milliards d'euros, comme l'année précédente, mesdames et messieurs les sénateurs, voici les principaux éléments des concours de l'État aux collectivités en 2023 devant les défis qui sont les nôtres, notre pays, nos collectivités ne manque pas d'atouts, et nous avons toujours su construire au cours de notre histoire, dans ces situations de crise des consensus responsable au service de l'intérêt général, je sais que ce sera une nouvelle fois le cas car au-delà du débat démocratique indispensable, nous espérons que les postures et les effets de manche, qui ne font plus illusion aux c'est n'auront pas lieu il ne satisferont pas d'une nouvelle représentation du sempiternellement rejouer du combat entre les montagnards et les Girondins, c'est collectivement que les Français nous jugeront sur notre bilan, nos réussites et notre capacité à améliorer comprennent concrètement leur qualité de vie, merci pour votre attention. Merci madame la ministre, dans la suite du débat donc la parole est maintenant à Hervé Maurey pour l'Union centriste pour quatre minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après le quinquennat de François Hollande, caractérisée par une baisse drastique des dotations à hauteur de 11 milliards d'euros, Emmanuel Macron, lors de son accession à la présidence de la République en 2017, a voulu donner des assurances aux collectivités locales en matière financière, ainsi, l'annonce d'une stabilisation du niveau de la dotation globale de fonctionnement a été accueillie favorablement malheureusement la désillusion fut rapide car dès l'été qui a suivi la nomination du gouvernement en 2017, celui-ci a pris un certain nombre de décisions dont je rappelle les les principales : la réduction de 300 millions d'euros de crédits dédiés aux collectivités locales, la suppression de la réserve parlementaire et la quasi-suppression des emplois aidés, quant à la DGF si son montant a bien été stabilisée globalement la réalité de chaque commune et tout autre puisque pour la moitié des communes de France, la, la, les dotations ont en fait diminué au cours des 5 dernières années, les collectivités locales ont également vu leurs leviers fiscaux considérablement réduit par les réformes fiscales qui se poursuivent aujourd'hui au détriment de leur autonomie financière, dans le même temps, les collectivités locales ont eu à faire face à de choc sans précédent, celui de la crise sanitaire et celui de l'inflation, le choc de la crise sanitaire a coûté 7 milliards d'euros aux collectivités, dont 3 2 milliards au bloc communal sur les 3 4 milliards de pertes de recettes, le bloc communal ne s'est vu qu'on pensait qu'à hauteur de 270 millions d'euros, les pertes de recettes fiscales et domanial et de 250 millions d'euros au titre du dispositif d'aide aux Speak et au SPA à présent c'est au choc de l'inflation, que les collectivités locales doivent faire face, je rappellerai, Madame la Ministre, que j'ai attiré l'attention du gouvernement dès le mois de février sur les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie, à l'époque, sans aucune écoute de la part du gouvernement, le gouvernement a renforcé ce choc en juillet en augmentant le point d'indice pour un surcoût de 2,3 milliards d'euros, le gouvernement n'avait pas jugé utile contrairement à ce que j'ai cru entendre de notre part de prévoir un dispositif de compensation pour les collectivités, c'est l'Assemblée nationale qui a introduit un filet de sécurité extrêmement limitées que nous avons, au Sénat, considérablement améliorée notamment aux apports grâce aux apports du groupe de l'Union centriste au quel genre d'appartenir. Ce filet de sécurité reste toutefois très limités, il devrait en effet bénéficier seulement à 5 à 8000 communes ou groupements et en 2023 seulement, alors que c'est aujourd'hui que l'ensemble des communes on va faire face à ces surcoûts ce dispositif pour ce question et je souhaiterais que ce débat puisse nous éclairer sur le système d'avance prévu quelles communes vont en bénéficier, quand et comment vous avez évoqué tout à l'heure, la nécessité de déposer un dossier, mais la plupart des communes ne savent même pas si elles peuvent prétendre à ce filet de sécurité, donc je crois qu'il y a vraiment besoin de de clarification et nous serions très très heureux de vous entendre sur ce point, concernant le projet de loi de finances pour 2023, dont nous reparlerons, à notre grande surprise, celui, celui-ci ne prévoyait pas, dans sa version déposée à l'Assemblée nationale de prolonger ce filet de de sécurité l'augmentation de 320 millions annoncés par la première ministre est présentée comme une première depuis 13 ans, je cite, représente en réalité une revalorisation une revalorisation de 1,2 pour 100 du montant total de la DGF quand l'inflation est de plus de 5 nous sommes bien loin de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, demandée par les associations d'élus, vous l'aurez compris madame la Ministre, les élus et plus particulièrement les mères sont inquiets des perspectives financières pour leur collectivité j'ajouterai que, en plus, dans le contexte de transfert de la taxe d'aménagement à l'intercommunalité, il y a des situations qui sont particulièrement compliquée, je rappelle que ce dispositif a été voté par l'Assemblée nationale, sans aucune concertation et il faudra que l'on en reparle lors de l'examen du projet de loi de finances que vous appeler à revoir la copie du projet du prochain projet Michel Oleg pour permettre aux collectivités de faire face à cette période particulièrement difficile. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Stéphane Ravier des sénateurs non inscrits. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a-t-il encore une décentralisation dans notre pays, la question mérite d'être posée, car si l'on décentralise les compétences, la fiscalité, elle reste jacobine, ce gouvernement fait preuve de la démo de démagogie démagogie fiscale sur le dos des collectivités territoriales, on a osé parler de suppression de la taxe d'habitation, mais rien n'est supprimé pour le contribuable, les propriétaires supporte la hausse de la taxe foncière et les locataires, la hausse des loyers qui en découlent, avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les communes finissent de père de toute autonomie fiscale peu de ressources propres et plus de ressources réellement dynamique prison pillage, elles sont contraintes de racketter les propriétaires en augmentant la taxe foncière avec la hausse des prix de l'énergie à plus de 250 % la flambée des matières premières de la restauration scolaire et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les communes n'ont plus de marge de manoeuvre en ce moment, les maires et leurs adjoints aux finances sont dans la préparation de leur budget pour 2023 il s'arrachent les cheveux, ils font face à une explosion de leur budget de fonctionnement, pourtant cela fait depuis le printemps dernier, que je demande au gouvernement un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie pour les collectivités, très cet été, on a eu droit en pleine canicule, à la fermeture de piscine, comme dans les Bouches-du-Rhône à Cabriès et cet hiver, on risque la suppression des décorations et fêtes de Noël et pendant ce temps, l'État obèse refuse de descendre de notre de notre dos et de sortir ses mains de nos poches, la crise qui s'installe montre encore l'inefficacité de l'État et la pertinence de la gestion locale, mais le gouvernement ne veut rien entendre l'État répond par des soins palliatifs à l'asphyxie des collectivités locales et des aides et des hausses de dotation, mais plus de ressources propres et comme il ne reste tributaire du bon vouloir de Bercy et en sont réduites à faire la manche, la Banque Postale et prévoit une baisse de 11,3 % de leur épargne brute cette année en 2023, il ne faudra que quelques mois pour que les communes est épuisé la totalité de leur budget de fonctionnement sans changement, nous allons vers un fiscale communale, la Cour des comptes dans son rapport de la semaine dernière, propose que les droits de mutation à titre onéreux soit recentrés sur le bloc communal, voilà une proposition qui permettrait aux communes de retrouver une ressource dynamique, dynamique, ce serait un juste retour de leur investissement constant pour l'attractivité du territoire qui leur permettraient notamment de financer leurs dépenses de fonctionnement décentralisé, la fiscalité, c'est garantir le principe constitutionnel de consentement à l'impôt de nos concitoyens, quiconque a les pieds dans le réel, comprendra que c'est un enjeu majeur rendre communes leur autonomie fiscale, c'est à ça et à rien d'autre que nous devons travailler mes chers collègues. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE pour cinq minutes.

c'était un peu mieux, a salué la tenue ce débat instauré par la loi organique de modernisation de la question vient c'est public adoptée à la fin de l'année dernière, c'est une nouvelle loi organique contribuer la difficile tâche de moderniser le cadre des lois défiance certains avaient envisagé l'instauration d'une loi spécifique pour au cas essence de la loi sur le financement de la Sécurité sociale, nous, on se contente aujourd'hui d'un débat, mais les enjeux politiques de différents des finances locales, conjugué à une technicité de plus en plus complexes, ça nous inévitable à terme la discussion d'un texte budgétaire spécifique, le dernier rapport, la Cour des comptes, de sa situation ne vient sur le coeur est éclairant, en particulier dans les comparaisons internationales, les finances locales ne représente en France que 20 % de la dépense publique, un niveau inférieur à la moyenne européenne, on le dit pense les dépenses des collectivités locales représentent plutôt 40 de ses dépenses publiques avec des modèles étatiques et des périmètres de compétence certes différent néanmoins cela remet en perspective le débat où les collectivités se voit toujours reprocher un manque de rigueur budgétaire, alors quelles sont les seuls à présenter cette année soldat l'équilibre si les collectivités représente donc un 5ème de la dépense publique, elles ont une contribution de quasi nul au déficit public au-delà de ces considérations dans le général, la situation financière des collectivités est évidemment très diverses global avoir avoir paradoxalement les collectivités sont sortis directives sanitaires avec des finances plus saines qu'avant la crise, grâce aux économies qui ont été réalisés et gel accordée par le gouvernement, toutefois, cela cache des situations lundi duel très contrastée, j'ai concentré mon propos sur les fiancés communal et les départements, le bloc communal a été le plus affecté par les dernières réformes de la fiscalité, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences vous principal et bientôt suppression complète de la CVAE si tire encore aujourd'hui les 2 tiers de ses ressources de la fiscalité locale, même si c'est le site en être remplacé par un transfert d'impôts nationaux, la question qui se pose aujourd'hui est bien sûr celle de l'autonomie financière, alors que la différenciation territoriale devient un enjeu politique majeur, c'était question concerne aussi les départements davantage financés par les impôts nationaux et les dotations, ils font face à une montée en puissance de leurs interventions dans le domaine social, je pense à particulier aux départements ruraux souvent déprise démographique accompagner le vieillissement de la population avec des ressources fiscales propres assez peu dynamique, bien sûr, la solidarité nationale doit jouer grâce au transfert d'impôts l'impôt nationaux mais là aussi, se pose la question de la soutenabilité de modèles de décentralisation ou on accepte de différencier, voire de donner à terme vous réglementer adaptation mais ça ne donnait une véritable autonomie financière correspondant à l'autonomie de décision bien sûr face retour un sur le gouvernement a pris en loi de finances rectificative des mesures qui ont aidé les collectivités à faire face et qui te salue alors qu'il a reçu un terrain de 432 millions d'euros visant à compenser la hausse des prix énergétiques et la revalorisation du point d'Annie, des fonctionnaires, néanmoins je ne pas l'inquiétude des élus pour 2023, qui souhaite que ce soutien, elle soit pérennisé en loi de finances, les amendements adoptés en commission la semaine nationale la semaine dernière, semble le confirmer, ce dont je me réjouis mon groupe soutiendra dans tous les cas, les mesures visant à donner aux collectivités les moyens correspondant à leur mission, dont on sait qu'elles sont indispensables à notre cohésion sociale, quoi qu'il a joint la principale mesure du projet de loi de finances pour 2023 et bien évidemment la suppression en 2 ans de la pointe par un stade de la CVAE cette compensation pour le versement d'une fraction de TVA est allongée à l'alors près pérenne et dynamique, nous vous prenons au mot la ministre ils veilleront, dans l'État, s'agissant par ailleurs de de l'État, le gouvernement poursuit sa politique du précédent quinquennat marqué par une grande stabilité la DGF reste de 26 à 27 milliards d'euros malgré l'inflation, les montant des dotations de péréquation pour la dissuader seront revalorisées dans le même montant que les années précédentes à l'état actuel des débats sur le 1er, loi de finances, il reste toutefois difficile d'entrevoir l'architecture financière qui sortira pour les collectivités, dans l'attente de la mise en oeuvre de l'article 49 3 dont on parle beaucoup et l'incertitude demeure, comme l'illustrent les déboires chaotiques autour du projet de loi de finance de programmation 2023 2000 27 au vu du contexte économique et sociale que traverse notre pays, les collectivités territoriales, comme tous nos concitoyens homogène de clarté de prévisibilité et de sérieux. Merci au président Riquier et la parole est maintenant président Karoutchi pour le groupe Les Républicains pour ça. Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le débat essentiel, c'est de se demander si nous respectons depuis un certain temps la constitution. Dans les articles 72 à 74 on nous explique longuement ce qu'est l'autonomie des collectivités en quoi est-ce que l'autonomie des collectivités, vous n'y êtes pour rien Madame la Ministre et respecté quand on supprime progressivement la taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la CVAE lorsqu'on met en place un encadrement d'état, alors ça s'appelle un coup les accordent le de Cahors du mais le pacte de confiance et puis plein de pacte plein de pacte mais une seule réalité les élus locaux perdent le pouvoir, les élus locaux perdent la capacité d'agir sur leur territoire parce qu'ils perdent la capacité de financer, alors vous allez me dire et vous l'avez dit vous-même, Madame la Ministre, on compense oui mais c'est pas la même chose. chose. Centralisé recentraliser l'impôt pour ensuite faire en sorte que les collectivités dépendent de dotations d'État, qui ne sont assez rarement remise en en en au niveau de l'inflation, ça n'est pas la même chose, ça revient à dire qu'en réalité la gestion des élus locaux et si peu fiable qu'il faut la recentraliser et que c'est l'État et son administration d'état qui par définition est bien plus doué que les élus locaux qui doit gérer le tout, alors il y a un vrai problème, moi je me souviens très bien, ici même, de Jean Marc Ayrault Premier Ministre qui, fin 2012 nous avez dit l'année prochaine nous remettrons à plat l'ensemble de la fiscalité nationale et locale et nous allons enfin trouver un équilibre, inutile de dire que nous n'avons jamais eu cette table ronde jamais cette remise à plat et que les gouvernements quels qu'ils soient, hein, depuis 20 ans continue très progressivement de rogner le pouvoir des élus locaux, les maires aujourd'hui sont à la fois étranglé sont responsables devant la population et non plus la capacité de leurs responsabilités et c'est ça le vrai problème, vous ne pouvez pas et Madame le Ministre, vous étiez maire de Beauvais il y a encore peu, et vous savez très bien que lorsque pendant le mandat de Hollande on réduisait les dotations lorsque ici ou là, on nous a dit : suppression de la taxe d'habitation, sans forcément de de négociation, hé bien il y a une perte de pouvoir des élus locaux, il y a une perte de capacité d'action, il y a une perte de réalité du lien entre la population, les collectivités locales et leurs élus, je viens de voir je j'espère que ça ne va pas prospérer que même sur la taxe foncière, un amendement a été voté à la commission des finances de l'Assemblée nationale pour fixer un maximum de hausse de la taxe foncière en disant que, au de là, hé bien l'État compenserait même sur la taxe foncière alors bientôt il y aura plus aucune ressource des collectivités locales et nous, on attendra que l'État veuille bien donner un minimum pour survivre, ça n'est pas ça l'autonomie et je vous rappelle que la Cour des comptes dit elle-même qu'effectivement au fur et à mesure des années, l'autonomie des collectivités locales et remise en cause, je regrette que la Cour des comptes n'aille pas plus loin en demandant clairement à l'état de cesser cette ce mouvement, ce mouvement qui dure depuis 20 ans, qui consiste à faire en sorte que les collectivités locales soient de plus en plus dépendantes de l'État et de moins en moins dépendantes de leurs projets locaux de leur population de la volonté de leurs élus, alors tout ça et dans un contexte totalement fou parce que, effectivement, avec les crises, on l'a dit Chris sanitaire la la crise énergétique, tout le monde essaye de trouver des solutions et nos collectivités vont clairement trinquer, il faut dire les choses, s'il y a pas de bouclier énergétique sur les collectivités s'il y a pas une capacité à trouver une solution vraiment acceptable sur la CVAE si il n'y a pas de capacité à dire à toutes les collectivités pas, vous l'avez dit, Madame la Ministre, vous dites 80 % des communes seront concernées et les 20 % autres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas totalement une capacité à dire on va faire en sorte que les collectivités locales puissent exister que les élus locaux, retrouvent leur pouvoir, parce qu'ils sont responsables et ils sont élus par leurs populations, ils sont responsables devant des gens qui leur disent : vous ne faites pas si vous ne faites pas ça, ils vont peut-être être amenées à supprimer des services publics locaux et tout ça en leur disant : vous êtes responsables électoralement devant vos électeurs mais vous n'avez pas la capacité financière d'agir, et ça c'est une profonde anomalie alors je partage le dit comme ça, je resterai dans mon temps limité la proposition d'Éric Berdoati qui l'a fait : ah ah, devant l'Association des maires d'Île-de-France, pourquoi pas, mes chers collègues envisagées il y a le PLF il y a le PLFSS hé bien faisons MPL FCL un PLF des collectivités locales, ça donnerait de la visibilité à ce qu'on fait au niveau des finances locales et ça nous remettrait peut être à l'équilibre avec l'État pour négocier les capacités financières et l'autonomie de nos collectivités merci. Merci, cher collègue, et la parole est maintenant à Emmanuel Capus pour les indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ont dit le Sénat conservateur mais et les des changements que nous accueillons bien volontiers l'organisation d'un débat sur les finances locales en amont du budget, c'est en effet une nouveauté qui a tout pour nous plaire. La réforme de la loi organique des lois de finances il y a un an, en a fait un jalon du début du débat budgétaire, c'est une première, c'est l'opportunité pour nous, avant de rentrer dans le dur des discussions de faire le point sur la situation des collectivités, le rapport de la Cour des comptes sur le sujet, présenté en commission la semaine dernière à poser un diagnostic clair et ouvert des pistes de réforme dont chacun peut s'emparer l'autre particularité de ce débat, c'est qu'il intervient en début de quinquennat et donc au début d'une nouvelle séquence politique nos discussions ne peuvent, à cet égard, faire l'impasse sur le programme du président de la République qui a été réélu, le président de la République s'est engagé à poursuivre le chemin tracé depuis la crise sanitaire et le plan de relance en baissant les impôts de production, notamment la CVAE ce n'est pas spontanément le souhait le plus partagé parmi les élus locaux que nous sommes. Nous aurons tout loisir pendant l'examen du PLF 2 débattent des modalités techniques et du les calendrier de mise en oeuvre de cette suppression, mais ce débat est l'occasion de prendre un peu de hauteur et de discuter des grandes orientations que nous souhaitons donner à la réforme de la fiscalité locale, je rappellerai donc d'abord pourquoi nous sommes favorables par principe à la réduction des impôts de production. En 2020 avant la baisse de la CVAE ses impôts représentaient plus de 5,3 % du PIB en France contre 2 6 % dans l'Union européenne et seulement 0,8 pour 100 en Allemagne 0 or ces impôts sont injustes pour les entreprises, parce qu'elle ne pèse pas sur les bénéfices, mais sur les facteurs de production, ils sont surtout contreproductif, car ils pénalisent tout particulièrement les entreprises industrielles, des territoires, la suppression de ses impôts et donc une bonne nouvelle pour notre industrie et indirectement pour nos territoires, si cela n'affectait pas les finances des collectivités locales, je crois que le Sénat ne pourrait que s'en réjouir mais c'est notre rôle de nous assurer que cette suppression sera aussi une bonne nouvelle pour les collectivités, or, en l'espèce, je partage certaines des craintes qui ont été exprimées ici en réalité n'est pas la suppression de cet impôt, mais bien son remplacement et ça territorialisation, vous l'avez rappelé : Madame la Ministre, l'affectation d'une fraction de TVA donne certes aux collectivités des ressources fiscales dynamique, elle est de nature à rassurer mais d'un autre côté, cela a été rappelé, elle les prive d'un levier de politique économique, cette nouvelle dépossession engagée après la suppression de la taxe d'habitation contribue à placer davantage les collectivités sous la coupe de l'État. Elle est mal vécu, vous le savez, pour être élu local, Madame la Ministre, même si la territorialisation que vous avez annoncé. Permet de rassurer la préservation de l'autonomie financière des collectivités qui a été rappelé par notre collègue Karoutchi ne doit pas se faire aux dépens de leur autonomie fiscale déjà réduite à peau de chagrin, je sais, Madame la Ministre, que vous partagez cet objectif de préservation de notre autonomie financière avec le ministre, Christophe Béchu, d'autant que les collectivités ont ont fait preuve de leur capacité à tenir les comptes Christine Lavarde l'a rappelé tout à l'heure à fin 2021 elle dégageait 5 milliards d'euros d'excédents budgétaires en raison des circonstances mais aussi parce qu'elles savent être extrêmement prudente, pourtant depuis ce moment depuis cet excédent la reprise en sortie de crise sanitaire et les tensions en Ukraine ont tiré les coups de fonctionnement à la hausse aujourd'hui les élus locaux font face à des augmentations qui les place, dos au mur, dans son rapport, la Cour des comptes propose plusieurs pistes de réformes afin de remettre à plat le financement des collectivités, l'une de ces pistes consiste notamment à partager la fiscalité nationale c'est une pièce qui a la main le mérite de garantir aux collectivités des ressources dynamiques qui suivent les cours de l'inflation, la Cour propose aussi d'attribuer un type d'impôts par strates de collectivités cette piste, a le mérite aussi de clarifier les choses, mais elle ne répond pas aux préoccupations des collectivités, l'urgence n'est pas de remettre à plat la fiscalité, l'urgence c'est de sauvegarder l'autonomie financière des collectivités, elles doivent garder la maîtrise de leur destin et de leur politique, particulièrement dans les crises comme celle de l'énergie que nous traversons, madame la Ministre, puisque nous sommes dans un débat, pouvez-vous nous rassurer à ce sujet, il en va de la préservation des services publics de proximité, nos élus locaux sont naturellement inquiets et ils attendent des engagements forts du gouvernement, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Daniel Breuiller pour le groupe écologiste solidarité territoire Monsieur le président. Madame et monsieur le la vice-présidente, Madame la Ministre, chers collègues, les précédents orateurs ont cité tous les chiffres, je voudrais, pour ma part, démarrer mon propos avec Pablo Neruda, je t'aime, d'une manière inexplicable de nature inavouable de façon contradictoire, je t'aime avec mes états d'âme, qui sont nombreux et mais changement d'humeur continuelle, c'est une déclaration d'amour magnifique et ce sont les mots que nous aurions aimé entendre de la part de l'État à l'endroit des collectivités territoriales, alors oui, c'est une vieille histoire entre l'État et des collectivités locales, une histoire constitutionnelle marquée par 19183 et les lois de décentralisation, et depuis, elles sont là, elles font preuve d'efficacité bouclier de proximité, acteur essentiel de l'investissement public de l'emploi des solidarités, votre gouvernement ne cesse de déclarer sa flamme et son soutien aux plus grandes entreprises, accordant des dizaines de milliards sans contrepartie ni écologique ni sociale, la situation de Total en est l'illustration ultime et caricatural, je vous rappelle que Total comme les 5 plus grandes entreprises fossiles réalise un profit cumulé de 2600 dollars par seconde, Madame la Ministre, les collectivités territoriales sont des entreprises de service public innovantes qui méritent soutien liberté d'action et confiance qui pendant la pandémie à organiser les distributions de masques de colis alimentaires, l'accueil et la désinfection des salles de classe pour les enfants, les profs des professions prioritaires, le suivi des personnes âgées isolées au malades qui a mis en place des centres de vaccination pour répondre aux enjeux de santé publique, que le président Macron annonçait qui a rétabli le dialogue durant la crise des gilets jaunes qui investit dans les transports collectifs, la transition énergétique et écologique qui permet que tiennent les solidarités locales, les collectivités locales sont un atout puissant et vous les mettez au pain sec quand le budget 2021 a offert 56 milliards aux entreprises du CAC 40 non conditionnée et largement redistribué en dividendes au nom de quoi l'État dont les déficits s'aggrave, veut-il contraint des choix politiques des collectivités dont la gestion est équilibrée, elle contribue à 70 % des investissements publics et par leur budget de fonctionnement, elle contribue à la cohésion sociale, car le fonctionnement n'est pas un gros mot, c'est l'outil nécessaire des services à la population. Les collectivités locales sont le laboratoire de politique publique innovantes et des transitions pour notre pays, transports propres bâtiments économes en énergie renaturation des villes, développement des énergies renouvelables, protection des forêts des littoraux de la biodiversité sont au coeur des dynamiques porté par nos territoires, la diversité de leur politique permet des expériences fructueuses si vous leur donniez la confiance mais sans le contrat Madame la Ministre, vous verriez les capacités à accompagner les défis de notre société en termes sociaux et écologiques, vous mettez en place un bouclier tarifaire pour tous les citoyens, même les plus riches d'entre nous, pour les entreprises et rien pour permettre aux collectivités de continuer à chauffer les écoles, les collèges, les lycées, les équipements sportifs, les médiathèques ou les théâtres, les centres de santé ou les crèches rien d'ailleurs pour les hôpitaux, non plus, autre sujet essentiel l'échelle moduler le versement mobilité pour faire face aux enjeux du transport en commun, laissez les taxer plus Serbie Hanegbi les résidences secondaires, les logements vacants, les hôtels de luxe, pour faire face à la crise du logement en zone touristique, la Cour des comptes a fait des propositions, suite à la saisie le notre excellente commission des finances, les associations d'élus portent haut et fort une contribution responsable et le parlement dans notre chambre, comme à l'Assemblée nationale, vous invite à nous entendre, pas seulement à nous écouter, mais bien à nous entendre, entendez nous entend délai ne supprimez pas la CVAE indexer la DGF taxer ceux qui font des profits exceptionnels dans ce contexte de crise et financer ainsi un bouclier tarifaire pour toutes les institutions publiques, supprimer les contrats mais faites, faites confiance à celles et ceux qui au quotidien sont au service de nos concitoyens et incarne le service public de proximité, c'est, c'est le désarmement financier de l'État et des collectivités et osez, osez la confiance aux équité ce jacobinisme surplombant pour un vrai partenariat avec les collectivités locales, oser la République décentralisée, les élus territoriaux ne veulent pas devenir des sous-préfets anémiée, qui savent ce qu'il faudrait pour leur territoire mais ne sont sont tout juste bons à expliquer à leurs concitoyens qui ne peuvent pas le faire. La parole est maintenant à Didier Rambaud du groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre président Claude Raynal, qui a demandé en janvier dernier à la Cour des comptes, une enquête sur les finances locales, les conclusions nous ont été présentés la semaine dernière et elle nous permettent de prendre un peu de hauteur dans ce débat, car derrière ce débat, nous touchons aux principes les plus structurant de l'organisation de notre République depuis la réforme constitutionnelle de 2003 les collectivités territoriales ont pris une place prépondérante prépondérante dans cette organisation, notre constitution reconnaît désormais la décentralisation comme l'un de ses principes fondateurs et consacre le caractère prioritaire de leur action et le principe de subsidiarité, c'est ainsi que la question de leur financement devient fondamental pour l'efficacité de l'action publique pour l'égalité entre les territoires et entre les citoyens, au fond, ne pouvons pas dissocier la question du financement de celles des compétences, le 1er président de la Cour des comptes a rappelé la semaine dernière que le système de financement des collectivités est à bout de souffle qu'il était illisible, imprévisible pour les responsables locaux pour les contribuables avec des inégalités qui se creusent entre certains territoires et ce n'est pas un fait nouveau, il y a 13 ans la Cour dresser le bilan des réformes territoriales et l'enchevêtre ment des compétences qu'elle relevé alors préfigure la sédimentation budgétaire que nous constatons aujourd'hui et l'essoufflement d'un modèle de financement, l'introduction de la clause de compétence générale a conduit à accélérer ce processus avec des transferts qui se sont opérés de façon désordonnée et Parakou la cacophonie budgétaire est souvent la conséquence des hésitations et ou des tergiversations du législateur et des changements de doctrine de l'administration, on finance par prélèvement sur les recettes de l'État, l'affectation d'une nouvelle compétence puis on prévoit une rétro compensation quelques années plus tard, qui ont la compétence se retrouve affecté ailleurs à la fin, plus personne ne s'y retrouve, il y a 13 ans, la Cour des comptes, rappeler que la nouvelle phase de décentralisation lancée en 2003, aurait pu être l'occasion d'un nouveau départ, l'échec était flagrant aux yeux des sages et les gouvernements de droite comme de gauche, qui se sont succédé ont échoué, 13 ans plus tard le constat sur les finances locales rejoint celui posé sur les compétences, alors si nous voulons débattre de ce sujet, il nous faut nous mettre d'accord sur le constat, je me contenterai de rappeler les éléments présentés la semaine dernière par la cour, les collectivités locales ont connu un excédent de 4 7 milliards d'euros fin 2021 en raison d'une dynamique des recettes très supérieure à celle des des dépenses, c'est une situation qui compte contraste très nettement avec la situation des autres administrations publiques et la crise sanitaire à renforcer, renforcer cet écart en 2021 est l'État porte la quasi-totalité du déficit à 89 %, alors que les collectivités locales sont en excédent, c'est la conséquence d'un fort soutien de l'État, tout au long de la crise, mais également des réformes successives de la fiscalité locale, compensée par des ressources pérennes et dynamiques, mais ne nous y trompons pas, derrière cette question, nous sommes face à un véritable choix de doctrine qui devra s'imposer dans les années qui viennent et les scénarios de la Cour permettent permettent d'en peser les conséquences la liberté qui va avec le levier de fiscalité locale s'accompagne nécessairement d'un recul de l'État dans son rôle de garant de la stabilité des ressources des collectivités, nous devrons donc faire des choix, Philippe Séguin, alors président, 1er président de la Cour des comptes, affirmait déjà, je cite, considérer qu'il les 3 acteurs autonomes de même niveau, l'État à la sécurité sociale et les collectivités locales n'est pas réaliste, en réalité, l'État est le seul maître du jeu car précisément, il fixe les règles du jeu, les finances publiques sont un tout et l'État portent la responsabilité pleine et entière de leur évolution, pour nous, parlementaires, élus locaux et citoyens, cela veut dire 3 choses : la première c'est que dans un contexte de contraintes fortes sous nos finances publiques, chacun doit prendre sa part du rétablissement des comptes de la nation et toute réforme des finances locales, devra prendre en compte ce juste équilibre entre l'État et les collectivités locales dans la réduction du déficit, élus de nos territoires, nous devons jamais oublier la responsabilité collective qui nous incombe vis-à-vis des finances de la nation, la seconde et c'est, et c'est ce qu'a affirmé le 1er président toute réforme d'ampleur devra se faire en concertation avec les élus, cela nous oblige à laisser de côté nos querelles du moment pour discuter avec responsabilité du juste niveau d'organisation et de l'adéquation des ressources au besoin, là encore, le rapport de 2009 et sans appel sur les échecs du passé pour atteindre une véritable péréquation, il aurait fallu accepter de remettre en cause certaines situations acquises, mais cela n'a pas été fait et je cite le 1er président à l'époque, l'objectif de péréquation est resté secondaire dans ce contexte est tributaire des erreurs du passé, ce PLF 2023 apporte la seule réponse possible, sans recours à une à une réforme radicale, de l'augmentation de la DGF pour compenser les variations à la baisse qu'aurait pu entraîner la péréquation, il s'agissait de trouver la la solution la plus équilibrée pour compenser les variations annuelles et préserver nos collectivités sans peser lourdement sur nos finances publiques, la 3ème enfin c'est d'accepter de revoir en profondeur le système de péréquation pour mettre fin aux inégalités de destin et rétablir l'égalité entre les territoires, je cite à nouveau le premier le président à sa présentation de 2009, la République, c'est la solidarité nationale et il ne faudrait pas que la décentralisation devienne l'alibi de son affaiblissement, la France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé, pour ce faire elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire la question qui doit dès lors nous occuper et celle de l'équilibre entre le principe d'autonomie financière, consacré au plan constitutionnel l'équité et la cohésion entre les territoires et la responsabilité de chacun vis-à-vis de nos finances publiques. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Isabelle briquet pour le groupe socialiste, écologie. Il a public. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les finances locales sont-elles devenues les variables d'ajustement des comptes publics de contrat de Cahors, un pacte de confiance l'autonomie financière et la libre administration des collectivités territoriales deux seront bientôt plus que de lointains souvenirs. Madame la Ministre comprenait l'inquiétude des élus locaux qui, de crise en crise doivent toujours faire plus avec moins, du fait des incessantes modifications de ressources que vous leur imposez, suppression de la taxe d'habitation sous le précédent quinquennat : suppression de la CVAE sous celui-ci, et cetera transformer ainsi des recettes fiscales en dotation pose problème à plusieurs niveaux, c'est une perte d'autonomie effective, c'est couper le lien avec le territoire. Et les habitants et c'est acté, de fait, une demi, une diminution des recettes. L'inquiétude se transforme en colère lorsque ces mêmes élus entendent ici et là que les finances locales se porte bien. C'est d'ailleurs ce que m'avait répondu le ministre des Comptes publics lorsque je l'avais alerté sur ce sujet en mars dernier, il est vrai qu'il était alors question d'une ponction de 10 milliards d'euros sur les finances locales. Depuis, avec l'augmentation du point d'indice augmentation nécessaire, la hausse du coût des matières premières des denrées alimentaires et de l'énergie, les collectivités locales sont au bord de l'asphyxie, enfin celles qui peuvent encore espérer, prenons l'exemple d'une commune que je connais bien pour l'avoir administré pendant 20 ans, comment peut-elle faire face à une augmentation d'un 1000000 d'euros d'électricité alors que son budget de fonctionnement dépasse à peine les 5 millions d'euros, beaucoup d'autres communes, petites ou grandes rurales comme urbaines doit faire face à la même situation, il en est de même pour les départements dont les finances sont déjà par le manque de compensation des dépenses liées au Ségur et aux hommes et aux allocations individuelles de solidarité particulièrement le RSA pour lequel le fonds d'urgence ne fera pas la maille ou de la même de leurs dépenses propres, les collectivités doivent aussi faire face aux difficultés des organismes ou établissements qu'elle finance la situation des Epad est particulièrement préoccupante et que dire de celle des SDIS, nous voyons bien cette crise financière, a des répercussions sur l'ensemble des services publics devant l'explosion des coûts, nous avons voté cet été un filet de sécurité si, initialement il était censé concerner 22000 communes, seul un tiers d'entre elles y seraient éligibles, il est donc urgent de revoir la copie, notamment les critères d'accès afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle, la réponse du gouvernement doit être à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui que nous proposez-vous les pactes de confiance, quelle que soit la manière dont on les nomme ces pactes constitue une double peine pour les collectivités, baisse des dotations du fait de la non-indexation sur l'inflation d'une part et contrôle de la dépense, d'autre part. Il s'agit purement et simplement d'un contrat léonin, au-delà de toute autre considération, comment imposer une réduction des dépenses à des collectivités, qui ne peuvent, en raison de l'inflation, a estimé leur coût pour la seule électricité selon des dates d'échéance des marchés, les choix énergétiques passer les modes d'indexation les surcoûts peuvent être de 10 100 300 voire 500 % même plus dans certains endroits de même difficile d'avoir un peu de lisibilité sur les intérêts des dettes, sauf à pouvoir prévoir les taux de 2023 dont personne ne peut, à ce jour, connaître l'évolution empoté amputé de toute marge de manoeuvre, quelles perspectives reste-t-il aux collectivités contribuer au seul redressement des comptes publics, c'est oublier le rôle primordial des collectivités en matière d'investissements publics, l'investissement, qui assure la bonne tenue du site du tissu économique local et contribue à la préservation de l'emploi, c'est oublier le rôle majeur que joue les collectivités dans notre pays et les actions qu'elle porte au quotidien au plus près des populations en finançant des services publics de proximité en tout point du territoire. Madame la Ministre, les communes, les intercommunalités, les départements et les régions, n'en peuvent plus d'être si peu considérer nos collectivités locales ont besoin de vraies relations de confiance avec l'état et non pas d'une mise sous tutelle déguisée. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Pascal Savoldelli. Du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

Madame la Ministre. Ce débat sur les finances locales, intervient dans un climat Madame la Ministre de défiance. Défiance réciproque entre l'État tutélaire et les collectivités asphyxiés par la hausse de leurs coûts de fonctionnement, ça a été dit par beaucoup ici, l'énergie, les denrées alimentaires, la revalorisation du point d'indice et la hausse du coût des matériaux menace directement les projets d'investissement, la colère des maires et partout, nous la soutenons, elle se heurte à des préfets démunis les garants de la puissance publique dans les territoires sont sans solution le gouvernement invite les collectivités à la sobriété mais il est temps de prendre la mesure des responsabilités, la sobriété mais pour qui un paradoxe, un paradoxe que la relance de l'économie soit mise à mal par des mécanismes de marché déraisonner, alors que les collectivités sont les premiers investisseurs publics français. Un paradoxe entretenu par une relation financière et politique hein sincère entre l'État et la démocratie locale, les élus communaux puisque jamais les conseillers départementaux et régionaux consacrent le plus clair de leur temps à devoir quémander lors du à l'État quémander des dotations qui ne viennent pas ce phénomène s'est accrue à cause du démantèlement de la fiscalité locale, mis en oeuvre dans le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français, a marqué une première atteinte grave à l'autonomie fiscale des collectivités, la baisse des impôts dits de production en a une 2ème achevée par une suppression totale de la TVA sur les 2 prochaines années ces 2 réformes ont affaibli en même temps l'État, les collectivités locales, mais aussi et surtout la relation entre le citoyen contribuable son territoire et l'activité économique, pire encore, les ménages, les travailleurs modestes en particulier, sont ceux qui financent des baisses d'impôts qui ne payaient pas et ça c'est une vérité, Madame la Ministre, alors que 93 % des ressources de TVA assise principalement sur la consommation de tous les ménages et les entreprises de moins de 10 salariés étaient destinés à l'État en 2017, cette part a diminué pour atteindre 50 6 % en 2021 ce sont donc 41 milliards qui échappent à l'état et sans cette évaporation fiscale, le déficit du budget général serait résorbé de près d'un tiers l'État procède à un transfert de fiscalité en s'employant avec peu de succès à éponger sa dette sur le dos des collectivités territoriales, nous ne le rappelleront jamais assez, elles sont à l'équilibre toujours malgré et envers tous malgré les transferts de compétences, malgré les baisses de charges malgré la disparition de la principale part de fiscalité économique ces renoncements sont ceux de gouvernements successifs et pourtant ce sont les PME et les travailleurs qui devraient payer pour compenser cette forme de l'acheter cette accélération sans précédent de la quasi-disparition de l'autonomie fiscale des collectivités épuise un début d'encouragement dès la loi de finances rectificative pour 1982 dans laquelle l'État a institué et pris en charge des allégements de la part salaires de la base de la taxe professionnelle des allégements pour les ménages et sur la taxe professionnelle, lourd de conséquences puisque compensé par l'État, il devient alors le 1er contribuable local la démocratie tourne sur elle-même, quand le contribuable perd de vue l'utilité de ces prélèvements sociaux et fiscaux dès 2010, le Conseil des prélèvements obligatoires, relevait, je le cite une comptabilité de plus en plus compromise entre d'une part une évolution du dispositif par des aménagements à la marge successifs et sédiment et et d'autre part, les objectifs d'efficacité économique de rendement budgétaire d'équité sociale et d'accès stabilité la situation que nous connaissons est l'aboutissement d'une logique qui conduit nos collectivités dans le mur, elle ne peut faire que des perdants dès lors que les collectivités constate une décorrélation entre leurs charges et leur capacité budgétaire le fruit des compensations dépassé par l'évolution démographique par une inflation qui érodent en euros constants ces transferts et par des besoins sociaux et environnementaux nouveaux face à la hausse de prix de l'énergie et la décision du gouvernement de revaloriser seulement à 3 5 % le point d'indice, le fameux filet de sécurité votée à l'été, comporterait je l'entends ici ou là des trous dans la raquette à ce niveau là, il s'agit pas de jouer au tennis avec une raquette de ping-pong, Madame la Ministre, 430 millions d'euros, c'est son montant ne serait-ce que le point d'indice, c'est 1,14 milliards d'euros les factures énergétiques augmentent elle entre 30 et 300 % ça se selon l'Association des maires de France, les réponses de mon groupe sont claires, ambitieuse et responsable Madame la Ministre, le, dès le budget de la DGF sur l'inflation de fac sont pérennes, c'est la demande des élus, c'est la continuité des services publics sanctuarisé dans la Constitution l'autonomie fiscale des collectivités territoriales au 1er rang desquels les communes maintenir la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la CVAE et refondre un impôt économique territoriale avec une liberté tôt pour les communes, élargir les tarifs réglementés de vente de l'électricité à toutes les communes, pas qu'à certaines communes et revenir sur la suppression annoncée des tarifs réglementés du gaz madame la Ministre, les élus locaux sont responsables conclure et font face et nous leur et leurs représentants et n'en déplaise au gouvernement, vous pouvez le voir là et ben les oppositions c'est utile, madame la Ministre. Merci, cher collègue, la parole est à Jean Michel Arnaud pour l'Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, questionné les finances locales revient à s'interroger sur les relations entre l'État et les collectivités territoriales, c'est la dernière décennie, ces relations ont largement été bouleversé par les réformes successives portant sur l'organisation territoriale, la fiscalité et les concours financiers de l'État. Dans un récent rapport sur le financement des collectivités territoriales, la Cour des comptes souligne l'augmentation des ratios d'autonomie financière, alors que l'autonomie fiscale se réduit l'autonomie financière croit pour des raisons mathématiques et n'est absolument pas le témoin d'un renforcement des marges de manoeuvres financières des collectivités locales quant à l'autonomie fiscale se réduit comme peau de chagrin, a une emprise plus forte encore de l'État central sur les collectivités territoriales et notamment sur les communes, après la suppression de la taxe d'habitation ou le reversement obligatoire d'une fraction de la taxe d'aménagement des communes aux intercommunalités a été annoncée par votre gouvernement, la disparition progressive de la CVAE notre groupe Union centriste souhaite un report. De la mise en oeuvre de cette réforme afin de pouvoir porter le débat en profondeur et qu'on nous fasse pas le coup de dire qu'on porte un coup au aux entreprises, il s'agit de protéger l'autonomie fiscale des collectivités locales et protéger le lien important entre les collectivités locales et leurs entreprises, nous avons donc à faire une nouvelle fois à une fiscalité aussi par procuration téléguidé par l'exécutif national et alors que la libre administration des collectivités et toujours et encore structurellement grignoter les contraintes progresse toujours dans son rapport publié ce mois-ci la Cour des comptes, indique que l'évolution des dépenses de ces dernières 4 % des dépenses de fonctionnement 2021 s'explique en partie par l'accroissement des compétences des collectivités sous l'effet de la décentralisation, or la réalité s'avère bien plus complexe, cette tendance s'explique par une triple évolution, la multiplication des normes imposées aux collectivités locales un milliard d'euros sur le projet de loi de finances dont on va discuter, dans quelques semaines, je rappelle que l'indexation de la DGF équivaudrait à un milliard d'euros de d'euros de dépenses complémentaires, il faut effectivement comparer les choses 2ème cause l'élargissement des périmètres des intercommunalités qui a conduit, il faut le rappeler à une forte hausse des coûts mais également le rôle croissant de l'échelon local pour amortir les impacts des crises : écologique, économique et sanitaire, je pense en particulier au Covid car oui, ne l'oublions pas, mes chers collègues, nos communes, intercommunalités,

l'exécutif a également appelé récemment à la mise en place d'un énième pacte de confiance en soi, nous ne pouvons être que d'accord avec cette proposition, mais cela ne doit pas se traduire par l'instauration de contrats léonins, comme cela a été dit par une collègue précédemment, si le 1er mandat d'Emmanuel Macron fut décevant en matière de décentralisation à l'image de la décevante loi 3DS et parfois houleux concernant les relations avec les collectivités territoriales, ce pacte doit être envisagé comme un facteur d'aide à la croissance et non pas comme un outil de qu'on traite de la gestion locale, pour cela, il faut fixer des objectifs communs en laissant des libertés locales permettant à chaque territoire de les atteintes, selon les circonstances locales plus en cours, j'en appelle à la différenciation territoriale et à la confiance envers les élus, par exemple, à court terme, la révision des valeurs locatives doit prendre en compte le taux d'inflation indispensable à la sécurisation des ressources locales entre illustration : je ne veux pas que Jean Baptiste blanc l'évoquera également le financement nécessaire à la mise en oeuvre, Dusan est une variable à intégrer dans les discussions afin qu'elles soient comptabilisées dans les futurs concours financier de l'État madame la Ministre, nous allons ouvrir le débat sur le PLF, je souhaite que ce débat se fasse dans la confiance en direction des collectivités locales, mais aussi en leur assurant les moyens de pouvoir agir pour le dernier kilomètre auxquels nos concitoyens sont particulièrement sensibles, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Jean-Baptiste Blom. Pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport sur les finances publiques locales annexé au projet de loi de finances c'est un document de 208 pages riche en chiffres et en information mais en effet merci Jean Michel Arnaud quasiment rien sur la règle nouvelle qui soulève des inquiétudes considérable dans de nombreux territoires en fusion souvent celle du zéro artificialisation nette que nous appellerons Lausanne cette règle a été défini, sans les outils qui permettraient d'en assurer la mise en oeuvre, laissant les collectivités démunies face à un tel écart entre l'objectif qui leur est assignée et les moyens à leur disposition, je veux alerter le gouvernement une nouvelle fois sur cette question et relayer les inquiétudes très nombreuses non ne font par tous les élus locaux sur tous les bancs et que j'ai constaté, tout particulièrement en faisant un tour de France, un département sur 2 quasiment avec sur la mise en oeuvre du Dusan la quasi-absence du mot artificialisation dans les différents rapports du gouvernement est caractéristique de l'insuffisante réflexion du gouvernement sur la manière dont les obligations donner aux collectivités seront financés premières pistes c'est certes celle du Fonds friche il il a révélé un nombre important de dossiers qui pouvait émerger pour revitaliser les espaces délaissés et auquel il manquait seulement un équilibre économique, que devient le fond friche chez le président de la République a annoncé sa pérennisation, vous en avez parlé aussi dit ne constitue plus que un volet du Fonds d'accélération de la transition écologique ou fond Vert et son objectif est de limiter désormais à 1000 hectares de friches recyclés, parents et documents budgétaires. N'indiquent pas clairement ces ces crédits, ce n'est pas suffisant et les collectivités auront besoin d'un soutien beaucoup plus important pour mener à bien les indispensables : action de recyclage urbain, il est nécessaire, ensuite d'appuyer également sur le levier fiscal, c'est peut-être là le message principal : la fiscalité locale n'est pas adapté à la politique de sobriété foncière, on ne peut pas imposer aux communes contraintes aussi forte sur l'aménagement local sans que les communes en particulier est une incitation alors qu'les réformes successives de la fille qui été le distant de plus en plus le lien entre leurs ressources et le résultat de leur action, la commission des finances, a donc saisi le Conseil des prélèvements obligatoires, afin qu'ils fournissent des pistes sur la manière dont la fiscalité notamment locales pourrait favoriser l'atteinte de l'objectif, le CPO présentera ses résultats le 26 octobre et ces analyses pour nourrir les débats, notamment sur la loi de finances a en effet plus d'un an après la promulgation de la loi climat et résilience les lois de finance successives reste muette ou presque sur la question du financement du Zan, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit certes une adaptation mineure de la taxe d'aménagement, les collectivités pourront exonérer les constructions réalisées sur les sites qui ont fait l'objet d'une opération de dépollution, cette mesure n'est de toute évidence pas à la hauteur de l'enjeu, d'autant qu'il s'agit d'une exonération faculté. Si son coût pour les collectivités ne sera pas compensée par l'État, alors que l'objectif est la mise en oeuvre d'un d'une politique d'intérêt national, la taxe d'aménagement fait pourtant bien partie des pistes à explorer, on évoque aussi d'autres pistes telles que la taxe sur les logements vacants ou l'ancien versement pour sous-densité mais aussi des incitations directes aux particuliers, tels que le dispositif de Normandie, les dispositifs fiscaux présentent chacun des avantages mais aussi des risques de contournement ou d'effet rebond, c'est pourquoi nous aurons besoin bel et bien de cet éclairage du CPO dont les rapports sont une référence, je regrette que l'administration déjà interrogé à moultes occasions n'est pas déjà conduit cette réflexion, des propositions claires sur le financement, Dusan aurait permis d'apaiser certaines inquiétudes sur sur suscité dans les territoires Les collectivités sont en effet soumis à des injonctions contradictoires, on le sait, touchent désormais par coeur là doivent développer le logement notamment social et a tiré des activités économiques mais sur quel terrain, une enquête du cinéma et de la DC. Publié le mois dernier, montre que la pénurie de foncier d'ores et déjà une réalité pour la majorité de nos territoires, mais comment peut-on réindustrialiser la France et les collectivités ne peuvent pas accueillir des activités les collectivités consacre actuellement un travail considérable à l'élaboration de solutions et à la modification des documents d'urbanisme et dans le cadre de la mission conjointe de contrôle sur Lausanne avec la présidente Valérie Létard et les membres de la mission, nous constatons un au niveau de réflexion des élus et des acteurs locaux qui ont des propositions à vous faire madame la ministre et décret de mise en oeuvre qui ont été publiés hâtivement doit être corrigé, un autre ministre, elle a lui-même reconnu dans cet hémicycle, la nomenclature fait encore l'objet de travaux des urbanistes et un certain nombres de grands projets engagés au prévus risque de consommer beaucoup trop de foncier autorisé dans les 10 années le sujet est donc bel et bien explosif, madame la ministre, il faut adapter, on le sait tous aussi les recettes fiscales locales aux nouvelles missions des collectivités locales, bon, celle de 37 transition écologique et celle du than donc aux 3 options polaire mises sur la table par la Cour des comptes, je propose d'en rajouter une qui est celle de la climatisation sans délai du than et de la fiscalité locale merci beaucoup. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Thierry Cozic pour 4 minutes. C'est le président, madame la ministre, mes chers collègues, au gré de nos déplacements dans nos circonscriptions, une chose est certaine, pour nos élus du bloc communal, l'inquiétude est palpable. Elle les car les dépenses contraintes des mairies s'envole littéralement, cela peut vous paraître triviale, Madame la Ministre, mais il faut bien que les villes chauffe et éclaire leurs équipements publics. Sur mon territoire pour Le Mans Métropole, cela représente 4 5 millions d'euros de surcoûts rien que pour l'énergie. Il n'est pas inutile de rappeler que nos communes fournissent la nourriture des restaurants scolaires et construisent ou rénovent leur afin d'éviter d'éviter qu'ils ne tombent en décrépitude. Pourtant, ce sont précisément toutes ces dépenses liées au fonctionnement du quotidien qui sont en nette hausse à cause de l'inflation galopante des matières premières. On sait déjà que pour la seule année 2022, elles vont globalement grimpé de 15 % pour les communes. Je rappelle que chaque année les communes doivent équilibrer leur budget. C'est cette obligation d'équilibre qui oblige certains maires à se demander s'ils pourront boucler leur budget 2023 sans être contraint de fermer des services publics. Dans ce contexte que fait l'état. Clermont, pas assez. Pour une aide réellement efficiente la DGF doit faire l'objet d'une revalorisation à hauteur de l'inflation. Je défendrai cette mesure avec mon groupe lors de l'examen du prochain PLF. Ce n'est pas la maigre rallonge de 320 millions d'euros supplémentaires qui bouchera le trou dans la raquette de la facture énergétique du bloc communal. Karl, je leur rappelle, il reste toujours près de 900 millions d'euros non comblés après l'aide de l'État. Si nous en sommes à lutter bec et ongles, lors des débats budgétaires pour obtenir plus de moyens. C'est parce que vous avez placé nos collectivités dans une subjective dépendance à l'état et ce, en rognant depuis 6 ans sur leur autonomie financière. Vous avez supprimé la majeure partie des impôts dont elle percevait les recettes éprouvées moduler les taux. Par vos réformes ou siphonner de manière systémique les recettes, plaçant ainsi de fait les communes je vous pouvez perfusion de dotation que vous pouvez moduler de façon discrétionnaire. Je le dis sans ambages ce mode opératoire est insupportable pour la démocratie de proximité qui oeuvrent au quotidien au sein du bloc communal. à en croire les déclarations récentes de Bruno Lemaire, cela ne semble pas aller en s'améliorant. Interrogé sur la gestion financière des communes en difficulté. Il a déclaré en septembre dernier, je cite. Vous avez des collectivités bien géré et d'autres qui sont moins bien gérées, ces dernières ne pourront pas se prévaloir de l'aide de l'État. Cette déclaration trace les contours de vos mal nommé Pacte de confiance déjà rejetée à l'Assemblée nationale dans votre projet de loi de programmation des finances publiques, bien que celle-ci semble avoir peu de chances d'être voté, qui a rappelé loin : vous êtes aujourd'hui minoritaires. Une chose est certain. Et certaines vous êtes animé par une volonté d'entrer dans une relation transactionnelle avec les collectivités territoriales, voir même d'en personnaliser ses relations avec l'État. J'en appelle à tous les bancs de cet hémicycle, un grand débat doit être mené sur une refonte idéologique fondant la relation État, collectivités territoriales, ce débat doit sortir des contingences matérielles et budgétaires et doit être d'une ampleur supérieure. Il doit interroger notre rapport à l'impôt local et la fonction démocratique que représente la possibilité que ce dernier puisse être votée par nos élus locaux. Si rien n'est fait, alors le gouvernement accélérera encore la mise sous tutelle budgétaire des collectivités territoriales, obligeant nos collectivités à devoir à l'avenir, négocier chaque ligne budgétaire. Et cela, je le redis, n'est ni acceptable ni supportable.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'avenir des finances des collectivités locales, interpelle dans sa dimension immédiate comme dans ses perspectives à moyen terme au regard du moment présent, je voudrais évoquer tout d'abord le traitement dont elles font l'objet dans le cadre de la loi de finance en mettant un focus particulier sur le bloc communal, le gouvernement conforté par l'appréciation de la Cour des comptes vient d'évoquer leur bonne situation financière et d'ores excédents qui friserait l'insolence au sortir de la crise financière, je souhaiterais nuancer cette assertion, comment justifier la relativité de la perception, les collectivités locales ne sont pas régis par les mêmes règles de gestion que l'État et c'est tant mieux, bordé par la règle d'or, elles ne peuvent utiliser la dette à des fins de fonctionnement et doivent gérer leurs finances par la pratique de mise en réserve et d'une gestion prévisionnelle pluri annuelle, il est donc curieux que l'État observe une lecture de leur situation à l'aune de règles qui ne sont pas les leurs, alors qu'il devrait plutôt songer à s'en inspirer dans leurs pratiques vertueuses et s'obliger à ce qu'il entend imposer aux autres, je veux évoquer par là le contrat dit de confiance je je rappellerai à cet égard que notre République leur garantit pourtant la libre administration au terme de l'article tout ça 72 de la Constitution, ainsi que l'a indiqué Roger Karoutchi tout à l'heure durant le quart de siècle écoulé les collectivités ont consenti des efforts financiers sans précédent, il m'apparaît de bonne justice de les évoquer, nonobstant le fait que des fonds qu'elles ont ainsi épargné entre positivement dans le solde maastrichtien pour le plus grand bénéfice de notre pays afin de permettre aux pays justement de conserver une trajectoire acceptable, elles ont ainsi renoncé progressivement la taxe professionnelle, comme à la taxe d'habitation en contrepartie de dotation moins dynamique, elles ont subi durant 4 ans, la contribution au redressement des finances publiques qui a amputé drame drastiquement leur DGF pour l'avoir ensuite figé et contributrice à la péréquation verticale, de sorte que si on avait pas paramétrer pour elle une loi de programmation spécifique sur cette période, on constaterait que c'était indifférent, celle de lors de 50 milliards qu'elles ont consenti à la nation aussi si malgré l'inflation et la crise énergétique nous ne revendiqueront pas pour elle, l'indexation d'une DGF en état de gagner de déliquescence avancée hé admettront le principe d'un filet de sécurité et de dotation ciblés sur les plus vulnérables, nous voulons dire haut et fort que le compte n'y a toujours pas et que c'est à bon droit que les collectivités n'admettent pas d'être fustigés par un État impécunieux pour ce qui concerne leur avenir à moyen terme, il n'est rien de dire qu'elle ne dispose d'aucune visibilité dans un système financier désormais menacée d'obsolescence, je veux m'en expliquer la suppression de la taxe d'habitation et la perspective de sa de la CVAE ont totalement achevé la désarticulation du Cadre sous-tendu par des indices, désormais privé de sens et elle ne dispose plus des perspectives nécessaires pour gérer leur dynamique et doivent s'en remettre à la diligence de la DGCL pour la mise en oeuvre d'une péréquation au fil de l'eau ainsi que vient de le confirmer le rapport établi par la Cour des comptes à la demande notre commission des finances, le système est devenu complexe et à bout de souffle les collectivités dans quelles sont désormais à la merci de la suppression ou de l'affectation nouvelle d'un impôt décidé d'en haut et ne dispose plus d'aucune visibilité dans un monde devenu qui plus est aléatoire et complexe et alors qu'elles sont aux prises avec un système financier devenu incohérent, nous nous sommes attelés au Sénat résoudre cette équation, mais elle, elle est devenue un seul face au scénariste aussi plurielle que ceux évoqués par la Cour dans ses travaux, faute d'une boussole pour ce faire, il faudrait que l'État mette fin au démantèlement erratique des ressources des collectivités et initie les bases d'une réforme dans un dialogue construit avec elle est dotée d'une nouvelle gouvernance, les collectivités sont un acteur majeur de notre République au plan démocratique et sociétal et réalise 70 % de l'investissement public, elle ne mérite, madame le ministre : quand allez-vous mettre cet ouvrage sur le métier. Merci, cher collègue, vous étiez donc le dernier intervenant des groupes. Madame la ministre, vous avez un temps de réponse à l'ensemble des interventions ton de réponse assez limité puisque la règle c'est cinq minutes vous pouvez dépasser un peu parce que vous avez choisi de pas intervenir au fil du débat, mais allez-y, vous avez la parole. Oui, vous pouvez venir là. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vais m'efforcer dans le temps qui m'est dévolu, de répondre à la majorité de vos interventions, je commencerai par répondre à certains points précis qui ont été abordés sur les mesures du PLF 2023 avant d'répondent plus globalement sur les enjeux qui ont été soulevées sur la nécessité d'une réforme de la fiscalité locale et sur la nécessité d'un nouvel élan décentralisation dans notre pays pour les questions les plus techniques qui ont été évoqués, je reviendrai vers chacun d'entre vous pour vous apporter une réponse circonstanciée, monsieur le sénateur pu sur la CVAE comme j'ai pu le dire dans mon intervention liminaire sa suppression n'entraînera pas, je le redis, n'entraînera pas une baisse des ressources des collectivités territoriales, bien au contraire sa compensation intégrale par l'attribution d'une nouvelle fraction de TVA et de sa dynamique garantira aux collectivités une meilleure prévisibilité et une meilleure visibilité sur leurs recettes, alors que la CVAE était très volatile, ensuite sur la compensation à l'écoute des élus, nous avons justement souhaité introduire un mécanisme de moyenne pour lisser la volatilité de la CVAE d'une année à l'autre en intégrant l'année 2023 dans le calcul. La compensation l'année prochaine, pose correspondra aux sommes que l'État aurait dû verser aux collectivités en 2000 23 au titre de la CVAE, rien ne sera conservée par l'État, la dynamique de cette compensation sera territorialisé je le redis, un territoire accueillant plus d'activité recevra plus de TVA, monsieur le sénateur Cozic sur la question de la non-indexation de la DGF sur l'inflation, je voudrais souligner tout d'abord que le choix de ne pas l'indexer la DGF sur l'inflation ne date pas d'hier ne date pas d'aujourd'hui, taux, mais des années 2010 pour autant pour autant notre gouvernement a pris la décision inédite depuis 13 ans, d'augmenter la DGF de 320 millions d'euros, je rappellerai qu'entre 2008 et 2014, c'est les dotations des collectivités avait subi une baisse de plus de 11 milliards d'euros, par ailleurs, nous avons aussi fait le choix d'une action ciblée avec un filet de sécurité et un bouclier tarifaire ou encore avec le fonds d'urgence pour les communes en difficulté financière, cela nous permet de sorte de soutenir en priorité ceux qui en ont le plus besoin, quand, comme vous le savez, les situations de chaque collectivité sont extrêmement diverses, mesdames et messieurs les sénateurs, d'une manière plus générale, je pense que les interventions des sénateurs gainé Rambo ont permis d'offrir non pas une synthèse exhaustive mais en tout cas l'ensemble de l'une synthèse de l'ensemble de vos doutes de vos interrogations qui repose sur le même constat que nous partageons tous en réalité notre modèle des finances locales est aujourd'hui complexe et marquée par une longue sédimentation compte accentuer les réorganisations successives du partage des compétences entre les différentes strates, des collectivités territoriales, une situation qui parfois peut donner l'impression d'affecter les principes cardinaux qui préside aux finances locales notamment l'autonomie des collectivités territoriales, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, dont votre chambre a eu l'heureuse initiative, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit là d'une impression que d'une réalité l'autonomie financière telle que mesurée par les ratios définis en 2004 progressent, c'est la part d'attribution croissante de la fiscalité nationale au sein des ressources propres des collectivités qui nourrit chez les élus, le sentiment d'une perte de maîtrise d'une déconnexion de leurs ressources avec les réalités du territoire, je pense que le président de la République a été très clair dans son discours prononcé en Mayenne, le 20 octobre sur sa volonté de lancer le nouveau chapitre de décentralisation dans notre pays a besoin je crois en effet que notre modèle est à repenser, c'est-à-dire à remettre à plat à simplifier, pour qu'il fasse nouveau sens pour chacun, pour les élus locaux comme pour nos concitoyens, il faut repenser notre système pour que les responsabilités accompagne à chaque niveau, le pouvoir normatif et les financements, alors bien sûr, cela impliquera nécessairement des choix politiques forts, le rapport de la Cour des comptes, le souligne des choix que notre gouvernement est prêt à faire, mais cette refonte de notre système de décentralisation ne peut être conduit et le rapport de la Cour des comptes, le souligne également qu'en étroite concertation avec l'ensemble des parties concernées avec les collectivités territoriales, avec les et avec bien sûr le Parlement avec vous afin de parvenir à un consensus pour l'intérêt général de notre pays aussi, je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur le détail du scénario envisagé par la Cour des comptes, il s'agit d'un travail prospectif particulièrement précieux qui alimentera sans aucun doute le grand chantier que nous souhaitons mener à cet égard, je vous remercie également pour vos interventions qui nourrissent ma réflexion personnelle sur ce sujet, mais notre démarche de coconstruction ne serait pas véritablement sincère, vous en conviendrez, si nous cherchions en amont à déterminer le débat par des positions arrêtées, nous avons bien sûr un objectif une boussole des convictions qui nous guideront dans nos échanges à venir, mais ce n'est en aucun cas un schéma préconçu puisque cet ensemble que nous construirons le nouveau modèle déconcentrée de notre pays, monsieur le sénateur, qui dans votre intervention, vous mettez en garde contre les promesses illusoires et je suis d'accord avec vous et je citerai Jean-Pierre Raffarin, qui n'a pas quitté c'est bon depuis si longtemps, la politique ne peut plus promettre des lendemains qui chantent et repousser toujours la résolution des problèmes du quotidien, le nouveau chapitre de décentralisation que nous souhaitons ouvrir n'est pas le retour d'une vieille antienne : c'est la réponse nécessaire aux limites de notre système, cette refonte que nous souhaitons construire avec vous impose pour tous pour l'État mais aussi pour les collectivités de jouer le jeu de cette remise à plat, qui remettra nécessairement en cause de nombreuses situations établies, je vous remercie pour votre attention. Merci madame la ministre, et pour conclure le débat, la parole est maintenant à Christine Lavarde, vice-présidente de la commission des finances. Merci monsieur le Président, alors je suis certaine que le rapporteur général à qui il aurait appartenu de faire cette conclusion aurait fait remarquer avec malice au gouvernement qui doit avoir un problème de dictionnaire parce qu'après avoir expérimenté une nouvelle définition du dialogue, nous venons de vire ce soir une nouvelle acceptation du mot débat nous aurions je pense certainement souhaité quelque chose de plus interactifs tels que c'était l'esprit en tout cas de la réforme qui avait été prévu par la loi, ensuite, Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire qu'à certains moments, vous avez fait une sorte de réécriture de l'histoire, vous avez même persévéré pour ce qui consiste au filet de sécurité ce filet de sécurité, il n'a pas été voulue par le gouvernement, il a été imposé par les députés et ensuite complété par les sénateurs, au moment du projet de loi de finances rectificative donc je je voudrais que ceci soit bien rappelée par ailleurs également pour ce qui concerne l'indexation des valeurs locatives professionnel mais vous ne faites pas un cadeau aux collectivités, vous ne fait qu'appliquer le droit depuis plusieurs années, les valeurs locatives évoluent comme l'inflation constatée à l'indice du mois de novembre donc aujourd'hui vous ont de fait juste que ce qui est prévu par la loi, plusieurs intervenants ici ont rappelé et notamment par exemple Pascal Salvodelli des erreurs de votre, de la majorité à laquelle vous appartenez désormais notamment le lien qui s'est complètement distendue entre les usagers des services publics locaux et le coup de fourniture de ces services publics locaux alors nous ici, nous n'avons pas changé puisque je me rappelle avec émotion, c'était l'objet de ma première question d'actualité dans ce gouvernement, en octobre 2017, donc ça fait 5 ans que nous constatons ces égarements et dans lesquels vous semblez vouloir continuer avec la suppression encore annoncé de la CVAE alors plusieurs intervenants l'ont demandé, ici, et notamment Roger Karoutchi nous avons besoin, les collectivités ont besoin d'une certaine visibilité à moyen long terme, pour pouvoir mener des projets pour pouvoir s'engager cette visibilité pourtant l'ancien gouvernement nous l'avait annoncé, puisque je me souviens encore que dans deux lors d'audition du ministre à la commission des finances canton demandé par exemple l'affectation d'une partie des recettes de la TICPE aux collectivités locales pour venir financer les dépenses de transition écologique, on ne répondez : c'est pas le bon moment, attendez la loi de financement des collectivités locales, alors cette loi, elle n'est jamais arrivé plusieurs ici viennent encore de vous la réclamez ce soir alors Madame la Ministre, je sais que vous ne pouvez pas être insensible au courage de la vérité, que les sénateurs ont eu ici ce soir, les différents orateurs ont ex qui c'est des pistes d'évolution pour les textes budgétaires à venir, alors le rapporteur général qui a suivi tout ce débat, puis je lui vous fait passer un message, il me fait dire que si vous savez écouter la chambre haute, alors tout devient possible. Mes chers collègues, je je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 22 pour l'examen de la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, la séance est suspendue.

Merci